La séance est ouverte.-- Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué. Nous n'avons pas reçu d'observation. Il y en a-t-il en séance.-- Je n'en vois point le procès verbal est donc adopté sur les réserves d'usage.-- Notre jour appelle les questions d'actualité au gouvernement mais auparavant je reformule. Pour chacune et chacun d'entre vous. Les meilleurs voeux pour cette année qui a maintenant commencé et nous aurons qu'à l'occasion de revoir la semaine prochaine pour les formuler plus plus d'Éric directement et spécifiquement. Je vous rappelle que notre séance et retransmise en Direct sur Public Sénat sur notre site internet. Chacun sera attentif. Au respect qu'il s'agisse du respect des uns et des autres ou du respect du temps de parole. Mais je voudrais saluer la présence de notre nouvelle collègue madame Monique Del Fabbro. Sénatrice de la Meurthe-et-Moselle qui remplace Philippe. Dagmar. Je lui souhaite la bienvenue. Je vais

Jean-Claude Requier pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Monsieur le président vous avez la parole.-- Merci monsieur le président, ma question s'adresse à Madame, la Première ministre. Avec la réforme des retraites. Il y a le quoi faire sauter plusieurs gouvernements. Affirmé Michel Rocard ancien 1er ministre de François Mitterrand. C'est donc avec courage madame, la Première ministre et que vous vous attaquez à cette réforme. Vous avez au cours des dernières semaines beaucoup consulté vont politique et bien entendu les syndicats comme président du groupe et RDSE, vous m'avez reçu à l'hôtel Matignon avec mon collègue Henri Cabanel en prennent à 10 minutes du centre-est Nous en séparent de nos préoccupations et nos interrogations et au cours d'une discussion sera jus ouverte. Vous avez donné des précisions sur la pénibilité et les joueurs professionnels. La question des carrières longues. L'emploi des seniors. L'avenir des régimes spéciaux et l'augmentation des pensions minimales vous avez dévoilé hier votre projet au sein duquel l'âge légal de départ à la retraite. Sera finalement fixé à 64 ans en 2030 au au lieu des 65 ans envisagés sur ce point qui cristallise de nombreux mais mécontentement. Pourquoi ne pas maintenir l'âge légal à 62 ans et tenir compte uniquement des trimestres cotisés qui déterminerait le montant des pensions une modulation de la durée de cotisation. Selon les situations. Le CNT par le système le plus équitable et à une compromis dans la tradition. Mais sa radicalité. Pour vous répondent. La parole est à madame la Première ministre. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, Monsieur le Président requiers je voudrais tout d'abord présenter mes meilleurs voeux à toutes les sénatrices et sénateurs à leurs équipes. Et au service du Sénat. Monsieur le le président Ruquier le système de retraite par répartition est au coeur de notre modèle social. Les Français ils sont profondément attachés. Nous l'avons évoqué à plusieurs reprises. Je sais que vous-même et votre groupe l'aussi. Je partage cet attachement et avec mon gouvernement. Nous sommes résolus à agir pour préserver notre système de retraite par répartition. Mais aujourd'hui, chacun le sait le nombre de personnes qui travaillent par rapport au nombre de retraités diminuent menaçant notre modèle. Aussi, après des mois de concertation. J'ai annoncé hier. Notre projet pour garantir l'avenir de nos retraites. Un projet d'équilibre d'abord. Nous refusons d'augmenter les impôts ou de baisser les pensions. Le seul chemin possible, c'est donc de travailler progressivement plus longtemps. Comme vous l'avez dit, nous porterons l'âge légal de départ à 64 ans en 2030 et nous allons également accélérer la mise en place de la réforme Touraine pour atteindre 43 années de cotisations en 2027. Comme vous le voyez cela rejoint les grandes lignes du dispositif voté par le Sénat. Depuis plusieurs années. Quant à l'âge d'annulation de la décote. Il est et restera à 67 ans. C'est important pour les nombreuses femmes qui doivent aller jusqu'à cet âge pour ne pas avoir de décote sur leur pension. Grâce à cela notre système sera à l'équilibre en 2030. Alors je suis bien consciente de ce que cela signifie pour beaucoup de nos compatriotes. C'est pourquoi nous avons construit un projet de justice. Celles et ceux qui ont commencé à travailler plus tôt pourront partir plus tôt. Les carrières des femmes souvent incomplètes ou haché seront mieux pris en compte la pénibilité des métiers sera mieux reconnue, nous continuerons à tenir compte des plus fragiles, un départ à 62 ans sera toujours possible pour les personnes en invalidité en incapacité ou en inaptitude. Au total, 4 Français sur 10, souvent les plus fragiles, les plus modestes. Celles et ceux qui ont des métiers difficiles pourront partir avant 64 ans. J'ajoute que la justice c'est aussi fermé la plupart des régimes spéciaux car le même métier doit donner la même retraite. Et ce n'est pas tout notre projet sera porteur de progrès social. Conformément à l'engagement du président de la République. Nous allons augmenter la retraite minimale pour une carrière complète au niveau du SMIC à 85% du SMIC, soit une hausse de 100 euros par mois et ce dès cette année. Nous avons aussi entendu l'appel de plusieurs groupes politiques et d'organisations syndicales et patronales et je vous confirme que l'augmentation de la retraite minimale concernera bien les retraités actuels. Au total près de 2 millions de Français verront leur pension revalorisée dès cette année, ce sont d'abord des femmes, ce sont d'abord des commerçants et des artisans qui ont travaillé toute leur vie, c'est un progrès social majeur. Enfin, nous voulons rendre aux salariés proches de la retraite toute leur place en entreprise. Avec davantage de transparence sur les politiques des employeurs avec l'assouplissement de la retraite progressive. Et avec un cumul emploi-retraite plus avantageux. Monsieur le Président Ruquier aujourd'hui mon ambition avec mon gouvernement avec tous ceux qui veulent préserver notre système de retraite par répartition c'est de convaincre autour de ce projet c'est de chercher à l'améliorer avec le Parlement et je sais que le Sénat il prendra toute sa part c'est de construire ensemble un système juste équilibré et porteur de progrès social. Je vous remercie. Merci madame, la Première midi sur le président qui. Merci la vraie ministre. Au Sénat, il n'y aura pas la. Trois, il n'y aura sûrement pas les questions préalables dans le débat ira à son terme et nous il y a pour nous l'autre groupe. Il prendra toute sa part. Et permettez-moi un petit rappel historique. Au début du siècle au début du règne de Louis XVI. Turgot, qui a été appelé comme contrôleur général des finances. Parce qu'il du déficit. Il a proposé des mesures audacieuses ambitieuses certaines suppression de privilèges et il a eu cette formule la réforme plutôt que la révolution. Quelques années après, il y a pas eu de réforme. Quelques années après, il y a eu la révolution. Eh bien il a j'espère que cette réforme de des retraites n'amènera pas la révolution. La parole émeutes en de notre collègue Raymond pour ses manches pour le groupe écologiste solidarité et territoires. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, vous avez présenté hier une réforme des retraites qui allonge de nouveau de 2 ans l'âge de départ à la retraite. Vous avez balayé nos solutions alternatives pour combler un déficit que vous dramatisez sciemment et qu'il n'aurait jamais dû être un problème si le fonds de réserve des retraites n'avait pas été siphonnés mais alimenté comme prévu. Vous vous gardez de présenter le bilan de la contre-, réforme de 2000 disques, vous vous apprêtez à copier soit la baisse tendancielle du montant des pensions et de la durée de vie à la retraite selon l'adresse en 2016 la réforme de 2010 avaient déjà fait presque un an de durée de retraite à la génération 80 en cumulant toutes les réformes depuis 2010 plusieurs générations perdront jusqu'à 20 mois de durée de la retraite. Non seulement ces réformes ont affecté au travail. La grande partie des gains d'espérance de vie. Mais votre réforme va empiéter sur les années de vie à la retraite en bonne santé et il n'y a rien de plus inégalitaire quand selon l'INED, l'écart de vie en bonne santé de 10 ans entre catégories socioprofessionnelles votre réforme s'attaque au droit au repos de tous les travailleurs mais cogne plus dur sur les classes populaires, les ouvriers, les employés comme va allonger le sas de précarité des ni en emploi, ni en retraite pour une partie au chômage ou au RSA dont vous réduisez dans le même temps les droits. L'attaque contre le monde du travail, la protection sociale et frontale et systémique et des voix ce que recouvre le credo du travailler plus pour perdre sa vie à la gagner et détruire l'habitabilité de notre retraite pensez-vous qu'après une crise sanitaire qui a interrogé la place et le sens du travail à l'heure des urgences, il est responsable d'imposer une réplique de la contre-, réforme inégalitaire de 2010 et ce, contre une très large majorité des Français et des représentants syndicaux. Pour me répondre. La parole est au ministre du Travail. Mais non. De l'insertion monsieur Olivier Dussopt. J'avais la parole. Merci, merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs. Madame la sénatrice, forcément. Finalement, au travers de votre question, vous nous dites et ce qu'il faut faire une réforme des retraites. La réponse est oui. Elle est, oui elle est positive pour 3 raisons, trois raisons que vous retrouverez dans le rapport du conseil d'orientation des retraites. Que dit ce rapport, ce rapport dit d'abord que le système est déficitaire. Déficitaire dès 2023 avec une perte d'un milliard 8 déficitaire en 2027 avec un déficit de 12,5 milliards d'euros déficitaire en 2030, avec presque 15 milliards d'euros, puis 20 milliards d'euros par an en 2035, 25 milliards d'euros en 2040 et l'enjeu de cette réforme, c'est aussi de préserver un système de répartition de le préserver avec d'autant plus d'attention que les chiffres que je donne à l'instant, ce sont des chiffres qui sont prévues par le conseil d'orientation des retraites. Dans l'hypothèse où nous aurions atteint le plein emploi, c'est-à-dire une hypothèse à laquelle nous participons que nous souhaitons mais qui reste une hypothèse optimiste et si le plein emploi n'était pas au rendez-vous les chips serait encore plus dégradée et le système serait encore plus en danger. Du premier acte de solidarité, c'est de permettre aux générations qui viennent de conserver un système de répartition et de le faire sans être étouffé par la dette ni assommés par les impôts. La 2ème. Raison pour laquelle il faut faire cette réforme, c'est parce que si nous ne la faisons pas là aussi c'est le rapport du COR qui le dit. Le niveau de vie des retraités va baisser et je ne suis pas sûr. Madame la sénatrice que vous souhaitiez retrouver la situation des années 70 quand les retraités étaient les pauvres du pays alors même que notre système par répartition a permis aux retraités justement d'avoir un niveau de vie qui soit identique à celui. De l'ensemble des Français. Et puis il y a une 3ème raison c'est une raison démographique que la chef du gouvernement a exposé. À la fin des années 70, nous étions trois actif à cotiser pour un retraité, aujourd'hui, nous sommes un tout petit peu plus de 1,5 actifs pour un retraité. C'est la démonstration que ça ne tient pas puisque ça ne tient pas, il faut réparer, réparer avec des mesures d'accompagnement sur la sur la pénibilité sur les carrières longues pour protéger les plus fragiles réparer dans le débat et je le dis devant le Sénat parce que la responsable de votre parti. La responsable des Verts au niveau national a appelé de ses voeux que l'Assemblée nationale se transformer ZAD. Ça n'est pas notre conception de la démocratie et je souhaite comment ici nous puissions mener un débat apaisé. Quelques secondes. Que oui, Monsieur le Ministre, la réponse sera donné le 19 par la mobilisation des Français auprès des organisations syndicales et des partis de la gauche et écologistes. La parole est à notre collègue Franck Menonville pour le groupe les indépendants République et Territoires, mon cher collègue. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. En raison de hausse exorbitante des coûts de l'énergie dans mon département de la Meuse, ce sont déjà 7 boulangers qui ont cessé leur activité. Pour faire face à l'augmentation des prix des matières premières, certains boulangers ont déjà dû réévaluer leurs prix de vente. Une nouvelle augmentation tarifaire seraient aujourd'hui inenvisageable. Mais pour grand nombre d'entre eux, la situation est aujourd'hui intenable. Face à cela, différentes mesures à destination des boulangers ont été annoncés le 4 janvier dernier. Je ne reviendrai pas sur les conditions d'éligibilité néanmoins concernant le bouclier tarifaire 80% des boulangeries ne peuvent aujourd'hui prétendre car elle dépasse le seuil de 36 kilowatts avec utilisation des fours des chambres froides des pétrin et des vitrines. Certes l'amortisseur électricité devrait pouvoir s'activer mais nos boulangers nous alertent régulièrement sur le prix de 180 euros le mégawatt, qui selon eux restent trop pénalisant et encore pas assez protecteur. Les conditions d'éligibilité ne sont pas suffisamment adaptée aux difficultés rencontrées par la profession et les démarches et les démarches sont perçus comme trop complexe. Pour que les dispositifs soient accessibles et rapidement applicables. Il faut s'appuyer. Sur les les les le le réseau local et notamment faciliter la compréhension de ces dispositifs. Les accompagnements annoncées vont certes dans le bon sens mais force est de constater qu'ils sont insuffisants au regard de l'intensité des difficultés de la profession, monsieur le ministre, est-ce que le gouvernement entend proposer un dispositif plus protecteur pour les TPE, les plus impactés. important et urgent d'envisager un déplafonnement de la puissance de 36 kilowatts pour étendre ainsi le bénéfice du bouclier tarifaire. Ce serait là une mesure simple et bien comprise.

Vous avez aujourd'hui à peu près de 1 million de très petites entreprises, moins de 10 salariés. Moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires.-- Vous l'avez rappelé 1,5 millions d'entre elles sont protégées par des tarifs régulés parce qu'elles ont une puissance électrique inférieure à 36 kilovoltampères, donc elles, elles sont totalement couverte par le bouclier tarifaire, elles n'auront pas d'augmentation de leur facture d'électricité de plus de 15%. Je rappelle qu'il n'y a aucun autre pays européen qui propose cela à c'est très petites entreprises. entreprises. 600.000. Très petites entreprises, alors on aurait pu effectivement étendant le TRV à ces 600.000 entreprises. Le coup était de 3 milliards d'euros. Et j'aurais certainement bénéficier à quelques milliers de boulanger. Mais il serait il. Des centaines de milliers d'autres entreprises qui n'en ont pas nécessairement besoin alors qu'il faut aussi protéger les PME aussi protéger les entreprises de taille intermédiaire industrielles exposé à la concurrence internationale. C'est pour ça qu'avec la Première ministre ont fait un choix différent mais très protecteur. Nous avons obtenu des fournisseurs que la facture moyenne ne puissent pas dépasser les 280 euros le mégawattheure. En moyenne sur l'année 2023. Je rappelle que beaucoup de boulanger. Vous avez raison de le souligner, sont pris en tenaille entre l'augmentation du prix de la farine, l'augmentation du prix des matières premières. Et des coûts de l'électricité qui pouvait atteindre 700 800.000 euros le mégawattheure, là ils ont la garantie que leur facture sera plafonné à 280 euros en moyenne le mégawattheure. C'est une protection majeure est nécessaire pour les boulangers. Si certains ont encore des difficultés, ils peuvent bénéficier du report de charges de l'amortisseur sur l'électricité et du guichet sur lequel pourront venir réclamer des subventions, s'ils en ont encore besoin qui peuvent amortir la facture de 40% très sincèrement que nous avons pris avec Élisabeth Borne toutes les dispositions nécessaires pour protéger une profession à laquelle nous sommes profondément attachés, les boulangers et protégeant priorité toutes les très petites entreprises de France bien entendu, ma porte est celle d'Olivia Grégoire reste toujours ouverte à la discussion. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Jean-François Husson, pour le groupe Les Républicains. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre, Bruno Lemaire, finalement, acteurs économiques acte de Monsieur le Ministre j'entends votre brevet d'autosatisfaction mais il y a quelques instants encore, j'avais. Un chef d'entreprise au téléphone qui regroupe les demandes de nombreux acteurs économiques, les boulangers, ça a été dit, vous l'avez dit, il en manque et c'est grave mais également l'ensemble des acteurs économiques qui aujourd'hui ne comprennent pas l'absence de vision stratégique du gouvernement pour venir en aide et en soutien. Quand vous parlez de 280 euros. C'est, grosso modo, jusqu'à 350% d'augmentation par rapport à des prix récent. Quand et comment les acteurs économiques peuvent-t-il tous subir cette concurrence le risque et vous le savez, c'est d'avoir un mur de cessation d'activité, voire de faillite Bpifrance dit près de 70.000 euros. Monsieur le Ministre, considérez-vous aujourd'hui avoir pris toutes les mesures pour répondre aux besoins de l'ensemble des entreprises qui font vivre la maison France. maison France. La parole est au ministre de l'Économie et des Finances Bruno Lemaire.-- Monsieur le. Rapporteur général, on n'est jamais certain d'avoir pris toutes les mesures.-- C'est pas la première crise que j'ai à gérer. Nous avons géré avec le gouvernement, la crise du Covid. Avec votre soutien, votre compréhension. Nous avons mis en place un quoi qu'il en coûte, parce que la richesse français s'était effondré la production s'était effondré et il y avait un risque de faillite par vagues successives et d'une explosion du chômage de masse. Et on m'avait averti de ce risque là, il ne s'est rien passé.-- Nous avons protégé le monde économique. Protéger les entrepreneurs protéger les entreprises éviter un chômage de masse. Nous avons géré avec efficacité la crise du Covid. Face à la crise de l'inflation le quoi qu'il en coûte n'est pas la bonne solution. Le quoi qu'il en coûte c'est jeter de l'essence sur l'incendie et ne pas se débarrasser de l'inflation. Vous nous reprochez de pas avoir de vision stratégique. Je pense que nous avons une vision stratégique qui est de faire baisser l'inflation dans le courant de l'année 2023 et ne rien faire qui puisse prolonger l'inflation dans les années qui viennent le quoi qu'il en coûte aujourd'hui sans doute que ça servirait immédiatement certaines entreprises. Mais l'ensemble de la population française se verraient exposés au maintien d'un niveau très élevé d'inflation avec tous les dommages que ça représente pour les entreprises et tous les dommages que ça représente pour les ménages. Donc nous avons choisi une voie qui est plus difficile mais j'ai toujours considéré que la voie difficile étaient en général la meilleure. Celle qui consiste à cibler les entreprises qui en ont le plus besoin, les très petites entreprises a été signé et tout à l'heure et qui n'ont pas les reins suffisamment solides pour réagir. Elles ont des tarifs préférentiels. Elles ont une protection, elles ont un guichet qui était maintenu au 1er janvier, elles ont le report des charges elles ont dans chaque département un numéro d'appel un 06 d'un conseiller qui peut les aider. Elles ont la possibilité d'étaler les prêts garantis si elle le souhaite. Reste les PME avec lesquels nous sommes en discussion. Nous voulons protéger notre outil industriel protéger nos PME protéger nos entreprises de taille intermédiaire qui elles sont exposées à la concurrence internationale et ne peuvent pas augmenter leurs prix parce que sinon elles perdront leur marché, là aussi, nous ferons le nécessaire. Notre vision stratégique c'est protection immédiate de ceux qui en ont besoin. Faire baisser l'inflation sur le moyen terme pour se débarrasser de cette plaie et sur le long terme continuer une politique de l'offre qui favorise la compétitivité de nos entreprises. Je sais que vous nous rejoindre et sur ce point là. Monsieur le Ministre. Vous avez. Il y a peu expliqué que vous souhaitiez parler aux fournisseurs d'énergie. Bah, écoutez, vous en avez un qui est tout trouvé sous la main et que vous contrôler entièrement, il s'appelle EDF. Donc, mettez-vous au travail et rapidement pour apporter des solutions. Je rappelle, je rappelle que pour EDF, nous payons ici les choix funestes menée depuis 10 ans pour arrêter la production d'électricité nucléaire on en payent très chèrement le prix. Monsieur le Ministre.-- Je l'ai dit, nous avons besoin d'avoir une vision stratégique. En domaine énergétique pour travailler sur les énergies renouvelables pour travailler sur l'autonomie énergétique et pour travailler sur notre souveraineté énergétique, notamment dans le renouvelable et dans le nucléaire. Tout ça doit en plus améliorer le solde de notre balance commerciale et enfin Monsieur le Ministre TPE PME ETI, grandes entreprises, les entreprises de France ont besoin d'un soutien adapté mais encore faut-il travailler en constance avec ses représentants notre prise il compte sur vous. La France a besoin d'un État fort à ses côtés. Merci. La parole est à notre collègue Catherine Morin-Desailly pour le groupe de l'Union centriste. Merci monsieur le président, mes chers collègues comme mes 2 prédécesseurs, ma question s'adresse au ministre de l'Économie et porte sur la situation des boulangers en en France. Il y a quelques semaines, je voudrais attirer votre attention sur ce fait était annoncé l'inscription de la baguette française au Patrimoine immatériel de l'UNESCO mettant en valeur la filière de la boulangerie ses traditions et ses savoir-faire serait-elle alors menacé. En effet dans nos départements en ce moment les maires. Nous alerte sur les graves difficultés rencontrées par les boulangers qui doivent faire face et ça l'a été rappelé. À une explosion de leurs factures d'électricité. Alors Monsieur le Ministre, vous avez bien exposé les mesures annoncées par le gouvernement le mois dernier la possibilité de recourir à l'amortisseur électricité le report du paiement des impôts et des cotisations sociales l'étalement du paiement des factures d'énergie. Les fournisseurs, vous l'avez aussi rappelé ont d'ailleurs accepté que l'ensemble des TPE et ceux qui ont signé un contrat d'électricité. Au cours du second semestre 2022 ne paie plus de papa. Plus de 280 euros par mégawattheure. En moyenne sur l'année 2023. Alors tout cela est, est très bien, mais les dispositifs sont complexes, a été rappelé, et surtout ça va se mettre en oeuvre qu'à la fin du mois. Or 13 immédiatement les boulangers nous alertent sur leurs problèmes, ils font immédiatement face à une hausse considérable du coût des matières premières c'est plus de 30% plus de 30% répercuter sur leurs charges et ils peuvent pas augmenter perpétuellement les prix sous peine de voir leur clientèle. Baisser donc l'heure est grave, Monsieur le Ministre et nombre de boulangers sont au bord de la faillite du dépôt de de bilan donc c'est dramatique pour eux mais ça l'est aussi pour nos territoires, mes chers collègues, la boulangerie le commerce le plus élémentaire en zone rurale. Celui qui maintient la vie dans dans nos villages, que comptez-vous faire Monsieur le Ministre, particulièrement peut être en lien avec les grandes régions qui disposent de la compétence économique et qui oeuvre aussi à trouver des solutions. Je vous remercie.-- Pour vous. Parole est au ministres. De l'économie et des finances monsieur Lemaire.--

Qui me demande de me mettre au travail. Je vous rassure, je suis au travail et je n'ai pas un très grand goût pour la fainéantise. Madame Morin-Desailly pour être tout à fait concret et répondre à nos amis boulanger.-- Aujourd'hui, la seule chose que nous demandons à nos amis boulanger c'est d'aller choix sur leur site dédié, soit sur impôts Point gouv Point FR de se déclarer comme très petites entreprises puisqu'il se trouve que EDF, je reste sur le si monsieur Jean-François Husson, je reçois EDF au minimum toutes les semaines avec Agnès Pannier-Runacher et avec Olivia Grégoire. Donc nous sommes en contact très régulier, il faut qu'il se déclare comme très petites entreprises, parce que les fournisseurs d'énergie ne le savent pas et il faut qu'il déclare puisque nous venons de modifier le formulaire qu'ils souhaitent bénéficier du tarif garanti à 280 euros en moyenne. Donc tous les contrats qu'ils ont pu signer à 500 600.000 euros le mégawattheure. Ils sont résiliés et automatiquement, ils auront droit ce tarif à 280 euros le mégawattheure. C'est une protection massive et pour ceux pour lesquels ça ne suffit pas, je le rappelle, guichet unique amortisseurs qui réduit de 20% l'augmentation de la facture et décalage du paiement des charges parce que c'est vraiment nécessaire. Donc je crois que le maximum a été fait. Reste maintenant et je vais en dire un mot. Les petites et moyennes entreprises des entreprises de taille intermédiaire qui elles sont confrontées à la même augmentation des tarifs et qui sont exposés à la concurrence internationale. Je prends juste un exemple très concret, j'étais à Charleville-Mézières il y a quelques jours, j'ai vu une entreprise industrielle qui fait des plaques en aluminium pour refroidir les véhicules électriques. Hé bien et son acheteur qui était en l'occurrence un constructeur automobile allemand lui dit vous ne pouvez pas augmenter les prix, sinon je me fournis ailleurs. Comment est-ce que fait cette entreprise qui est confronté à un acheteur qui dit je ne bouge pas. Mépris et et à une augmentation des prix de l'électricité, il faut qu'on leur apporte des solutions, on y travaille. Aujourd'hui, nous ne voulons pas affaiblir notre base industrielle à cause de cette crise énergétique. Oui. Merci la parole est maintenant à notre collègue Marie-Claude Ryan pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste n'avait la parole. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. J'aurais pu vous adresser, monsieur le ministre ma question par la Poste. Mais il aurait fallu que je prenne mon mal en patience. Que je fasse le choix du thème revers et son délai désormais de J plus 3 ou alors que je paie une lettre hier une e-être rouge que je devrais scanner avant de l'emporter sur un site Internet afin qu'un agent des postes l'imprime et la transporte jusque chez vous. Cet agent aurait même accès à ma correspondance aussi confidentielles. Le timbre rouge n'est plus et vous entendez faire passer cela comme une lettre à la Poste expression voué à la désuétude selon vous. La mesure effective depuis le 1er janvier est un pas de plus vers la désagrégation du service public qui doit assurer l'égalité et l'équité. Et il n'y a pas de plan B cette dématérialisation synonyme de déshumanisation ignore la fracture numérique, qui concerne selon l'Insee, 13 millions de Français vont-ils devenir des sous-citoyens. En conséquence, vous lancer dans 68 communes, l'expérimentation de la réduction de fréquence du passage du facteur. Derrière la tournée du facteur. Monsieur le Ministre, l'accueil à un guichet, ce sont des Liens humains qui se tissent bien souvent avec les plus fragiles et les plus défavorisés. Or nous savons que tout ceux qui coupent les Liens sociaux abîme la démocratie. ce que nous dit à nouveau cette mesure c'est que la machine à exclure tourne à plein régime. Monsieur le Ministre quand allez-vous stopper cette opération de casse du service public essentiel pour la population quand le gouvernement va-t-il entendre qu'un service public n'est pas voué à être rentable.

Monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Vargas vous interroger le gouvernement sur l'évolution de la politique de courrier du groupe La Poste à laquelle. Nous sommes très attentifs et et vigilant avec la Première ministre et le ministre de l'Économie et des Finances et il ne nous a pas échappé qu'effectivement les les nouvelles. Les et vous les évolutions nouvelles ont suscité de la part de nos concitoyens, certaines questions et inquiétudes légitimes légitimes par de vous rappeler les les 2 raisons pour lesquelles la Poste fait évoluer aujourd'hui son offre de courrier. La première c'est que les usages de nos concitoyens ont évolué là où ils ont envoyé 45 lettre prioritaire en 2010, il n'en envoie que 5 en moyenne en 2021, ce qui ne veut évidemment pas dire qu'il ne faut pas en envoyer et que par ailleurs les évolutions prévues par le groupe de la Poste permettrait selon les calculs du groupe d'économiser 60.000 tonnes. De CO2 par an, soit 25% de la consommation conséquent, grâce notamment à à l'arrêt du transport aérien dans l'Hexagone. Ceci étant dit, si vous voulez bien me laisser terminer mesdames et messieurs les sénateurs, quelques éléments qui je l'espère, seront de nature à vous rassurer d'abord les timbres qui ont été les timbres rouges qui ont été achetés avant la fin de l'année sont évidemment fonctionnelle. D'autre part, la présence du facteur, six jours sur sept, n'est pas remise en question. Tout usager pourra. Se faire conduire au bureau de poste à tout moment par un facteur, c'est un engagement du groupe La Poste et enfin le. La lettre service plus qui arrive après deux jours et la lettre verte qui a qui arrive après 3 jours seront évidemment disponible enfin, s'agissant de l'expérimentation que vous avez évoquées. Elle ne remet en aucun cas en question la présence tous les jours du facteur sur les territoires et pour toutes les activités de distribution de la Poste. Je vous remercie. Monsieur le mythe.-- Le tien avec mon groupe, c'est qu'après l'hôpital. Le rail, l'énergie, la disparition du timbre rouge. Monsieur le Ministre symbolise le démantèlement de nos services publics Patrimoine de ceux qui n'en ont pas avec l'attaque contre notre système de, de retraite, c'est l'ensemble du dispositif de solidarité qui est mis en cause sous les injections de Bruxelles l'exaspération des Français est à son paroxysme en ce début d'année. Allez-vous enfin les entendre. Pour le groupe du Rassemblement des démocrates, progressistes et à des. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre, mes chers collègues. Nous changeons d'années mais les défis liés à l'actualité, eux, persistent. En ce début d'année où les cérémonies de voeux rythme nos soirées, nos semaine nous sommes tous ici. Interpellé par les élus locaux, les professionnels des TPE, des PME et nos concitoyens sur la crise énergétique actuelle. Interpellé à de nombreuses reprises sur les conséquences mais aussi sur la réponse politique et économique du gouvernement. Être entrepreneur requiert du sang-froid et beaucoup d'abnégation. La période actuelle en exige encore davantage. En effet, cela a été dit par mes collègues précédemment à l'image des boulangers de notre pays, parfois rares survivants du commerce de proximité dans nos territoires et particulièrement impacté par l'inflation des coûts liés à l'énergie. De nombreux professionnels des TPE, des PME n'arrivent pas toujours à identifier le niveau d'aide dont ils peuvent bénéficier et il ne dispose pas toujours du temps nécessaire pour décrypter les différents dispositifs mis en place par le gouvernement. Des dispositifs inédits. Pertinents et adaptés qui gagneront à être rappelé collectivement au plus grand nombre. Alors face à la désinformation parfois la la démagogie et aux approximations pour que tout artisan boulanger de notre pays puisse bénéficier des aides considérables en vigueur et continuer de travailler avec davantage d'optimiste je souhaite profiter de ces séances Madame la Ministre. Pour vous interroger sur le travail qui a été menée pour les Françaises et les Français. Au delà de leurs modalités ces dispositifs sont-ils efficaces sont-ils suffisants. Les réponses apportées aux boulangers, symbole des professionnels impactés ont-elles été entendues et enfin concrètement pour que chacune et chacun puisse bénéficier des aides. Comment l'État entend-il accompagner les professionnels pour faciliter leurs démarches. Merci. Merci monsieur le président, Monsieur le début le sénateur Rambo.-- Nous nous adaptons à la situation, une situation qui est compliqué pour nos artisans et pour nos boulangers en particulier. De 3 éléments. 12 milliards d'euros mobilisé au moment où on se parle 12 milliards d'euros pour aider nos PME nos TPE. Plus vous êtes petits. Plus vous êtes exposé. Plus vous êtes protégés. Vous êtes un boulanger 80% sont les chiffres de la Confédération des boulangers dépasse les 36 qui le VA ça été mentionné plafond du TRV tarif réglementé de vente. Vous avez un prix garanti de 180 euros le mégawattheure. Vous n'avez qu'une chose à faire une chose à faire. Remplir une case. Je suis une TPE sur l'attestation qui se trouvera à différents endroits pour être sûr que vous la trouviez en tant que boulanger sur votre espace professionnel sur votre fournisseur en ligne là où vous recevez vos factures mais aussi dès maintenant sur le site impôts Point gouv Point FR sur la page d'accueil, l'attestation est disponible, on peut la télécharger on coche une cache une TPE je veux bénéficier des conditions tarifaires et ce sera mise en oeuvre dès les prochaines semaines sur votre facture. Si ça ne suffit pas, l'amortisseur vient c'est très pratique, là c'est pareil, rien à faire, vous avez coché la case TPE, rien à faire. La facture tiendra on prendra en compte 15 à 20% de baisse directement sur la facture. Si vous êtes une TPE, mais aussi une PME ça suffit pas impôts Point gouv Point FR et là je me permets là aussi de répondre à Monsieur Husson

Ça fait juste six mois que les aides sont sur impôts Point gouv Point. FR. Il me semble important de rappeler que les aides, je passe mon temps à ça. Expliquait jusque sur les aides d'octobre novembre décembre on peut en disposer dès le 16 janvier en allant sur impôts Point gouv Point. FR. Une dernière chose, quand on est un artisan, on a confiance en celui qui déclare votre TVA tous les mois on travaille avec son expert-comptable. Je travaille avec les experts comptable qui sont aussi aux côtés de nos artisans en cas de doute, appelez les nous travaillons ensemble pour mieux accompagner au niveau des artisans boulangers, je vous remercie. La parole est à notre collègue Monique Lubin pour le groupe socialiste écologiste. Monsieur le ministre, hier soir, en écoutant les annonces de madame, la Première ministre et j'ai pensé à des amis des connaissances Isabelle Jean-Marc Philippe. La première travaille dans l'agroalimentaire. Depuis 40 ans et elle devait prendre sa retraite à 62 ans elle devra travailler un an et 3 mois de plus. Le deuxième il les charpentiers il entrent dans le dispositif carrières longues mais qui sera repoussée donc il devra travailler plusieurs mois de plus. Le troisième vient de perdre son emploi à 60 ans, peu d'espoir d'en retrouver un, et une durée d'indemnisation du chômage que vous venez généreusement de réduire et la perspective d'un meilleur revenu produit par la retraite qui s'éloigne. Vous allez faire payer votre réforme idéologique par ceux qui travaillent depuis longtemps déjà qui cotisent depuis longtemps déjà et qui ont les métiers les plus difficiles et les moins bien rémunérés et par les précaires et dans le même temps vous ne demander aucune contrepartie aux employeurs. Vous refusez obstinément de mobiliser les gains parfois faramineux engrangés par certains depuis quelques mois. Alors Monsieur le Ministre, vous qui ne cessaient de mettre en avant la valeur travail, pourquoi maltraitez-vous à ce point les travailleurs.

La réforme est nécessaire. J'ai évoqué. La raison pour laquelle il fallait la faire pour sauver le système par répartition. J'ai aussi dit qu'il fallait faire avec le plus de justice possible. Il y a 2 éléments qui répondent très précisément à votre question. Le premier élément c'est que nous avons dans le cadre de la concertation, que j'ai menée depuis plusieurs mois travailler avec l'ensemble des partenaires sociaux, tous les partenaires sociaux, tous les syndicats, toutes les organisations patronales et avec les groupes politiques que nous avons consulté et nous avons nous avons abouti nous avons abouti sur un certain nombre de convergence ça n'efface pas les désaccords sur l'âge mais il y a des convergences sur la question de la pénibilité. Nous modifions contre le le compte de personnel de prévention. Avec l'ensemble des secrétaires pour en faciliter l'acquisition des points nous créons la possibilité d'un véritable congé de reconversion, nous faisons en sorte de mieux protéger ceux qui travaillent de nuit ou en équipe Posté, nous allons retravailler sur la question des ports de charges des postures pénibles des des vibrations pour faire en sorte que les accords de prévention soit là et c'est un milliard d'euros sur 5 ans, qui seront consacrés au financement de la prévention tout en renforçant la possibilité de partir de manière anticipée dans le cas d'un suivi médical renforcé sur les carrières longues. Vous l'avez évoqué, nous maintenons évidemment et bien évidemment le départ à 58 ans pour tous ceux qui ont cotisé cinq trimestres avant saison. Nous maintenons le dispositif existant, celui qui permet de partir avec 2 ans d'avance pour ceux qui ont cotisé cinq trimestres avant 20 ans et nous créons un nouveau dispositif qui va s'appliquer très certainement à ce que vous avez évoquées pour que ceux qui ont cotisé cinq trimestres avant 18 ans et je pense tout particulièrement aux apprentis que ceux-ci puissent partir avec 4 ans d'avance et à 60 ans sans qu'il y ait de bouger d'âge pour ceux qui ont commencé à travailler plus tôt la la vérité, madame la sénatrice. Elle est peut-être sur 2 points le 1er c'est que les exemples que vous avez cité les amis que vous avez auquel vous avez pensé, je souhaite pour vous que ce soit des amis imaginaires. Parce que le principal bouger le principal décalage de leur âge de départ, c'est la hausse de la durée de cotisation. Vous avez voté en 2013 et la 2ème, chose que je vais vous dire, c'est qu'en vous écoutant je, j'ai en tête les propos du responsable du parti socialiste qui s'est converti à la doctrine de Jean-Luc Mélenchon vous avez ainsi perdu le sens de la raison et la responsabilité. Monsieur le Ministre qu'il est doux à mes oreilles de vous de me faire des remarques à moins sur ce qu'a fait ma famille politique et ce que nous avons voté quand ça vient de vous Monsieur le Ministre. Vous et moi savons très bien. J'ai quelques souvenirs. Monsieur le Ministre, dans le département des Landes avec un de mes grands anciens qui s'appelait Henri Emmanuelli et que vous aimiez beaucoup à l'époque et dont vous appréciez beaucoup à l'époque. Voilà. Fallait Voilà. Fallait pas me tenter, Monsieur le Ministre, le corps le corps dit que la part des retraites dans le PIB, c'est 14% que ça ne bouge pas et que donc le système n'est pas en danger. Les critères de pénibilité que vous venez de donner, c'est vous qui les avait enlevés en 2018. Quand vous êtes arrivé au gouvernement. Et vous pouvez le traduire comme vous voulez. Monsieur le Ministre mais cette réforme vous la faites uniquement de payer par les salariés et par les plus modestes des salariés et j'ai entendu tout à l'heure des réactions quand je citais mes amis qui ne sont pas imaginaires croyez le. J'ai entendu. Or, mais quand on a travaillé 42 ans et qu'on demande de travailler un an de plus, c'est un an de trop. La parole est maintenant madame. La présidente Sophie Primas. Pour le groupe Les Républicains. Ma question s'adresse à Madame pas. Agnès Pannier-Runacher. Depuis un an notre pays traverse une crise énergétique effroyable. Le gouvernement allume bien sûr des contre-feux. Nous avons entendu quelques explications bouclier tarifaire amortisseurs filet de sécurité. 24 milliards d'euros en 2022, 43 milliards en 2023. L'échec comme mode de gouvernement sont très dangereux, vous le savez financé par de la dette mal calibrée complexes dans leur exécution insuffisant toujours insuffisant. À défaut de solution structurelle vous arroser le sable avec de l'eau. La solution structurelle, elle est européenne, car nous sommes aujourd'hui prisonnier de l'architecture européenne du prix d'électricité liant Électricité, gaz, charbon. Madame la Ministre l'état de guerre a pulvérisé le marché énergétique, la disparition du gaz russe la déséquilibrer profondément et probablement définitivement. Il faut donc tiré les conséquences de cet état de fait et abolir immédiatement les mécanismes de concurrence qui génère l'architecture du prix de conseil européen au Conseil européen. Nous ne voyons rien venir, nous ne voyons rien bouger. À défaut, pour la France d'avoir le poids désormais suffisant en Europe pour faire bouger les choses. Demander des dérogations immédiate d'autres l'ont fait, y compris dans des pays où l'interro par habilité et forte, madame la Ministre, c'est urgent, on ne peut plus attendre les prochains conseils européens. Notre économie ne le supportera pas. Merci de nous dire votre action. Merci beaucoup monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, madame la présidente Prima. Vous l'avez dit, nous avons d'abord agi au service des ménages au service des entreprises et au service des collectivités locales en prenant le plus rapidement possible, des mesures qui font qu'aujourd'hui la France. Offre ou permet assez différentes catégories d'avoir le prix de l'électricité, le plus bas d'Europe. Je veux le rappeler, car ce n'est pas une politique du chèque c'est une politique qui est assis aussi sur une contribution sur la rente infra-marginal c'est-à-dire le surplus de bénéfices que crée cette situation particulière de crise énergétique que vous avez souligné sur plus de bénéfices chez nos producteurs d'électricité, donc c'est aussi une approche où nous savons gérer le budget de l'État a de bonnes fin avec des aides proportionnée. Les ménages et les TPE étant les mieux protégés. J'ai obtenu, cela a été rappelé avec Bruno Lemaire Olivia Grégoire ce plafonnement du prix de l'électricité des contrats 280 euros du MWh. Vous soulignez très justement que l'action doit se passer aussi au niveau repères hein. Vous avez raison de le souligner parce que ce que nous subissons, c'est d'abord un acte de guerre, 40% de l'approvisionnement en Europe de gaz et d'origine russe, 22% de la production d'électricité européenne est basé sur le gaz. Ça c'est une réalité physique dont il faut prendre en compte. Vous savez également, on en a parlé encore ce matin en commission développement durable et Affaires économiques pour la présentation du projet de loi nucléaire que la situation de notre parc nucléaire nous rend aujourd'hui, dépendants de l'approvisionnement en électricité de la part d'autres pays européens et donc c'est une réalité également physique dont il faut prendre en compte. nous avons agi en européen tout ce qui nous permet aujourd'hui de passer cette crise. Et ce cet hiver avec une à une baisse des prix l'électricité certes pas satisfaisante mais nettement inférieur au début de l'année, grâce au stockage de gaz grâce au Flat plafonnement du prix du Est due aux décisions que nous avons pris au niveau européen et la Commission présentera au 1er trimestre grâce à l'action du gouvernement, une proposition sur le marché. L'évolution du marché de l'électricité dans le sens que vous appelez de vos voeux. Je veux remercier. J'ai encore quelques instants. Je rêve d'un pays fort en Europe, madame la Ministre, nous étions un pays fort en Europe capable d'imposer des décisions à l'Europe. Or là il y a urgence, il y a une grande urgence car à la fin du 1er trimestre quand tu l'Europe aura pris cette décision peut être nous aurons dépensé dans le budget de l'état des milliards d'euros au travers de chèques et nous n'auront toujours pas de solution structurelle. Donc, je rêve d'un pays fort capable de faire bouger l'Europe et de prendre des décisions au bénéfice de notre pays. La parole est maintenant à notre collègue Victorin Lurel pour le groupe socialiste, écologiste et républicain ordonné. Monsieur le président, mes chers collègues.-- Compte tenu de la gravité du sujet et de son caractère interministériel. Ma question s'adresse à Madame, la Première ministre. J'y associe mes collègues Catherine Conconne et victoire Jasmin. Elle porte sur le non-lieu prononcé le 2 janvier dernier dans l'enquête sur la contamination et la pollution au chlordécone. Je respecte les décisions de justice mais à l'espèce personne ne pourraient s'en satisfaire. Sa décision est une indéniable Denis. Denis pouvant allumer des brasiers puisqu'il n'y aurait ni coupable ni responsable. Bien qu'attendue, cette décision ajoute au scandale d'État. Un scandale judiciaire. Madame, la Première ministre. Au-delà des actions menées par tous les gouvernements et par le vôtre. Des plans mis en place et de la reconnaissance de la carence fautive des pouvoirs publics. Je considère, pour autant que l'État reste coresponsable. Majeur de cette tragédie et en reste donc encore comptable. 46 ans après les premières. Alertes. 16 ans après la première plainte vous ne pouvait rester indifférente. Alors je formule ici quatre demande au delà des suites que les parties civiles ne manquons pas d'intenter contentez-vous tout faire dans le respect du droit pour que le Parquet rouvre ce dossier. Êtes-vous prêt à créer un fonds d'indemnisation pour toutes les victimes. Êtes-vous prête à faire pour les victimes du chlordécone, ce qui a été fait pour les victimes de l'amiante. Êtes-vous prête à renforcer l'action de l'État dans la recherche fondamentale dans la dépollution des eaux et des sols. J'attends de vous une réponse humaine, débarrassée de toute vaine polémique. Jean-François caraco délégué en charge des Outre-Mer.-- Monsieur le président, monsieur le sénateur. J'ai eu l'occasion de le dire hier à l'Assemblée nationale. Je constate comme vous. La décision prise librement par les autorités judiciaires. Un membre du gouvernement ne peut qu'en prendre acte. J'ai bien lu les attendus de l'ordonnance. Il pointe une responsabilité collective dans ce scandale sanitaire. Mais vous l'avez dit cela l'amoindrit en rien la responsabilité de l'État face à ce scandale reconnu d'ailleurs pour la première fois par le président de la République en 2018. Et nous devons continuer d'avancer sur ce chemin.-- Notre priorité à tous c'est de protéger la santé de nos concitoyens. Des des les secteurs économiques impactés de renforcer la recherche. Avec Gérald Darmanin, que le ministre de la Santé. Le gouvernement s'est engagé et s'engage encore à répondre à ces enjeux. Puis y avancée forte j'insiste là-dessus ont déjà été obtenu. La reconnaissance du cancer de la prostate comme maladie professionnelle ouvrant droit à indemnisation. Analyse gratuit du taux de chlordécone dans le sang. Analyse des sols ou encore conséquent de travaux de recherche engagés pour la dépollution des sols. Le colloque scientifique, il les rencontre du terrain le terrain du mois de décembre ont été l'occasion de porter à la connaissance. Ses nombreuses avancées. Mais ils ont montré aussi qu'il y avait encore beaucoup à faire. Dans ce cadre. Je note vos propositions qu'il nous faut étudier avec attention les volonté d'aboutir. Si l'ordonnance et le droit et la chose jugée. Cela ne nous empêchera pas de continuer à avancer. J'aimerais en Martinique dès demain en partie pour cela la coordonnatrice du plan chlordécone m'accompagnera à cet effet. Je vous remercie. Madame, la Première ce regrette que vous n'ayez pas saisi d'occasion ici pour marquer votre considération aux populations de Martinique et de Guadeloupe, frappée de sidération est déjà marqué dans leur Chair. Monsieur le Ministre, vous me faites une réponse que je connais et qui est celle d'un communicant. Vous savez fort bien que tous les gouvernements ont engagé des actions et qu'aujourd'hui. les pleins. Connaît notamment le quatre était insuffisant. Il est sous-dotée et les sous-financé 2,4 millions pour la recherche fondamentale par an, ce n'est pas suffisant, il faudrait au moins 5 10,8 millions par an alors que nous mettions 12 millions en 2010 avec Monsieur Sarkozy et et 13 millions en en 2 et le 16 il faut c'était suffisant. Monsieur le président. Je demande que le gouvernement nous fasse bénéficier du préjudice d'anxiété. À l'instar de l'amiante. La parole est à d'autres collègues. Alain Milon. Pour le groupe Les Républicains. Merci monsieur le président. Monsieur le ministre de la Santé. Le président de la République a dit clairement, on a insisté de reconstruire notre système de santé pour l'adapter et satisfaire les attentes des professionnels comme des patients, mais pour y parvenir une réforme globale de l'organisation de ces soins de leur mode de financement et des synergies à mettre en oeuvre et nécessaire pour restituer une attractivité perdue et pour fonder un système innovant performant viable et humain. Hélas les orientations proposées, pose davantage de questions que de solutions efficaces et urgentes, le financement est absent totalement de ce discours présidentiel, sortir de la T2A, par exemple, dès le prochain PLFSS pour lui substituer une rémunération basée sur des objectifs de santé publique, négocier à l'échelle du territoire fondée sur un critère populationnelle non défini. Ça laisse perplexe. Comment imaginer que l'objectif d'efficience puisse être atteint tout en rendant la part de financement à l'activité minoritaires, c'est bel et bien à notre avis sonner le glas de l'hôpital. Quant aux 6000 postes d'assistants médicaux supplémentaires c'est pendant trois ans, l'assurance maladie qui paiera. Quid de l'après et comment l'assurance maladie pèsera-t-elle quand on sait que les 4000 assistants déjà mises en place coûte à celle-ci, 160 millions d'euros. Les propositions concernant la médecine de ville ne sont pas à la hauteur et ne permettent pas d'enrayer la crise de vocation ni la propagation des déserts médicaux. comment entendez-vous répondre avec précision et concrètement aux attentes des soignants hospitaliers et libéraux sans procéder à une refondation complète des modes de financement entre les différents sénateurs que les différents financeurs pardon que sont la sécurité sociale de pas, d'une part et les mutuelles. D'autre part.

Le 6 janvier dernier, le président de la République a tenu un discours devant les les soignants traçant un nouveau cap. Une feuille de route pour la refondation complète de notre système de santé avec un diagnostic lucide mais surtout un changement dans l'analyse et la méthode, vous le savez passer d'un système qui a été construit autour de l'offre de soins. Forcément concurrentiel vers un système pour plus répondre aux besoins de santé de nos concitoyens beaucoup a déjà été fait, que ce soit dans le Ségur, que ce soit entre autres la suppression du numerus clausus. Mais nous devons aller effectivement plus loin, plus vite pour répondre aux défis qui sont devant nous et qui d'ailleurs concerne l'ensemble des pays européens et d'une façon générale, l'ensemble des pays industrialisés. Il y a des axes forts régler le problème à l'échelle de chaque territoire sortir de cette le Juke concurrentiel pour travailler en complémentarité ville hôpital hôpital clinique. Médecins, paramédicaux médicaux administratifs et puis retrouver des collectifs à l'échelle humaine, comme en particulier les chefs des services pour l'hôpital, redonner du temps médical de redonner du temps de soins est un enjeu majeur car comme l'a précisé le le président ce n'est pas tout de suite que nous aurons les médecins que nous attendons, après la suppression du numerus clausus. Alors comment faire, laisser les soignants faire ce pourquoi ils sont formés, c'est-à-dire le soin développer des assistants médicaux en l'aidant à cette installation. Les maisons de santé pluri-professionnelles à l'hôpital en intégrant les logisticiens des administratifs au plus près du service, il faut utiliser les mieux les compétences de chacun. La plus-Value de chaque professionnel au sein d'équipe traitante autour du médecin traitant ou au sein des services de l'hôpital raisonner, territoire par territoire. Réformer, vous l'avez dit, le financement de notre système de santé en particulier en sortant de la T2A, qui n'est qu'un financement qu'à l'acte en s'ouvrant vers un financement certes toujours à l'acte pour certains mais qui répond aux besoins de santé de la population et qui ait un financement à la qualité à l'efficience. Nous l'avons fait déjà pour les services d'urgence. Nous allons continuer à le faire pour l'ensemble des médecins généralistes sont déjà dans cet axe. Ce sont des engagements forts envers les soignants envers nos concitoyens pour leur santé et soyez assurés que nous allons les développer très rapidement parce que les échéances sont courtes et que je serai totalement motivés et mobilisés pour ce faire cela.-- merci Monsieur le Président, les propositions que vous venez de nous faire ce sont des propositions que nous faisons depuis des années on a déjà entendu sous différents ministre depuis Madame Marisol Touraine, en passant par Madame Buzyn et par monsieur Véran. Il y a finalement rien de nouveau à ce niveau là, il y a donc aucune vision alternative qui structure la réflexion du gouvernement. Moi je vais vous en donner quelques-unes, si vous permettez, dans le système de santé qui se construisent. Il y a les soins primaires il y a le panier de soins réguliers, il y a la mise en réseau obligatoire il y a un pilotage fort et décentralisé, on n'a jamais parlé de décentralisation dans le pilotage des ARS et c'est bien dommage. Une réflexion globale sur le financement et non pas simplement une réflexion telle que vous la donner mais, réflexion sur l'ensemble du financement, en particulier sur les dépenses. Merci. La parole est à notre collègue Pierre-Antoine Levi. Pour le groupe de l'Union centrer. Merci monsieur le président, mes chers collègues. Question s'adresse à Monsieur le Ministre délégué chargé du numérique. Monsieur le Ministre, comme ma collègue, Paris à tout à l'heure et beaucoup de Français et beaucoup de Français, je me pose cette question, où va le service public postal aujourd'hui. En effet, depuis le 1er janvier, le timbre rouge réservé aux envoie de l'aide prioritaire ne sont plus commercialisés. La modernité selon La Poste c'est soi-disant là y'lettres rouges. Il faudra donc se connecter en ligne pour rédiger au scanner une lettre qui sera ensuite retranscrites puis imprimés par un agent de la Poste avant d'être envoyés. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Oui la confidentialité dans 10 écrit dans ce nouveau process. Cette prétendue révolution peu surtout le problème de l'accès de tous au service public postal. L'égalité, pourtant l'un des grands principes de la notion de service public dans notre pays. La réalité c'est qu'en pratique l'illectronisme touche près de 14 millions de nos concitoyens. Surtout en milieu rural. Alors certes, ils pourront toujours aller dans un bureau de poste pour envoyer leur lettre prioritaire. Si bien sûr il y en a un, il n'est pas fermée. Mais comment expliquer aux citoyens qui fasse est président utiliser un automate une borne pour faire envoyer leurs lettres après avoir scanner des documents. De plus, en pratique, les agents de ces bureaux de poste ne pourront pas toujours aider ces personnes lorsque l'affluence est très importante, seront laissés seuls devant l'automate. Cette réforme donne comme une impression de rajouter de la complexité à quelque chose qui était à la base, fort simple. En fait nous apprenons également qu'à partir du mois de mars. Le courrier ne serait plus distribué tous les jours, mais un jour sur deux, puis pourquoi pas un jour sur 3. Cette réforme est à l'expérimentation dans certains départements, mais elle risque d'être généralisé à toute la France. Mais le risque est grand que cette réforme désorganise le service postal et qu'elle aboutisse in fine et à la suppression de nombreux emplois. Alors ma question est simple, monsieur le ministre et vous n'avez pas répondu tout à l'heure. Allez vous blessés continuer à se déliter ce service public historique. Il est urgent d'agir avant que nous devenions tous timbrés, je vous remercie. On vous réponde. La parole est au ministre délégué en charge des télécommunications. les constats qui ont conduit le groupe La Poste a à prendre ses décisions, mais je veux réaffirmer une nouvelle fois. Le profond attachement du gouvernement à l'univers. À l'universalité du service postal qui est d'ailleurs inscrite dans la loi, redire une nouvelle fois que la présence du facteur est maintenu, six jours sur sept que tout tu t'as usagers rencontrant des difficultés ayant la nécessité d'effectuer un envoi prioritaire pourra se faire accompagner, enfin par un facteur au bureau de poste et qu'enfin les services. Liés à la lettre. Plus qui arrive 2 jours après à destination et la lettre verte qui arrive 3 jours après à destination seront évidemment S'agissant de l'expérimentation que vous citez. Elle vise à tester de nouvelles modalités distribution dans les 68 communes que vous évoquiez, mais en aucun cas elle ne remet en question la présence tous les jours du facteur sur l'ensemble du territoire. En revanche, monsieur le sénateur. Je ne pourrai laisser dire sur d'autres bancs, peut être que ce gouvernement ne se désintéressent de la fracture territoriale. Avec 2600 Maison France service répartis sur l'ensemble du territoire avec Action coeur de ville avec Petites Villes de demain avec territoires d'industrie avec 4000 conseillers numériques qui ont accompagné 1.300.000 personnes depuis un an sur le territoire national, c'est ce gouvernement qui a mis fin à une quinzaine d'années d'aveuglement sur l'aggravation de la fracture territoriale. Et je crois que vous en conviendrez, soyez monsieur le sénateur, mesdames et messieurs les sénateurs, convaincu de l'attachement de ce gouvernement, à la résorption de la lutte contre la fracture territoriale.

le confirmeront, La Poste ne distribue pas six jours sur sept mais certaines fois 4 jours ou 5 jours et que cette expérimentation inquiète énormément de Français dans tous les territoires. Donc je vous le redis qu'allez-vous faire pour éviter le délitement du service public. La parole est à notre collègue Hugues Saury. Pour le groupe Les Républicains. à la fin du mois de décembre, les autorités en place à Ouagadougou. On te demande des sous d'obscurs prétextes. Le départ de l'ambassadeur de France, nouvel épisode des tensions qui émaillent nos relations avec le Burkina Faso n'est pas sans rappeler le scénario qui s'est déjà produit au Mali et en Centrafrique. Il illustre surtout le fait que dans cette partie de l'Afrique, où elle a pourtant tant oeuvré. La France est récemment devenu indésirable. Malgré l'engagement de nos militaires contre le terrorisme islamiste et le sacrifice de 53 d'entre eux. Malgré le niveau considérable de l'aide au développement déployés dans cette zone prioritaire. Jamais la France n'y a été tant critiqué étant rejetés nous quitte ses concitoyens expatriés en subissent, malheureusement les effets mais plus largement c'est bien dans l'ensemble du continent africain que l'influence économique politique diplomatique ou même culturel de notre pays ne cesse de s'éroder ses parts de marché ont ainsi fondu de moitié par rapport au début des années 2000 et ce recul ne fait que s'accélérer depuis l'année dernière. La France n'est plus le 1er partenaire commercial d'aucun des pays du Maghreb dans de nombreux pays la langue française voit son influence reculer et maintenant concurrencé par l'anglais jusque dans les programmes scolaires voir comme au Rwanda en tant que langue officielle. Et si la France reste le 1er pays de destination des étudiants africains sa capacité à attirer, pour les former sur son sol les futures élites et désormais en recul par rapport à d'autres destinations avec ces formidables atouts aussi bien humains que naturel, l'Afrique est à n'en pas douter un continent d'avenir mais cet avenir. Si nous ne sommes pas capables de remettre à plat l'ensemble des politiques que nous y menons. Ces dernières années, risque fort de s'écrire sans la France depuis 2017, la situation s'est dégradée et nous envoyons aujourd'hui les conséquences. Alors Madame la Ministre quelles stratégies. Le gouvernement entend-il, mettre en oeuvre au cours de ce quinquennat pour enfin enrayer le déclin général de l'influence française en Afrique On vous réponde. La parole est à la madame la Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, madame Colonna.-- Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur. Disons les choses. En Afrique comme ailleurs, les manipulations de l'information ne cesse de prendre de l'ampleur et dans plusieurs pays, la France est visée par des campagnes des campagnes qui n'ont rien de spontané. On le sait, et nous le savons bien, parce que la secrétaire d'État aux partenariats internationaux étaient hier encore au Burkina Faso, je la remercie de cette visite elle est allée porter un message qui était clair, comme vous l'avez vu. Face à cela, nous devons agir mais nous devons agir avec les moyens les outils d'une démocratie et c'est ce que nous faisons nous opérons un triple changement j'ai demandé à mon ministère de le mettre en oeuvre car oui nous devons changer l'Afrique change et nous devons également changer un changement de contenu. Il s'agit de mieux expliquer la réalité de nos partenariats ou l'innovation, les entreprises, les artistes, les jeunes ont une place centrale. Changer c'est aussi se placer au soutien de ceux qui journalistes fact-checkers. Lutte contre la désinformation. Changement de support, ensuite il s'agit pour nous d'être partout présent, beaucoup plus qu'auparavant partout présent où se forment les opinions africaines, y compris sur les réseaux sociaux et permettre ainsi de nous adresser à un public plus jeune. Et enfin, changement d'échelle par l'accroissement du volume de ce que nous produisons et par la mobilisation du réseau diplomatique est en prise avec les réalités et les interlocuteurs locaux tout ceci Monsieur le Sénateur, en complément de nos relations humaines de nos relations économiques qui persistent qui changent, elles aussi, l'enjeu est considérable. Vous l'avez dit, soyez assurés que notre mobilisation l'est tout autant si je suis arrivé avec quelques instants de retard après le début de cette séance, je vous en. Présente mes excuses c'est que le président de la République recevait le président des Comores et après cette session. Je me rendrai à Addis Abeba avec ma collègue allemande, siège de l'Union africaine. Donc nous sommes actifs. Vous le voyez, je vous remercie.-- Merci la parole est maintenant notre collègue et oui ils viennent tous mes rôles pour le groupe socialiste écologiste.-- Merci monsieur le président. Chers collègues, ma question s'adresse à monsieur le ministre de la Santé et de la prévention. La pénurie de médicaments sujet quasiment inexistante dans les années 2010 devient un problème majeur de sécurité et de souveraineté nationale avec une aggravation des tensions depuis la crise Covid en 2023 nous d'une bande non encore et toujours de l'Inde et la Chine en particulier, à qui nous achetons plus de 80% des matières premières, moins de 40% des médicaments sont fabriqués en Europe. Pourtant dans le monde d'après, tout serait différent. Le président Macron nous l'avait assuré la France allez retrouver sa vous venez sa souveraineté industrielle. Or les pénuries et les tensions n'ont jamais été aussi forte en particulier sur les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur et à l'hôpital. Certains anti-cancéreux ou immuno-suppresseurs utilise dans les greffes du rein par exemple manque obligeant à choisir les patients pouvant en bénéficier. C'est une perte de chance. Inadmissible pour les patients. Et d'autres pénuries de médicaments aussi courants que le paracétamol ou l'amoxicilline oblige les pharmaciens à délivrer les boîtes au compte-gouttes alors Monsieur, Monsieur le ministre, ma question est simple, quelle est votre stratégie pour retrouver une production en France ou pour le moins en Europe.

Je partage en partie votre diagnostic mais je vais préciser un petit peu les choses. 2 années de crise sanitaire, celle que nous avons traversées ont bouleverser complètement notre consommation et entraîné à la clé, des difficultés d'anticipation des volumes de production par les industriels. Parallèlement à cela, nous constatons une forte reprise de la consommation, plus 13% par exemple en France. Oh pour le paracétamol et également dans des pays comme la Chine, on le voit bien, c'est une situation qui ne concerne pas que la France n'aime pas que l'Europe qui est une situation aujourd'hui mondiale. Notre système d'alerte nous permet d'anticiper.-- Autant que faire se peut. Cette situation grâce à un suivi de nos stocks stratégiques mais je, je comprends bien sûr et je vois l'inquiétude des gens qui vont chercher les, les médicaments dans les pharmacies, tout en sachant la mobilisation remarquable des pharmaciens qui se mobilisent très fort pour trouver les différents produits. Alors face à ce diagnostic. Nous avons mis en place un traitement. Nous avons agi tôt nous interdisons les exportations à l'étranger ce qui est en France reste en France nous contingent on les stocks nous adaptons pour avoir une répartition homogène sur l'ensemble du territoire. Nous échangeons avec les laboratoires concernés pour prioriser certaines formes de médicaments. Nous avons autorisé la reproduction d'amoxicilline par des laboratoires en France. Nous adaptons la dispensation en officine, vous l'avez dit au juste besoin des patients et nous travaillons avec les professionnels sur les alternatives thérapeutiques ça c'est des actions immédiates nous allons plus loin en reconstruisant notre souveraineté industrielle mais ça va pas se refaire en cinq minutes, bien évidemment la France investit massivement depuis plus d'un an. Dans le cas de France relance dans le cas de France 2030. Des projets de relocalisation très concrets sont en train de voir le jour. Je pense au paracétamol dans le projet c'est 15 également des masques, des gants nitrites et puis à Arras une usine pour la production de médicaments dérivés du sang. À partir de plasma sanguin. Donc oui nous sommes dans l'axe pour regagner notre souveraineté en France au sein de l'Europe sur les médicaments et en attendant, nous faisons le maximum pour que tous les Français puissent avoir les traitements qui leur sont nécessaires. Je vous remercie.--

plusieurs solutions et en particulier le renforcement de nos capacités de production publique avec la pharmacie centrale des hôpitaux des armées ou la possible réquisition d'entreprises et il faut surtout un plan concerté de réindustralisation en France et en Europe. Les industriels argue d'un prix trop bas des médicaments alors mettons cartes sur table sur la fixation des prix qui est aujourd'hui protégé par le secret des affaires pour qu'ils tiennent compte des aides publiques directes ou indirectes dont ils bénéficient. La loi du marché et le libéralisme ne peuvent gouverner notre politique en matière de produits de santé rembourser une fine et par la sécurité sociale, donc l'argent de tous les contribuables pour construire une véritable indépendance de la production, il faut une politique publique forte et volontaristes. Merci la parole est à notre collègue Christine Lavarde. Pour le groupe Les Républicains. monsieur le président, Monsieur le Ministre là. L'édition 2023 du CES de Las Végas se vient de se clôturer. Elle a laissé une part large aux automobiles et à cette occasion, le PDG de Stellantis, Carlos Tavarès a lancé une nouvelle charge charge contre le niveau du prix extrêmement extrêmement bas des véhicules chinois zéro émission qui met en péril l'industrie européenne et cette industrie pour le seul territoire national ces 210.000 emplois Directs, auxquels il convient d'ajouter tous les emplois indirects si j'en crois les les objectifs affichés par 3 constructeurs chinois pour les cités. Jelly sec et Great Wall, à eux 3 ils envisagent d'importer un million de véhicules sur les territoires européens d'ici 3 ans, ils sont déjà en train de construire le système de distribution qui leur permettra d'atteindre cet objectif. certes sur le territoire national, les véhicules électriques progressent, plus 46% d'immatriculations en 2021, mais 80% de ces véhicules sont importés et la presse ne s'y trompe pas, elle écrit d'ailleurs le loup chinois est dans la bergerie en effet la Chine c'est 50% de la valeur totale d'un véhicule électrique c'est 75% de la chaîne de valeur valeur des batteries c'est 90% des moteurs électriques produits dans le monde, et face à tout ça. L'industrie européenne est en très grande difficulté, elle ne parvient même plus à pénétrer le marché chinois. Alors dans cette bataille qui vient de commencer, Monsieur le Ministre quelles sont nos armes avez-vous choisi une guerre de position et donc de continuer à subir les assauts chinois ou entendez-vous sortir de notre tranchée et lancer une guerre de mouvement. de mouvement. La parole est au ministre de l'économie et les finances. De la souveraineté industrielle. Monsieur Bruno Lemaire. Merci monsieur le président, madame la sénatrice. Remercie protection de questions me répondre très clair, nous sommes favorables à une guerre de mouvement. Avec de l'offensive et de la défensive. L'offensive s'être capable d'avoir au XXIe siècle, une industrie automobile électrique en France, en Europe aussi performante que celle que nous avons eu sur le véhicule thermique au XXe. Je rappelle que c'est ce gouvernement cette majorité qui a pris l'initiative il y a maintenant près de 4 ans de mettre sur pied une filière de batteries électriques pour être moins dépendant de la Chine. Nous allons ouvrir les deux premières usines de batteries électriques. Nous avons un objectif à 2030 de produire environ 100 à 120 gigawatts de puissance électrique avec des batteries produites en France sur les territoires français, vous savez, vous avez travaillé dessus que nous nous voulons rouvrir une usine de lithium que nous voulons diversifier nos approvisionnements. Nous voulons également être indépendant en matière de semi-conducteurs qui sont absolument indispensables. Ce véhicule électrique. Nous avons obtenu l'investissement de GlobalFoundries sur le site d'STMicro pour pour développer massivement la production de semi-conducteurs qui serviront aussi aux véhicules électriques, donc l'objectif est très clair, être indépendant en matière de production de véhicules électriques. Ça c'est l'offensive. Les matériaux. Les batteries. Les semi-conducteurs et au bout du compte, comme l'a annoncé d'ailleurs Stellantis la production ces véhicules électriques sur le sol français et croyez-moi l'offensive sera très volontariste près il y a une question que vous soulevez qui était majeur et moi je vous invite à participer aux travaux tous auront lancé sur le projet de loi de réindustrialisation verte. Jusqu'où allons-nous dans le volet défensif. Est-ce que par exemple, nous réservons les aides 7000 euros aujourd'hui par avec l'électrique à des véhicules produits et assemblés uniquement en France, en Europe, la question est légitime après tout d'autres le font. Faut-il renforcer le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières pour dire ça ne concerne pas uniquement le ciment, l'acier, l'aluminium, mais ça peut aussi concerner des vrais biens manufacturés par exemple des automobiles. Je n'ai pas la réponse à ces questions, mais le défensif, être capable d'avoir l'audace de poser ses questions de discuter avec tous les sénateurs et les sénatrices que souhaiterait, dans le cadre du projet de loi sont vertes. Nous sommes clairs avec la Première ministre a met sur pied des volet défensif pour être autonome sur le véhicule électrique. Alors Monsieur le Ministre, certaines des questions que vous venez de poser, pourtant vous avez donné la réponse en octobre dernier devant la plateforme automobile, vous avez dit qu'il fallait pas de se laisser envahir et qu'il fallait réserver les aides à des véhicules produits en Europe, c'est ce que vous a proposé le Sénat, nous avons ici adopté un amendement qui venait de diminuer de 500 millions. Ces aides qui sont versées essentiellement aux industriels chinois. Vous l'avez retirée. C'était pourtant une mesure de souveraineté et qui venaient aussi à améliorer notre déficit budgétaire et vous ne l'avez pas gardé. C'est bien dommage. La parole est à notre collègue Jean-Pierre Vogel. Pour le gros plairait public hein. Merci. Merci. Si monsieur le président, ma question s'adresse à Madame, la ministre Olivia Grégoire. La filière équine représente plus de 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires 20.000 entreprises et 66.000 emplois Directs cette filière irriguent notre territoire. Elle est présente dans 91% des cantons avec plus d'un million de chevaux. L'équitation, c'est aussi 2 millions de pratiquants, dont 700.000 licenciés et donc la 3ème fédération olympique et le 1er sport féminin. Le monde du cheval, enfin plus de 827 millions de recettes directes pour l'État à travers les Parisi. Et 295 millions d'euros à travers la TVA. Dans la période que nous traversons. Oh beaucoup de Français ont du mal à boucler leurs fins de mois, les activités qui ne constitue pas un luxe mais une force économique pour nos territoires ruraux et la passion d'un grand nombre de nos compatriotes. Comme vous le savez, à la suite d'une décision de justice européenne la filière se bat depuis plus de 10 ans pour retrouver un taux de TVA conforme à son caractère agricole et lui permettant d'être compétitive. Je rappellerai juste qu'en Irlande concurrent Direct de nos éleveurs. La TVA est à 4,1%. Alors que le Sénat avait voté dans le PLF, un amendement permettant de revenir à un taux réduit pour la filière et au lendemain de l'adoption du budget 2023 par le 49.3. La déception est grande. Le président de la République avait pourtant obtenu en 2022 la révision de la directive TVA pour permettre à la France de revenir au taux réduit antérieures et s'était engagé à les appliquer dès que possible. Ma question est donc simple, Madame la Ministre quand et par quel véhicule législatif. Le gouvernement donnera la filière équine un cadre fiscal garantissant sa pérennité et son développement et le respect de la parole donnée. On vous répondre. La parole est à madame Olivia Grégoire ministre délégué. En charge et petite dévoyée d'entreprises du commerce et de l'artisanat. Monsieur le sénateur Vogel. Merci pour votre question qui me permet de me permet de souligner remercier d'ailleurs la constance de la position du gouvernement sur la question du cadre fiscal de la filière équine. Ça vous a été. Rappelé je crois lors des débats sur le projet de loi de finances pour 2023, la cohérence du système fiscal repose sur une application du taux réduit de la TVA de 5 5. Qui est comme vous le savez bien réservé aux biens et services de première nécessité évidemment des denrées alimentaires mais aussi des appareillages des équipements pour les personnes handicapées ou encore le logement et la nourriture dans les maisons de retraite dans ces deux petits qu'généraliser le bénéfice de taux réduits de TVA à 5 5 à toutes les ventes d'équidés ainsi qu'aux prestations liées à ces animaux ne serait pas justifié ça poserait aussi des difficultés en termes d'équité à l'égard d'autres disciplines éducatives, sportives. Aussi dignes d'intérêt. Le gouvernement est attentif à la filière équestre, il apporte son soutien significatif à ses différentes composantes. Je rappelle que l'IFC eux que vous connaissez bien. Institut français du cheval et de l'équitation il par exemple aujourd'hui d'un budget de quasiment 43 millions d'euros au bénéfice de la filière équine. Ce qui témoigne de l'engagement constant et de la parole de l'État dans ce domaine. Les échanges entre le gouvernement et la filière sont sont approfondies sont réguliers. Et nous souhaitons vraiment qu'il le demeure, pour continuer à accompagner la filière dans le changement de doctrine européenne que vous avez souligné, Monsieur le Sénateur. Et surtout dans la valorisation des savoir-faire des pratiques des activités sportives et culturelles essentiel. Sans oublier le tourisme équestre, le tourisme équestre qui représente en France 1 million de pratiquants et qui permet une découverte inédite de notre Patrimoine de nos régions, je vous remercie et à Bercy, on se tient à votre disposition si vous souhaitez que nous poursuivions les échanges. Les dispositions actuelles sont insuffisantes car le contexte économique défavorable mais surtout la distorsion de concurrence entre pays en matière de fiscalité, de TVA pour la filière équine provoque l'annulation de certaines courses en France. Faute d'un nombre suffisant de partants et entraîne des pertes de recettes pour le PMU et donc pour la filière et pour le budget de l'État l'application de taux réduits de TVA conforme au caractère agricole de la filière et donc urgent. ça c'est pour les sénateurs, nous réaliserons notre photographie officier qui n'avait pu être prise en 2020 en raison de la crise sanitaire. Et je vous remercie de noter dans vos agendas, d'être présent. À 14h 20 précise dans l'hémicycle mercredi prochain. Je me permets d'insister sur l'horaire parce qu'un début. À compter du début de prise de vue qui doit être panoramique. Il ne sera plus possible d'entrer dans l'hémicycle et pratiquer l'injection de photos. À posteriori, n'est pas. La bonne formule. Je compte donc sur vous et nous allons nous retrouver. Tout à l'heure pour le débat. À partir de 16h 35 pour le débat d'actualité sur la crise du système de santé. Merci madame, la Première ministre, mesdames et messieurs les Ministres, la séance est suspendue.--

L'ordre du jour appelle le débat d'actualité sur le thème de la crise. Le système de santé, je rappelle dans ce débat. Que le gouvernement. À la faculté s'il le juge nécessaire de prendre la parole immédiatement après chaque orateur. Pour une durée maximum de 2 minutes. Orateur dispose alors à son tour à droite répartis. Pour une minute. Et le temps de réponse du gouvernement à l'issue du débat. Est au maximum de cinq minutes. Si vous le souhaitez. Madame la Ministre répondent après chaque orateur. Vous pourrez donc le le faire. Donc je donne immédiatement la parole. À notre collègue Patricia Schillinger pour le groupe du Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants. Monsieur le Président Madame la Ministre, mes chers collègues. Nous la souhaitons en masse les 1er janvier, nous trinquons étrangement d'ailleurs en son nom. Nous, nous nous rendons compte d'autant plus que de son importance depuis 3 ans. Nous savons à quel point elle nous est précieuse. Oui la santé, est et doit demeurer au coeur de nos politiques publiques car elle est au coeur de nos vies, nous l'avons dit mais je crois qu'il faut toujours le répéter et la triple épidémie à laquelle nous faisons face, nous le rappelle, les professionnels de santé sont cités certes tiennent à notre pays. Leur importance est connu de tous les, tous, et pourtant le constat demeure alarmant encore trop de Français sont sans médecin traitant et trop de professionnels de santé surmenés face à un flot de patients qui ne baisse pas encore trop. De nos concitoyens aux urgences, faute d'accès à un médecin de garde et trop des services d'urgences surchargées par des vagues de 2 nue non nécessaire face à cette situation inquiétante, je souhaite rappeler ici que de nombreuses mesures ont déjà été prises ne pouvons notamment rappelé les 19 milliards d'euros investis à travers le Ségur avec des revalorisations allant de 180 à 400 euros par mois également l'augmentation du nombre de places ouvertes ouvertes aux infirmiers et infirmières. La mission flash urgence répandant pour partie à la difficulté des services d'urgence le renforcement des champs de compétence de plusieurs de nos professionnels de santé ou encore la montée en puissance du parcours d'infirmières en pratique avancée. Ces mesures ont ainsi pu être des outils pour panser les plaies de notre système pour un temps, mais les mouvements de grève nous démontre qu'il reste encore beaucoup à faire. Plusieurs chantiers, nous attendent en effet et je souhaiterais ici m'arrêter sur l'un, de tout particulièrement l'enjeu de l'égal accès aux soins assurer cet égal accès aux soins sur l'ensemble de notre territoire nécessite de répondre à un double enjeu, permettre à chacun de nos concitoyens de pouvoir être soigné près de chez lui dès qu'il en ressent le besoin tout en répondant au surmenage de nos professionnels de santé, un travail d'équilibriste Jean course c'est ce sujet même qui avait motivé la rédaction d'un rapport avec mon collègue Philippe mouiller sur les collectivités à l'épreuve des déserts médicaux, l'innovation territoriale en action dans celui-ci, nous avions proposé des pistes de réflexion pour améliorer l'accès aux soins dans les territoires. Le tout avec le concours des collectivités territoriales, car elles sont évidemment central dans la mise en oeuvre d'une politique de santé ambitieuse, elles sont avec leurs élus parmi les premières à constater et subir les inégalités géographiques dans l'accès aux soins en dépit des moyens limités, dont elle dispose en matière de santé. Elles sont pourtant nombreuses à mettre en oeuvre des initiatives afin de répondre aux difficultés d'accès aux soins de leurs administrés, création de centres de santé ou des maisons de santé pluridisciplinaires, développement de la médecine ambulante ou encore de la télémédecine, les collectivités ne manquent pas d'imagination et de volonté pour apporter des solutions au problème, à l'accès aux soins. Plusieurs mesures présentées par le président lors de ses voeux bon dans ce sens, je pense notamment à l'amélioration des conditions de vie de nos soignants afin de renforcer l'attractivité de ces métiers, dans tous nos territoires je pense également à la suppression du plafond de 20% des télé consultation car sans être une solution unique. Ce nouveau mode de consultation représente un outil indiscutable indiscutable pour répondre à la pénurie de nos médecins et notamment de spécialistes dans certains de nos territoires je pense enfin à l'engagement pris de permettre aux 600.000 patients atteints de maladies chroniques, d'avoir un médecin traitant a tiré. Avant de la fin de l'année. Le président a également annoncé vouloir travailler sur les rendez-vous non honorés, je m'en félicite ayant présenté des amendements allant dans ce sens lors du dernier projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Le temps médical est précieux et il n'est pas juste que certains de nos concitoyens de le gâche en ne respectant pas les rendez vous pris renforcer le temps médical de nos médecins nécessite aussi de faciliter les différentes tâches administratives qui leur incombe, ou encore de leur apporter un soutien nécessaire face à ces mesures, un enjeu important d'importance perdure et je sais qu'il concentre toutes nos notre attention la permanence des soins. Je crois profondément heureux que pourront avoir les CPTS dans l'organisation de notre de cette dernière. Je crois également que les professionnels de santé ont leur rôle à jouer, afin de garantir à nos concitoyens, partout en France, un égal accès aux soins. Chaque fois qu'ils l'ont ils en Aucun Français ne devrait se sentir désemparés et seules pour protéger sa santé face à une pathologie ou face à l'imprévu. Des travaux sont en cours et je pense évidemment aux nombreuses discussions qui ont pu avoir lieu au sein du CNR de santé dans nos territoires le dialogue la Corée ordination et la collaboration sauront nous permettre de répondre au chantier qui s'ouvre à nous pour assurer cet madame la Ministre, suite au CNR santé et aux concertations, quelles sont les premières solutions que vous pourriez proposer pour assurer cet égal accès aux soins et notamment pour assurer la permanence des soins. Sur tous nos territoires. Je vous remercie. Merci ma chère collègue. Madame le Ministre de soutien. On va attendre que l'orateur. Et rejoint sa place. Madame la ministre.-- Monsieur le président. Tout d'abord mesdames et messieurs les sénatrices et les sénateurs, je tenais à Casino. Cette première première réponse de l'année vous présenter tous mes vous mon voeu et comme vous l'avez dit et madame la sénatrice. Une bonne santé, ça va un petit peu nous aider si nous pouvons tous en très bonne santé. Vous répondre en 2 minutes à la grande question que vous m'avez posé est assez. Difficile mais puisqu'il y aura l'occasion d'avoir plusieurs questions, je vais essayer de vous répondre. Au fur et à mesure de ce débat tout d'abord tout d'abord vous là, vous avez commencé par cela souligné la coordination nécessaire entre les collectivités, les soignants, les élus l'ARS. Et temps pour répondre aux besoins de santé de nos concitoyens de nos concitoyens, nous l'avons vu pendant la crise sanitaire à quel point les collectivités ont apporté. Leur aide nécessaire pour pouvoir notamment répondre à l'enjeu de la vaccination et cette coordination. Nous pensons qu'elle est nécessaire. Je suis Ministre de l'organisation territoriale et dans tous mes nombreux déplacements je vois à quel point la volonté des élus locaux de participer à l'organisation des soins à répondre aux besoins de santé de nos concitoyens est forte et la nouvelle méthode souhaitée par le président de la République, c'est celle-là, c'est avec les territoires à partir des territoires et ensemble que nous répondrons aux besoins de santé de nos concitoyens. C'était l'enjeu du CNR de conseil national de la refondation. Plus de 300 réunions ont eu lieu et nous sommes en train au ministère de le dernière réunion a eu lieu le 16 décembre et avec le ministre François Braun. Nous présenterons fin janvier début février, le résultat de ces consultations qui viendra complet qui viendront compléter les propositions faites par le président de la République le vendredi dernier lors de ses voeux aux acteurs de la santé, mais nous allons pouvoir ensemble répondre aux besoins de santé de nos concitoyens à la fois avec la refondation à l'hôpital mais aussi à la fois avec la refondation du système de ville parce que l'un ne marchera pas sans l'autre, c'est une absolue nécessité et l'enjeu est devant nous, mais ensemble nous allons-y arriver.-- Merci la parole est à notre collègue Bernard Jomier. Pour le groupe socialiste, écologiste et républicain.-- Monsieur le président, madame la miss. Mes chers collègues. J'imagine que si le président et le bureau du Sénat nous ont invité aujourd'hui à débat de sujet c'est évidemment eu égard à l'état de notre système de santé aujourd'hui. Beaucoup de Français. Beaucoup de nos compatriotes se demande comment il est possible que dans un pays qui consacrent 55% de ses moyens, à la dépense publique, plus 9 points en 20 ans la justice soit dans un tel état les infrastructures ferroviaires, soit dans un tel état et le système de santé que nous croyons jusqu'à quelques années, être le meilleur au monde est en train de s'effondrer à l'hôpital comme en ville.-- il faut fournir une réponse car si on ne fournit pas une réponse. On se trompe dans l'établissement du cadre politique de réponse.-- Quand on regarde cette dépense publique qui a progressé de 9 points en 20 ans. Ce qu'il a progressé, ce sont les transferts vers les ménages et vers les entreprises, c'est plus 10 points en 20 ans et le financement des services publics lui-même a régressé. Le financement des services publics dans la dépense publique ne représentent plus qu'un tiers de celle-ci et c'est là l'explication princeps de l'état actuel de nos services publics. Et la santé. N'a échappé que très partiellement. À cette évolution. Car si elle a bénéficié depuis les années 80 elle d'une hausse de 8% dans la part de dépenses. dans le même temps, par exemple, la population des plus de 60 ans qui génère l'essentiel de la dépense, elle, elle a progressé de plus de 30%. nous consacrons aujourd'hui en 2022 2023, moins de moyens. À la santé que nous en consacrions. À la fin du septennat de Valéry Giscard d'Estaing. Et quand vous prenez la rémunération des professionnels inclus ceux qui sont dans le privé, car il y a des acteurs privés, mais le financement, vous le savez très est essentiellement public hé bien la part allouée à la rémunération elle elle a baissé de 2% en part du PIB depuis 1995. Alors, Monsieur le président, mes chers collègues, nous pouvons.-- Entré dans tous les thèmes importants et tous les débats importants sur la gouvernance sur la répartition des tâches entre les uns et les autres sur la conception du système. Tous les points qu'Alain Milon a listé tout à l'heure d'ailleurs dans sa question d'actualité. Tant que nous resterons dans ce cadre général. Nous gérerons une pénurie. La maison France sous finance ses services publics depuis au moins 20 ans. Et ça n'a pas changé ces 6 dernières années. Ça continue puisque nous avons adopté un budget de la Sécurité sociale qui pour la première fois depuis que l'Ondam existe sera inférieur au niveau de l'inflation en progression. Ce sont des faits, ils sont incontestables. Alors malgré tout, il faut se pencher sur les différents chantiers. Et j'ai entendu, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt. Le chef de l'État. Il y a 6 ans j'étais comme un certain nombre d'entre vous à l'Élysée.

Les propositions portées par le chef de l'État sont les mêmes. 6 ans plus tard 6 ans de perdus. La réforme de la T2A, elle était déjà dans dans ma santé 2022. Elle est nécessaire, elle n'a pas été menée et l'épidémie de Covid n'explique pas tout, loin de là. Il y a donc une nécessité politique de dire que la santé est une politique première de notre pays santé le service public de santé c'est préserver au niveau de soins pour nos concitoyens et un égal accès aux soins et ensuite seulement on pourra discuter de ces différents thèmes et faire de sorte que ces discussions ne soit pas une gestion de pénurie mais impulser un nouvel élan à la politique de santé dans notre pays, je vous remercie. Madame la Ministre.-- Monsieur le président. Monsieur le sénateur, je vais essayer de, de répondre à votre, à votre question. Tout d'abord je vais. Permettre de vous rappeler 2 chiffres depuis 2017, le budget consacré à la santé a augmenté de 53 milliards pour être supérieur à 240 milliards, c'est 20% d'augmentation.

Vous avez raison. L'enjeu, l'enjeu qui est le nôtre, c'est à la fois de faire en sorte que ces moyens soient mis au bon endroit pour les bonnes personnes. C'est vraiment l'enjeu qui est le nôtre, l'objectif qui est le nôtre, c'est de fidéliser les soignants puisque nous savons très bien que par exemple à l'hôpital, ça n'est pas parce qu'il n'y a pas les moyens que Delhi ferme, c'est parce qu'il n'y a pas de personnel, donc l'enjeu c'est vraiment fidéliser les soignants, c'est rendre les métiers attractifs et notamment ce qui a été fait ce qu'il n'a, j'avais jamais été fait, c'est un rattrapage sur les salaires, vous l'avez souligné le Ségur a a permis une augmentation avec une enveloppe de 12 milliards pour les salaires des professionnels soignants de 19 milliards en investissements, en 2018, le président de la République avait clairement fait un diagnostic, ce qui n'a fait. vendredi dernier à Corbeil-Essonnes. C'est pas le diagnostic c'est la feuille de route, le cap qui nous est tracé, avec un objectif ambitieux et si la réforme de la T2A, n'a pas pu se faire depuis ma santé 2022 c'est que vous n'avez pas oublié qu'entre temps il y a eu la crise sanitaire et que les soignants avaient peut-être autre chose à faire et les administratifs et autre chose à faire qu'à réformer le système de financement de l'hôpital.-- J'ai donner l'apparence. Notre collègue Laurence Cohen pour le groupe communiste républicain citoyen. Et écologistes.-- Monsieur le Président Madame la Ministre, mes chers collègues. Vendredi dernier, le président de la République lors de la présentation de ses voeux aux personnels de santé a reconnu que notre système de santé connaissait une crise multifactoriel et qu'il fallait le réorganiser mais sans moyens supplémentaires. Ainsi, alors que l'hôpital est à l'agonie que la médecine de ville est en grande difficulté, aucun financement exceptionnel ne sera dégagé par le gouvernement, Emmanuel Macron a acté l'épuisement des soignantes et des soignants constaté que de nombreux patients n'ont plus de médecin traitant déploré que de plus en plus d'étudiantes et d'étudiants infirmiers abandonnent leurs études en cours de route autant de problèmes que nous avons dénoncés dans cet hémicycle sans que les ministres banc ne le prenne en compte et le président Macron continue dans la même veine prescrit les mêmes remèdes qui ont aggravé les maux de notre système de santé pour répondre à la grogne des médecins libéraux, notamment concernant le poids de leurs charges administratives, il la prime promis de créer 10.000 postes d'assistants médicaux d'ici fin 2024, mais sans instaurer une régulation à l'installation. Il a également misé sur une forme de récompense pour celles et ceux qui accepteront de prendre plus de nouveaux patients. Quant aux gardes de nuit et le week-end au lieu de revenir sur le décret. Qui a supprimé en 2002 l'obligation pour tous les médecins d'y participer. Il en est resté à des mesures d'incitation particulièrement inefficace. Je vous rappelle Madame la Ministre que notre groupe demande depuis des années à rétablir cette obligation de permanence pour les généralistes, mais également pour les spécialistes. Face aux nombreuses luttes en cours du côté des médecins libéraux et des hospitaliers des alertes de plus en plus forte avec la triple épidémie Covid bronchiolite et grippe ajoutant du désarroi et de la colère chez les soignants, on aurait pu espérer que les réponses du président change radicalement la donne. Alors que les personnels sont épuisés que toutes et tous se remettent en cause les conditions et la charge de travail qui entraînent des départs hospitalier en nombre, les 35 heures seraient à l'origine de la désorganisation de l'hôpital. pourquoi ne pas s'interroger Madame la Ministre sur le nombre d'embauches qui auraient dû accompagner cette baisse du temps de travail. Pensez-vous motiver les équipes au bout du rouleau en leur demandant de gérer la pénurie de personnel, les revendications sont sur la table depuis longtemps, revalorisation des carrières et augmentation des traitement indiciaire de la fonction publique. sur les fermetures de services d'établissement ainsi que sur les suppressions de lits depuis 2017 21.000 lits d'hospitalisation ont été supprimés, soit 5% des capacités d'accueil, mais surtout il y a urgence à mettre en place un plan de recrutement dans le service public hospitalier avec la création de 100.000 emplois comme le demandent les syndicats et les collectifs de défense de l'hôpital. Parallèlement, il faut revenir sur Parcoursup, supprimer le numerus apertus et augmenter les capacités de formation des universités et pour mieux articuler soins hospitaliers et soins de ville, il faut développer partout des centres de santé en leur donnant les moyens nécessaires. Madame la Ministre, mes chers collègues. Ce qui ressort des nombreuses auditions qu'on a pu faire à la commission des affaires sociales. C'est la déshumanisation de l'hôpital et les réside un hôpital entreprise aussi pour redonner de l'attractivité à l'hôpital. Faut-il redonner de la bientraitance institutionnel comme le souligne le Docteur Gérard Kierzek, Médecin urgentiste cela passe outre les améliorations des conditions de travail que j'ai déjà évoqué par la mise en oeuvre de la démocratie sanitaire ainsi la création d'un tandem administratif et médical est une mesure positive qui répond à une demande très forte des soignants hospitaliers mais il faut l'accompagner la suppression des pôles au profit des services du retour d'un conseil d'administration avec une meilleure représentation des personnels des élus mais aussi des usagers avec droit de véto sur le budget et aussi. Droit de véto sur le projet d'établissement. Alors bien sûr qu'il faut rompre avec la T2A. Mais l'essentiel est d'arrêter de faire voter un budget de la Sécurité sociale insuffisant chaque année car les conséquences nous les vivons dans la dégradation quotidienne de l'offre de soins pour toutes et tous sur l'ensemble du territoire. En conclusion, madame la Ministre, je voudrais vous poser la question suivante, allez-vous enfin financer l'assurance maladie à la hauteur des besoins. Donc augmenter les recettes, au lieu de réduire les dépenses, mettant à mal l'hôpital et la médecine de ville. Merci. Madame la Ministre.-- Monsieur le président, madame la sénatrice. Ah oui vous avez raison, la crise est multifactoriel. C'est bien pour ça qu'il nous faut absolument refonder notre système de santé et quand je dis refonder notre système de santé, c'est à la fois travailler sur l'hôpital mais aussi sur la ville on marque on arrivera pas à faire en sorte que tout à faire en sorte que tout aille bien, sinon on ne travaille que sur une des jambes. Il nous faut absolument travailler sur à la fois la ville et à la fois sur l'hôpital. Je vous le redis, 20% d'augmentation du budget consacré à la santé depuis du 2017 12 milliards. Pour l'augmentation des salaires, qu'il ne s'agissait que d'un rattrapage, nous en sommes convenus 19 milliards d'investissements. Décréter qu'il faille embaucher 100.000 personnes. Oui, je vais vous donner un chiffre, l'AP-HP en 2000 en 2022, a embauché 2200 infirmières.-- Entre temps, 2800 sont partis.-- l'enjeu, je le redis, il est à la fois de mettre en oeuvre tous les moyens pour fidéliser les personnels en place et de rendre le métier attractif comment fidéliser le personnel en place. Vous l'avez dit, tout d'abord ce rattrapage sur les salaires qui a eu lieu cette qualité de vie au travail qu'il nous faut travailler retravailler et co-construire ça passe aussi pour, comme l'a dit le président de la République refaire à l'échelle des services les emplois du temps et redonner du sens c'est permettra. Aux soignants de rester dans le même service de ne pas aller peut-être comme certains le pensent ils disent boucher les trous dans le service d'à côté mais c'est aussi arrêter cette spirale négative et réussir collectivement aussi à dire que ce sont des beaux métiers. Ovi envie aux jeunes de s'engager dans ces métiers de la santé, nous le savons tous aussi qui sont des beaux métiers et on leur donnera envie que si aussi on a un moment collectivement, on arrive à en parler. et puis je le rappelle que notamment en ce qui concerne les indemnités de nuit, elles sont prolongés dans le cadre de la mission d'urgence, qui avait été fait. Cet été.-- Donc Cohen. Réagir. Oui, oui, monsieur le président. Je vous remercie, madame la ministre. Mais si vous faites tout, si bien que ça. Eh bien, notre système de santé ne serait pas dans l'état dans lequel il est et puis on va parler chiffres, excusez-moi mais c'est 1,7 milliards de moins pour le budget de de de la la santé c'est ça la réalité, c'est ça que vous avez fait voter et quand vous parlez de l'argent, mais l'argent il existe. Simplement, ce sont les choix politiques que vous faites pas il y a 70 milliards en moins dans les caisses de la Sécurité sociale, du fait d'exonération de la, de, des cotisations patronales. Hé bien si là-donc il faut puiser parce que ça n'est pas créateur d'emplois, ça n'est pas vrai. dire les besoins au réflexe hors inflation sont estimés à 10 milliards d'euros supplémentaires pour la santé. Donc vous voyez je vous donne des recettes d'un côté 70 milliards de l'autre côté 10 milliards mais vous ne voulez pas faire ce choix là et vous êtes en train de mettre notre système de santé à à genoux et il y a des personnels qui sont en souffrance et qui ne se satisfont pas de vos paroles regarder tous les mouvements qui se développent partout.

Monsieur le Président Madame la Ministre, chers collègues, l'importance du sujet de notre débat m'invite à commencer mes propos par une citation de William retour le pessimiste se plaint du vent l'optimiste c'est espère qu'il va changer et le réalisme ajuste ses voiles. Crise des urgences tensions générées par la triple épidémie du Covid grippe et bon colite déprogrammation de soins médicaux déficit criant de personnel hospitalier postes vacants démission soignant le burn-out, la liste des notes. De cette triste mélodie hé bien longue. La session de l'hôpital continue d'inquiéter dans un contexte où la demande augmente du fait du vieillissement de la population, nos services publics d'urgence connaissent des sous-effectifs chroniques et reste sous tension pour faire face à un afflux important de patients. Cette situation inadmissible qui continue à se dégrader depuis l'été 2022 et le révélateur de la crise profonde qui traversent notre système de santé et témoigne du poids important de l'hôpital en particulier l'hôpital public dans la prise en charge des urgences l'engorgement des urgences résulte d'une conjonction d'éléments défavorables. D'abord l'accès à une consultation c'est d'un médecin généraliste devient de plus en plus compliqué, dans un délai raisonnable. La question du temps médical disponible continuera de s'aggraver avec la croissance des départs en retraite non remplacés. Ensuite les praticiens ne s'installe pas de façon géographiquement harmonieuse, le problème des déserts médicaux et récurrent non seulement secteur rural outre-mer mais aussi en zone urbaine. Enfin, il existe un déficit d'information sur la conduite à tenir en cas de problème de santé ainsi de nombreux patients qui se rendent aux urgences de leur propre chef le Fonds faute d'une meilleure orientation il importe pardon de mettre en place des mesures alternatives pour accueillir des soins non programmés, afin de répondre aux besoins des patients pour un mal qui ne relèvent pas de l'urgence vitale comme la petite bobologie, il serait aussi pertinent d'inciter les médecins de ville installés dans des maisons de santé de maintenir une permanence particulièrement les week-end afin de pouvoir désengorger les urgences. Néanmoins, ce dispositif ne peut être imposée au niveau national tant les situations sont différentes d'une région à une autre. En revanche, les agences régionales de santé peuvent jouer un rôle moteur dans différentes expérimentations je met cependant en garde à trop de m'attendre. La voix de l'obligation de garde finira par s'imposer. Au-delà des adaptations du terrain s'avère nécessaire une meilleure coordination des soins, un meilleur partage des compétences, une meilleure répartition du pouvoir de décision et des responsabilités entre médecine de ville et hospitalisations. Augmentation des capacités d'accueil en médecine de ville accompagnement au travail collectif, développement de la télémédecine, de manière bien encadré et bien évidemment, amélioration de qualité de vie au travail, réduction des pertes de temps dans les démarches administratives sont d'autres pistes de réflexion. La pénurie de soignants d'infirmiers et de médecins risque de s'installer dans la durée. Force est de constater que l'augmentation des salaires prévue dans le cadre du Ségur de la santé n'a pas entraîné une nette évolution des recrutements afin de résoudre le problème de ressources humaines en santé. Il est essentiel d'établir un plan pluriannuel, mais chers collègues face à cette crise, aucune solution simple n'existe. Mais pour reprendre les mots de Winston Churchill, mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne vous prenne par la gorge. Je crois que c'est fait. Madame la Ministre notre retard et significatif n'attendons plus alors que plus de 6 millions de Français n'ont pas de médecin traitant une transformation ambitieuse notre système ça pose celle-ci nécessite l'engagement de toutes les professions de santé dans une démarche collaborative pour améliorer l'accès aux soins et garantir la qualité des pratiques à l'aube de cette nouvelle année oh construisons ensemble notre système de santé avec mes collègues du groupe Union centriste, je souhaiterais savoir Madame la Ministre votre vision réformatrice, ainsi que le plan d'action du gouvernement en matière de prévention, de gestion de crise pour répondre dans l'urgence au défi auquel est confrontée l'ensemble de notre système de santé. Avec ses 2 piliers. Le public et le privé. Je vous remercie de votre attention. Et. Merci ma chère collègue. Madame la Ministre.-- Merci monsieur le président, madame la sénatrice 87% de la France est un désert médical. L'hôpital ne va pas bien et c'est bien pour ça, je le redis, je pense que je vais le redire a encore beaucoup de fois qu'il est nécessaire, et vous l'avez souligné, de refonder notre système de santé à la fois sur la ville et sur l'hôpital mais à la fois travailler sur la coordination public-privé. Et vous avez bien fait de le souligner. Je suis maintenant depuis. 6 mois j'ai à peu près fait 40 déplacements et des gros déplacement. Je peux vous assurer, est ce que vous avez dit est très juste, que nous ne pouvons pas appliquer la même méthode en Île-de-France qui est le plus grand désert médical que dans la Drôme où je suis allé récemment, donc c'est bien à partir des territoires avec les territoires que nous allons construire les réponses. Je suis raisonnablement optimiste parce que dans les territoires, nous voyons des solutions qui marchent et vraiment la volonté des professionnels la résilience des professionnels, il faut le souligner, de tous les professionnels durant, j'allais dire optimiste raisonnablement et va nous pouvons Avec la feuille de route établie par le président de la République avec les solutions qui seront issus du CNR de vous faire des propositions. Ce dont nous sommes convaincus c'est que il nous faut répartir répartir et c'est tout à fait vrai dans la permanence des soins, la tâche. Nous ne pouvons pas laisser à seulement quelques médecins de supporter de supporter la permanence des soins. Il nous faut construire sur le thème de la responsabilité collective du gagnant gagnant et c'est ce qui est en train d'être au frais, notamment dans la négociation collective avec les médecins, il nous faut répartir la charge de la permanence des soins c'est ce sur quoi nous sommes en train de travailler, c'est une des réponses que je peux apporter à vos nombreuses questions.-- Merci. Je vais donner maintenant la parole à. Monsieur Stéphane Ravier pour la réunion administrative dessinateur de figurant sur la liste d'aucun groupe. Le. Il y a 3 minutes. Vous avez la parole Monsieur le Président Madame la Ministre, mes chers collègues. Selon le préambule de la Constitution de 1946, La nation garantit à tous la protection de la santé, mais ça c'était avant pourtant depuis le début d'une présidence en marche. Les Français avaient reçu tant de promesses dès 2018, le président Macron présente un grand plan pour la santé appelé ma santé 2022 sans structuré notre système pour les 50 prochaines années. En 2020, Ségur de la santé en 2021, plan Innovation Santé 2030 et en 2022, c'est l'annonce brutale de la refondation. Un système que vous jugez à bout de souffle. Notre système de santé envié par le monde entier et qui a été saccagé en quelques années, car la réalité de votre politique. La voilà, 4300 lits fermés à l'hôpital public en 2021 5700, fermées au coeur de la pandémie en 2020. Au total, 21.000 lits supprimés en 5 ans qui viennent s'ajouter aux 10.000 lits fermés sous François Hollande 37.000, Sousse, Nicolas Sarkozy. Près de 100.000 lits fermés en 20 ans alors que notre population augmente que son vieillissement nécessite davantage de soins et donc de moyens les déserts médicaux touche la France rurale mais aussi une partie de la France urbaine et jusqu'à nos hôpitaux où nous trouvons porte Close aux urgences avec un système qui encourage à faire du chiffre, qui ne promeut plus la qualité de soins et sort le personnel soignant les images qui nous viennent de tous les hôpitaux de France sont déplorables, 150 patients seraient morts aux urgences, faute de prise en charge depuis début décembre. Je vais aussi vous dire, Madame le Ministre des milliers de soignants non-vaccinés viennent de passer leur 2ème fête de Noël suspendu, sans salaire et sans chômage. La France est le dernier pays européen à ne pas les avoir réintégré le dernier vous qui n'avait de cesse vous référer en toutes circonstances à nos voisins européens. Qu'attendez-vous pour les imiter. Je manque de temps pour évoquer les les pénuries enregistrées par l'Agence nationale de sécurité du médicament. Conséquences de notre dépendance de la production étrangère, alors en ce début d'année. Où nous échangeons des voeux de bonne santé et je vous les adresses bien sincèrement Madame le Ministre quelles sont les actions concrètes engagées déjà par votre gouvernement destiné à creuser des oasis nécessaires au milieu de ce désert médical national. Madame la Ministre.-- Merci monsieur le président, monsieur sénateur.-- Une réponse. Vous avez parlé beaucoup d'Europe. Juste vous dire que, puisque vous regardez ce qui passe ce qui se passe à côté ben regardez dans quel état sont les systèmes de santé de nos pays européens, le manque de professionnels et mondial. Le manque de professionnels et mondial. On ne peut pas se satisfaire de cette réponse. Mais on ne peut pas dire non plus que l'herbe est plus verte à côté, regardez ce qui se passe en grande robe Bretagne. Regardez ce qui se passe en Allemagne, regardez ce qui se passe en Espagne et même aux États-Unis. Le manque de professionnels de santé et mondial. Il nous faut pour notre pays, trouver les moyens c'est ce que nous faisons et c'est ce que nous allons faire avec la feuille de route qui nous a été tracée par le président de la République. Monsieur Ravier vous vouliez réintervenir.-- Oui oui oui mais si Monsieur le Président, simplement, écoutez madame le Ministre, moi j'avoue être humble. Je suis sénateur français et c'est le système. Médical qui français qui m'intéresse ce sont nos compatriotes qui m'intéresse et je ne me contente pas de me dire que ailleurs c'est pire, pour justifier la la situation qui est la nôtre et qui est le résultat Direct des politiques et qui ont été menées par les, les gouvernements français un peu d'audace, un peu je dirais de réflexion un peu d'autonomie. Pour. Que les idées franco-française puisse permettre à notre système de santé d'évoluer dans une situation vers

vous avez la parole.-- C'est bien simple, trop de nos concitoyens ruraux en particulier ne trouve plus de médecins de ville et les médecins restant d'un peu plus. C'est tout le système de santé, qui doit donc se réinventer avec l'investissement de tous à la mesure de ses moyens et la responsabilité de chacun. Le président de la République a évoqué lors de ses voeux au personnel soignant quelques pistes d'action. Dans certaines mérite d'être précisée, parfois ce qui à Paris une bonne idée peut s'avérer complexe. Un exemple, celui de 600.000 malade chronique, un malade chronique peut avoir du diabète une entorse au pied et ou une dépression. Pas de chance, me direz-vous mais ou devra-t-il s'adresser car le médecin de ville et la personne à qui on parle de tout. Vous me permettez un effet d'adopter un point de vue, celui du patient qui cherche qui parfois peur et qui doit être aiguillé parce que ce n'est pas son métier. À ce titre le prêt adressage est essentielle. Nous souhaitons sur douter rapidement les cendres 15 et 8 18 dans chaque département. Nous demandons la mise en oeuvre rapide des plateformes de services d'accès aux soins prévue pour orienter convenablement les patients dans une logique depuis Nous pensons utile de généraliser des plateaux techniques avaient des infirmiers de pratique avancée permettant d'effectuer de la bobologie qu'cela est utile ou de prix adressée aux urgences avait des examens déjà fait le président de la République a évoqué un dos d'un pour établir des permanences de santé quand une consultation mieux rémunérer. Des maisons médicales de garde ouverte le week-end serait pour nous un objectif prioritaire. Les plateformes SaaS pourrait être dispose déjà disposer de créneaux de réservation de rendez-vous des médecins de ville de kiné ou des infirmiers. Nous souhaitons un retour que les rendez-vous non honorés soient sanctionnés qu'un l'abus est manifeste parce que ces créneaux sont des trésors. Nous avons besoin d'une réelle régulation publique décentralisée et pluridisciplinaire. Où concentrer nos efforts pour le moyen terme dans les territoires avec les acteurs locaux et ce dès le début de la semaine aura été supérieur de même que nous avons constaté que les plus jeunes médecins et infirmiers souhaitez pratiquer la médecine hein collégialité il faut je le crois, proposer la même chose à un autre étudiant nous déplorons tous ensemble que les jeunes médecins s'installent ailleurs que dans nos territoires ruraux ou sous-. Mais c'est oublier que la cassure territoriale se fait dès le premier stage d'internat. Nous proposons ainsi la création de lycées médicaux ou d'options médicales sur le modèle de lycée agricole. Nous croyons également nécessaire de réintroduire un entretien pour les inscriptions en école d'infirmiers et facultés de médecine pour éviter les abandons trop nombreux mais aussi de permettre le redoublement de première année pour éviter des fuites à l'étranger. Nous proposons l'agrandissement des IFSI et la création de petits centres universitaires médicaux décentralisé dans des villes moyennes adossés à des logements ainsi les étudiants en médecine insupportablement sous- payés pour en découvrir avec leurs amis de la réalité de nos territoires dans une démarche contractualiser ils n'auront plus à s'inquiéter de trouver un toit ni cherché à revendre leurs tours de garde à des camarades plus riche pour assurer leur subsistance. Les collectivités locales sont prêtes, les. Alpes-de-Haute-Provence, ils sont prêtes, car nous savons que soignants un devenir ou un plat c'est précieux. Ce qui me permet d'en venir à mon dernier point nos territoires sous-dotés enduit investir d'un des médecins intérimaires hospitaliers parce que rien ne marchait. Nous ne cautionnons pas ces pratiques mais il faut cependant faire avec l'existant. Le Conseil constitutionnel a censuré une disposition du projet de loi de finances de la Sécurité sociale limitant le recours, tandis que la loi risque prévoyez une restriction d'emploi au cours de cette année. Le flou profite déjà aux intérimaires qui effectuent des listes d'établissements à septembre c'est pratique et il est bien évident que nos établissements publics hospitaliers ne pourront pas s'aligner Madame la Ministre comment nos hôpitaux déjà exsangues pourraient-ils tenir. S'ils sont désertés. Du jour au lendemain par ces intérimaires ne pourrions-nous pas créer dans ces cas précis des postes fixes dans les structures concernées, je vous remercie de votre attention.-- Madame la ministre. Monsieur le président, monsieur le sénateur, vous avez essayé, vous m'avez posé beaucoup de questions, je vais répondre. Essayer de répondre à quelques-unes concernant les 657.000 de nos concitoyens sous ALD c'est-à-dire qu'ils sont suivi pour une pathologie chronique c'est l'urgence. Il nous faut répondre collectivement avec les médecins et pouvoirs. Et le cap a été fixé par le président de la République avant la fin de l'année que chaque patient sous ALD et accès à un médecin traitant. Ce travail, il va être fait avec la Caisse nationale d'assurance maladie où nous allons très vite pouvoir appeler chaque patient patient sous ALD et le mettre en contact avec un médecin traitant. Nous sommes dans la logique du gagnant-gagnant et les médecins sont les premiers j'allais dire concerné et ils veulent absolument nous accompagner pour pouvoir répondre à cette, j'allais dire nécessité puisque, en passant sous ALD qu'on pense par exemple sur la dette. On va le retrouver aux urgences, donc il nous faut travailler très vite sur ce sujet, nous avons déjà eu l'occasion de l'évoquer ici. La réforme, j'allais dire L'évolution. De du parcours de de formation de nos infirmiers et de nos infirmières et nécessaire, nous le savons, un taux de fuite en première année de 30 120% à la fin ça veut dire que 50% de nos jeunes qui rentrent dans le processus de formation pour être infirmier ou infirmière ne vont pas au bout. Ça veut dire qu'il y a un problème. Le rapport IGAS sur ce point est très clair, et nous allons très vite là aussi pouvoir faire des propositions pour. éviter éviter cet écueil sur les rendez-vous non honorés, là aussi, nous pourrons tous apporter des mesures si nos concitoyens aussi ne nous aide pas hein. C'est-à-dire les besoins de santé ne sont pas des, des besoins de consommation comme un bien de consommation comme un autre. Je prends un rendez vous, je le respecte, car si je ne vais pas ce rendez-vous. C'est quelqu'un d'autre qui n'a pas pu être prise en charge. Donc nous allons travailler et faire des propositions sur les rendez-vous non honorés. Sur les packs avec les collectivités. Souhaitée par le président de la République, il est nécessaire et là aussi mais nombreux déplacements montre à quel point l'investissement des collectivités pour rendre le territoire attractif pour accueillir, soit des jeunes internes, soit des jeunes médecins est intéressant. Je vais citer la maison des internes. La Maison des internes à Morteau. C'est un bel exemple de ce travail de coconstruction entre les collectivités, les ARS et les soignants, pour permettre aux jeunes de venir découvrir le milieu rural ou semi-rurbains et de pouvoir peut-être vouloir s'y installer, enfin sur l'intérim. Vous savez que nous avons pris la décision de la mettre en application à partir du mois de mars. Cette loi est votée, il faut la mettre en application. Nous avons avec les ARS avec les hôpitaux fait ce chemin les ARS sont prévenus. Mais bien sûr, il nous faut trouver est pour les personnels.--

Monsieur le Président Madame la Ministre, mes chers collègues. Lors de ses voeux aux acteurs du secteur, le président de la République a tenté de dresser un nouveau cap. Pour la santé dans notre pays. Ce cap était nécessaire et attendu après 3 ans d'une pandémie qui a épuisé les soignants et continue encore de les mobiliser au quotidien, il se devait d'aller au-delà d'une sorte de rediffusion de ma santé 2022 voire d'un auto-satisfecit presque gênant. Le constat dressé par le président de la République a largement connu et partager les annonces en revanche manque de contenu et de crédibilité concrète au service de la santé des Françaises et des Français. La médecine de ville en crise tiraillée entre des besoins plus importants de la population. Des déserts médicaux entre guillemets toujours plus préoccupant et des professionnels de santé qui en nombre insuffisant, peine à dégager le temps médical nécessaire. Face à cela, nous avons eu droit au catalogue des annonces relatives au système de santé des 5 dernières années. Quelle signification concrète pour la solidarité collective les revalorisations différencier la valorisation de l'exercice coordonné. Certes, ce n'est pas simplement une question de moyens mais nous sommes au milieu d'une négociation conventionnelle particulièrement tendue. D'un seul coup le seuil de 20% des consultations ne serait plus pertinent. Mais quelle médecine. Voulons-nous une médecine sans examens cliniques pratiquaient dans des centres d'appels éloignée des populations une médecine qui pourrait devenir une médecine à 2 vitesses vit dans un peu plus encore les territoires. La télémédecine un outil complémentaire mais ne doit pas être un substitut ubérisés à une médecine de qualité. Il faut embaucher davantage de mais d'assistants médicaux, nous dit le président soit mais pour ce qui est du financement, aucune précision. Bien sûr, le président de la République s'est aussi prononcé sur la délégation date estimant qu'il fallait qu'elle soit je cite simplifier généralisée et qu'il n'y ait pas de conflit entre les professions. Quels sont les choix concrets traduit par cette formule sibylline que veut dire concrètement apporter une solution de santé en incitant les acteurs de santé à coopérer à quid par exemple des infirmiers en pratique avancée à peine cité par le président. Au chapitre des solutions simples. Le président de la République a annoncé concernant les 6 millions de Français sans médecin traitant que les 600.000 malades chroniques qui n'en disposent pas s'enverrait prochainement proposer un parle c'est Caisse nationale d'assurance maladie et on se demande pourquoi cette annonce n'est pas venu plus tôt mais surtout se poser la question du nombre de France à son médecin traitant une chose se demander le rôle de ce dernier, aujourd'hui dans le système de soins en est une autre. Or sur cette seconde question. Nous n'avons pas vu de vision portées par l'exécutif. Le médecin traitant doit être la porte d'entrée mais pas le verrou de notre système en disant cela. Certes on ne fâche personne mais on ne résout aucun problème. Quelle est la feuille de route. Poursuivi par la multiplication désordonnée des accès directs comment ces derniers sont-ils justifiés mais en cohérence au delà d'être la porte d'entrée. Comment donner réellement médecin traitant les moyens d'être le pivot en Suède où s'est rendue la commission des affaires sociales. Le rôle du médecin traitant n'est pas la régulation et c'est souvent infirmier mais bien le diagnostic médical et la coordination des soins, mais est-ce le choix qui nous est annoncé. Du côté de l'hôpital dans une crise tout aussi profonde et durera malheureusement le discours présidentiel n'était pas beaucoup plus claire. Bien sûr l'annonce choc relative à la tarification à l'activité beaucoup couler beaucoup dans, derrière ce slogan d'une femme de la T2A. Le président de la République n'a fait que reprendre ce que la commission d'enquête du Sénat appelait de ses voeux l'an dernier un modèle de financement mixte, avec une part de dotation que l'on appelle communément populationnelle un financement lié à la qualité et bien sûr une part demeurant assis sur l'activité. Cette annonce ne suffira pas à rassurer les professionnels de santé. Car répétons-le, le problème de la T2A n'est pas de lier le financement l'activité mais bien d'appliquer un tarif qui ne couvre pas réellement les charges des établissements et se tromper de problème ça apporté une mauvaise solution. Par surcroît, on nous dit aujourd'hui qu'il n'y aura pas de transition avec le nouveau modèle sera votée dès le PLFSS 2024. Mais que de promesses quand nous voyons que le gouvernement n'a même pas conduit l'expérimentation d'un tel modèle financement pourtant voté en LFSS. Pour 2021 et que les réformes du financement des soins de suite ou la psychiatrie jamais passés à la tête de ça ne sont toujours pas effective. J'aimerai pour ma part que le gouvernement nous fasse l'exigeait du verbe précis une présidentielle quand il le programme on doit sortir la tarification à l'activité dès le prochain projet de loi de financement de la Sécurité sociale tout en annonçant plus loin une part de rémunération à l'activité qui est légitime et qui doit continuer. Surtout en évoquant un changement de modèle de financement. Le président Macron évites précautionneusement le sujet de la dépense et de sa régulation alors que l'on nous annonce des revues de dépenses et que la maîtrise de la dépense publique est une nécessité. Quelle par le gouvernement veut-t-il consacré réellement à l'hôpital car Madame si le nouveau modèle de financement n'est qu'une nouvelle règle de partage du même du même gâteau et qu'on nous ils ont nous des débats techniques et gardons le système actuel, le premier engagement, qu'il faut prendre à l'égard de l'hôpital, c'est celui de l'humilité. La commission d'enquête sur l'hôpital avait choisi de ne pas appeler à une nouvelle loi santé comme elle avait revendiqué de ne pas réengager de modification de la gouvernance, estimant que le cadre issu des réflexions du professeur Clarisse là c'est bien de la souplesse pour revaloriser le service d'une part et pour médicaliser la direction de l'autre. Donc, cessons d'annoncer des fausses révolutions des changements par Reading en trompe-l'oeil. Le vrai besoin des soignants. Aujourd'hui ce sont les effectifs. Où en sont les recrutements comment les hôpitaux sont-ils en capacité de renouer avec l'attractivité des postes des carrières et en capacité de financer davantage de soignants au lit des patients. C'est cela la réalité des prix Madame la Ministre et c'est cela la réalité de la politique que vous avez amené la feuille. De euros donné par le président de la République ne permet de déceler aucune ambition concrète pour les soignants et le système de santé qui le porte et je le crains n'annonce aucune politique structurée de la part du gouvernement face à la crise que nous connaissons. Vous l'avez compris, mes chers collègues, cette année 2023 commence par des annonces qui n'en sont pas pour des réalisations dont je crains qu'elle n'en sort pas et je dirais des mots, toujours des mots, les mêmes mots, rien que des mots, je vous remercie je vous souhaite néanmoins madame la ministre, une excellente année 2023.-- Merci madame la présidente. Madame la Ministre.---- Monsieur le président, madame la sénatrice. Alors je vais essayer par des mots mais qui seront suivies d'actes de vous convaincre. Tout d'abord sur les assistants médicaux, vous savez que l'objectif qui est celui du gouvernement, c'est bien de passer de 4000 à 10.000 assistants médicaux parce que un assistant médical, c'est 15% de temps médical gagner et donc 15%. Que le médecin généraliste pour un. Consacré. Au suivi d'un patient et prendre de nouveaux patients sur le financement, il faut être très clair, le financement il est annoncé ses 36.000 euros la première année, 27.000 euros la deuxième année 21.000 euros à partir de la troisième année. C'est-à-dire que le financement combien. Hé bien assuré après la troisième année. Le médecin traitant doit rester la Pierre angulaire de notre système de santé, le président de la République l'a clairement dit, c'est une volonté. Affichée et que nous assumons, il peut être le chef d'orchestre et ne sera pas leur mort Crest. Je crois que le président de la République là aussi dis donc vous l'avez forcément aussi bien noté mais quand tu le président de la République dit qu'il dote pas être le verrou. Ça veut dire que puisque nous avons 6 milliards de 6 millions de nos concitoyens qui n'ont pas de médecin traitant d'autres professionnels pourrait être la porte d'entrée pour amener ces patients vers. Un médecin traitant sur la télé consultation. Vous savez que la crise sanitaire a été. J'allais dire un accélérateur de l'usage de la téléconsultation. Nous avons presque gagné 15 ans sur le développement de la téléconsultation néanmoins lorsque le président de la République parle de ces 20%, ça n'est pas déréguler le système mais c'est prendre en compte que dans certaines spécialités, les 20% sont bloquants. Je pense notamment à la psychiatrie. On voit bien que l'usage de la téléconsultation pour la psychiatrie. Les 20% sont mi-temps donc c'est bien, ça n'est pas déréguler le système mais faire en sorte que on l'utilise au mieux pour certaines spécialités, mais aussi j'allais dire comme et nous partageons la même analyse. C'est un complément, et dans certains territoires, l'usage de la téléconsultation peut être. Intéressante, c'est bien l'objectif qui est fixé. Le président de la République n'a pas annoncé la suppression totale de la T2A, je vous le redis, c'était dans la feuille de route de 2018, nous le savons. Je le redis, qu'il était impossible de réformer le financement de l'hôpital avec la crise sanitaire que nous avons traversé dès 2020 mais que l'objet c'est bien de construire avec les

mais aussi de pertinence des soins, comment on évite certaines dépenses. Monsieur le sénateur millions le l'a évoqué tout à l'heure, donc tout ça est co-construire sans sortir complètement de la T2A puisque nous savons que une part de la T2A pourra être conservé et la réforme de pas être mises en place dès le PLFSS mais là puisque vous avez été aussi bien bien attentive au discours. Nous allons commencer le chantier dès le PLFSS 2024.--

Monsieur le Président Madame la Ministre, mes chers collègues, je voudrais tout d'abord saluer le travail des soignants.

la pandémie en a révélé et aggravé les contraintes qui pèsent sur notre système ceci malgré n'augmentation importante de l'Ondam 4% cette année, 57 milliards depuis 2017. Nous sommes maintenant un tourment. Nous ne pouvons plus laisser de notre système de santé se dégrader davantage. Et avec vous, madame la ministre, de nous devons trouver des solutions pour remédier à la situation. À la croisée des nombreuses difficultés que qu'on est que connaît notre système se trouve les systèmes d'urgence. Leur état d'engorgement est alarmant. Et mon propos ira dans ce sens alors que l'État doit pouvoir apporter des soins sur l'ensemble du territoire des urgences sont aujourd'hui devenus le dernier rempart médical pour un homme. Importante de nos concitoyens. Il est cependant essentiel que ses services reste focalisé sur les cas graves et pas être symbolisée par simplement des soins non programmés, qui n'ont pas trouvé de médecins. Pour qu'ils puissent accomplir au mieux leur mission. Les services d'urgence doivent être tout d'abord préserver en amont par une régulation efficace en Corrèze. 10% de plus de personnes sont allées aux urgences en 2022 après un doux après un doublement depuis 20 ans. La régulation doit permettre de distinguer ce qui relève de l'urgence et ceux qui n'en relève pas. Une bonne régulation doit aussi réorienter. À cet égard, il me semble indispensable que les médecins de ville qui auront à leur disposition des IPA qui auront des assistants médicaux cela pour libérer le temps de travail accepte de réaliser davantage de soins non programmés, notamment ceux qui ont et auront été réorientées depuis le. Les services d'accès aux soins qui sont à côté du médecin régulateur ces soins. Pourrait être assuré effectivement dans le cadre d'une CPTS communautés professionnelles de territoire et de la santé, avec des maisons de santé pouvant à tour de rôle de garde pour prendre en charge les soins non programmés. Il convient également. De soulager les services d'urgence en aval une fois la situation médicale du patient stabilisé, il faut le transférer hors des urgences. Alors là le problème arrive les fréquent que dans les autres services hospitaliers devenu hyper spécialisés refusent d'accueillir un patient qui ne relève pas de leur spécialité, les services d'urgence n'ont pourtant pas d'autre moyen. De conserver ses patients sans mettre en péril l'exercice de leur mission. Il faudrait mettre en place des services de soins polyvalent en aval destiné à accueillir des patients qui doivent être hospitalisés pour cela Madame le ministre. Il faut trouver les moyens de rouvrir des lits beaucoup de lits ont été fermés pour cause de manque de personnel. Ces dernières années. Pour les médecins. La suppression du numerus clausus bon j'en parle pas. Ce sera seulement après 2030. Mais actuellement, on peut faire des choses pour les avoir pour créer des davantage d'infirmières et d'aides-soignantes d'ailleurs ce besoin de ne fera que croître avec le temps. Au fur et à mesure que la population ne viendra plus dépendants, notamment en augmentant entre 2020 et 2030, la prévention sera nécessaire, mais aussi la prise en charge de nos aînés et actuellement la prise en charge est minuté dans les Ehpads et ça décourage des soignants. Le plan grand âge doit se mettre en place rapidement avec les 50.000 emplois annoncés par le ministre monsieur comme Il faut aussi un plan massif de formation, la validation des acquis de l'expérience semble une être une bonne piste. D'autre part, depuis le PLFSS les étudiants devront effectuer une 4ème année d'internat auprès de maître de stage il y en a pas partout et je suggère que les six derniers mois puisse réaliser auprès de médecin référent pour irriguer tous les territoires. Le médecin référent. Connaît bien la potentielle pâtissier en telle est tout à fait aptes à conseiller et orienter d'autre part, médecin dixième année qui a passé. qui en dixième année qui est aisé médecin enseignant doit être payé comme remplaçant, c'est-à-dire des consultations par jour maximum. Donc le défi que nous devons relever sont nombreux. Madame le Ministre ensemble le plus rapidement possible. Résoudre les problèmes en amont et en aval des urgences et embaucher massivement des infirmières et des aides-soignantes. Cela pour effectivement prendre en charge. La. Les le personne les personnes. un aménagement de la 4ème année et tout est obligatoire pour moi pour irriguer tout le territoire mais aussi bien sûr comme ça a été dit, aider les collectivités à embaucher des médecins salariés et aussi la téléconsultation peut aussi apporter quelques services merci. Merci.

Madame la Ministre.-- Au service de notre système de santé. Je partage pleinement la nécessité de bien assurer la gradation dans le recours aux différents niveaux. C'est par défaut que les services d'urgence sont aujourd'hui trop souvent la seule solution identifiée par nos concitoyens. Le manque de médecins en ville, en est sans doute le meilleur des exemples le déploiement du service d'accès aux soins sera une vraie solution pourrait orienter en cas d'indisponibilité de son médecin traitant vers une solution de soins non programmés à son état de santé. C'est clairement ce qui nous allons faire puisque les services d'accès aux soins à part après avoir été mis en place cet été dans le cadre de la mission d'urgence seront développés et apporte une vraie réponse en amont des urgences, nous sommes résolument engagés pour soutenir les services de régulation avec un plan massif pour attirer des candidats et former des assistants de régulation médicale mais aussi pour le médecin régulateur de nous avons déjà revalorisé financièrement la mission depuis l'été 2022. Vous avez raison, il nous faut aussi agir en aval des urgences pour fluidifier les parcours pour cela nous avons réactiver les cellules de gestion territoriale délits qui ont fait leurs preuves durant la crise sanitaire et permettent une vision complète des capacités de l'ensemble des établissements d'un territoire. Nous avons aussi autorisé face aux tensions induites par la triple épidémie des mesures dérogatoires pour avoir davantage de véhicules en charge de réaliser des transports, avec la possibilité que l'assurance maladie rembourse des trajets de. En sortie des services d'urgence ou que des équipages d'auxiliaire ambulancier assurent des transports ne nécessitant pas de surveillance médicale. La clé vous le soulignez réside dans les ressources humaines, qu'il s'agisse de former de nouveaux professionnels ou de convaincre ceux qui ont quitté le système de revenir ce sont tous les enjeux d'attractivité et de prise en compte de la pénibilité, que nous sommes en train de travailler actuellement et qui doivent pouvoir produire des effets très rapidement.-- Merci. Je vais appeler Madame, Mélanie Vogel. Pour le groupe écologiste solidarité et territoires. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre chers collègues nous débattons aujourd'hui du thème, la crise du système de santé et je crains malheureusement que cette question soit déjà obsolète. Notre système de santé n'est plus en crise, une crise s'est soudain une crise c'est brusquer momentanée et puis une crise ça passe. Notre système de santé n'est plus en crise. Notre système de santé n'est même plus au bord de l'effondrement. Notre système de santé s'effondre sous nos yeux. Qui aurait pu le prévoir. Eh bien toute personne s'étant renseigné sur le sujet aurait pu le prévoir. Car si notre système de santé s'effondre. C'est la conséquence mécanique logique et implacable de choix politiques politiques de mauvais choix politiques qui ont déjà coûté des vies, des vies parmi comme toujours les plus précaires et qui maltraite chaque jour des soignantes et des soignants. 36 des 38 infirmiers et infirmières et soignants du service des urgences de l'hôpital de Saint-Avold sont en arrêt maladie. 36 sur 38. il n'y a plus d'accueil la nuit à partir de 19h 90% des effectifs des urgences de l'hôpital de Pontoise, en région parisienne sont en arrêt maladie. Commence en arriver là. Je ne peux plus entendre que c'est la faute du Covid. C'est la faute de la grippe c'est la faute des bronchiolites ou comme on nous le rabâche tous les matins depuis des mois, c'est la faute des trois en même temps un système de santé existent pour éviter que les gens ne tombent malades et pour les soigner quand ils le sont un système de santé ne s'effondre pas à cause des maladies comme un système éducatif ne s'effondre pas à cause de l'illettrisme, comme un système judiciaire ne s'effondre pas à cause des crimes comme un système électoral ne s'effondre pas à cause des élections. Le système de santé et là, parce que la maladie existe parce que la prévention est nécessaire et parce que la guérison est possible c'est son objet, le sens même de son existence et s'il s'effondre parce que les gens ne tombent malades, c'est qu'il s'effondre de lui-même et s'il s'effondre de lui-même c'est pas ce qu'il a été sous-financés au point qu'il ne puisse simplement plus tenir. Je ne peux pas entendre non plus que c'est la faute des 35 heures. Quel déshonorant mépris à l'encontre de celles et ceux qui, à bout de souffle s'épuise chaque jour et chaque nuit et qui persiste à le faire malgré tout pour faire la mission qu'ils ont accepté soigner. Si pour soigner, il faut soi-même, être malade et épuisé si pour guérir les autres, il faut se tuer à la tâche si notre système de santé doit reposer sur des personnes condamnées à en avoir besoin qu'elle leur, elles ne sont pas en bonne santé. Tout ça n'a plus aucun sens. Alors non, la responsabilité de l'effondrement de notre système de santé publique. Ce ne sont ni les maladies ni les 35 heures la responsabilité elle encombre à celles et ceux qui ont organisé le désinvestissement de l'hôpital public. Le forfait patient urgences les salaires de misère, les conditions de travail indignes, la tarification à l'acte, les fermetures de lits, les fermetures de services et des déserts médicaux. Notre système de santé il subit l'enchaînement depuis plusieurs décennies de décision politique à courte vue dominée par une idéologie mortifère qui consiste à considérer que les services publics doivent coûter le moins cher possible et que la santé et de ne pas reconnaître que la santé est un bien commun et que le service public qui s'en occupe doit et cela fait tellement d'années qu'on le dit être organisé uniquement en fonction des besoins Il y a sans doute plus grave encore, c'est que pire arrive. Permettez-moi de vous lire quelques phrases. Selon un rapport de l'OMS de 2016 23 % des décès dans le monde sont directement liées au fait d'avoir vécu ou. Dans un environnement insalubre et ce sont les plus défavorisés qui supportent la plus forte charge de morbidité liées à l'environnement. Le changement climatique et l'appauvrissement de la biodiversité provoqueront des chocs écologiques de forte amplitude sur notre économie et la société dont la pandémie actuelle il date un peu le texte d'origine zoonotique n'est qu'une des premières manifestations notre protection sociale n'est pas suffisamment résilientes face aux risques environnementaux et l'État ne s'est pas dotée des outils prospectif pour faire face à la survenance plus fréquentes et plus aiguë d'événements climatiques et de crises imprévues dont les effets sur les finances publiques seront lourdes conséquences la pandémie l'montré avec force les chocs futurs risques que d'être encore plus violents. Il est donc urgent de changer de paradigme, avec des politiques publiques dont l'impact environnemental est prise en compte dès la conception et en développement en développant une culture de prévention d'adaptation et de résilience. Notre système de. Protection Protection sociale. Ces quelques lignes, c'est pas moi qui les ai écrites enfin pas directement. Elles viennent du rapport sénatorial adopté par notre chambre sur la sécurité sociale, écologique dont j'avais l'honneur d'être là. Rapportrice qui peut prévoir l'impasse vers laquelle nous fonçons hé bien ici tout le monde. Le seul truc c'est que tout le monde n'est pas ici au pouvoir pour l'éviter.

tout d'abord je je je vais le redire, c'est bien parce que nous ne pas de travers sont pas une crise mais que c'est bien l'enjeu de la réforme structurelle de notre système de santé qu'il nous faut. Accomplir que nous parlons de refondation. Comme toute activité humaine. Le système de santé et bien sûr sensibles aux enjeux climatiques. Le gouvernement fait de la santé environnementale, une de ses priorités dans la politique de santé. J'ai dans ma feuille de route la santé environnementale, j'étais ce matin aux travaux du Haut Conseil de la santé publique, sur lequel nous avons pu commencer à tracer quelques briques d'un projet de santé environnementale dont j'aurais sans doute dans les semaines à venir. L'occasion de venir vous parler. La France fait partie des États européens les plus engagés en matière de santé environnementale elle élabore tous les 5 ans un plan national santé-environnement déclinée en région, inscrit dans le code de la santé publique, ces plans successifs ont permis des avancées notables pour réduire l'impact de l'environnement sur la santé, une meilleure prise en compte de la santé environnement à toutes les échelles du territoire et le développement de programmes de recherche structuré le 4ème plan a été lancée en 2021, il comporte plusieurs axes pour réduire les expositions environnementales affectant la santé humaine ou mieux connaître les expositions et les effets de l'environnement sur la santé des populations et des écosystèmes. De même, nous intégrons les impacts environnementaux des activités de santé, la question de l'évacuation des déchets d'activités de soins à risques infectieux sans atteinte dans l'environnement ou en développant les possibilités de recyclage font ainsi l'objet de travaux avec l'ensemble des professionnels de santé. Ces enjeux concernent beaucoup de beaucoup de ministères et soyez convaincus que le gouvernement. Fait met tout en oeuvre pour que ce dossier soit traité de façon inter-ministériel et systématiquement, je suis aux côtés de Christophe Béchu et de Bérangère Couillard lorsqu'il s'agit de parler de problèmes d'air ou de problèmes d'eau parce que la santé la santé environnementale, c'est quelque chose dont nous devons nous préoccuper et c'est ce que nous mettons en oeuvre et puis prévenir c'est guérir. Donc la prévention est aussi un enjeu majeur de la politique que nous avons bien l'intention de mener ni un Ministre de la Santé et de la prévention et dans le cadre du Plfss. Nous avons déjà pris des mesures en ce sens. Merci madame la ministre. La parole est donc à monsieur Jean Luc. Pour le groupe socialiste, écologiste et républicain pour quatre minutes, chers collègues. Madame

Madame la présidente. Madame la Ministre, mes chers collègues. Tous les secteurs de la santé dans notre pays traverse une crise profonde. Médecine de ville, hôpital profession paramédical tous les acteurs de santé font état de leur épuisement et de leur découragement. La santé est un bien commun, chaque citoyen devrait pouvoir se faire soigner d'une manière optimale. Ce qui est loin d'être le cas depuis de nombreuses années. La crise actuelle renforce ma conviction profonde de la nécessité absolue de la création d'un nouveau service public de la santé fort rappelons une évidence. Le service public et le Patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Les réactions des différents acteurs de la santé à l'intervention présidentielle de vendredi dernier sont majoritairement marquée par un sentiment de déception. Le président Macron. Rend pardon.-- Le plusieurs Macron et fidèle à sa ligne politique avec par exemple la remise en cause des 35 heures à l'hôpital vieilles lunes de la droite, la réponse au malaise actuel de l'hôpital serait de faire travailler plus les personnels hospitaliers sans que ceux-ci gagnent plus. Rappelons que dans le cas de la loi de financement de la Sécurité sociale 2023. A été votée par la majorité présidentielle la possibilité pour les médecins, les infirmières de travailler jusqu'à 72 ans. Quel cynisme. Il est urgent de dégager de vraies solutions pour répondre à la pénibilité des métiers beaucoup d'infirmières par exemple abandonne, moins de 5 ans après leur diplôme.-- Certaines solutions. Préconisées peuvent sembler aller dans le bon sens, comme la remise en cause de la tarification à l'activité à l'hôpital la T2A ans. Mais attention aux modalités d'application. Et pouvez-vous nous préciser ce que sont les objectifs de santé à l'échelle d'un territoire évoquée par le président. Le président a aussi évoqué des conseils d'administration des hôpitaux qui semble-t-il se substituerait au conseil de surveillance actuelle peut-on être éclairé sur ce point.-- Il vous appartiendra Madame la Ministre de mettre en application les annonces présidentielles, mais force est de constater que vous apparaissait affaibli. Par la nécessité éprouvée par le président de la République de monter en première ligne.--

est. Dispositif qui était à son initiative d'ailleurs pas de contrainte non plus pour les gardes des médecins libéraux. Obligation de garde qui permettrait pourtant de décharger les urgences hospitalières des petites urgences aucune réflexion sur les conditions d'exercice pourtant difficile des internes en médecine hospitalière. Rappelons que 30% de nos concitoyens vivent dans un désert médical. 6 millions de Français n'ont pas de médecin traitant, dont 600.000 d'entre eux. Pourtant en affection de longue durée et les mesures annoncées vendredi dernier sur ce point précis ne rassure pas. La délégation de soins et donc la possibilité de prescrire aux paramédicaux est une orientation intéressante. Mais dangereuse si elle n'emporte pas l'adhésion des professionnels de santé et si elle n'est pas présenté dans le cadre d'un projet global. Le président de la République semble avoir totalement renoncé au volontarisme politique dans le domaine de la santé. Pas d'annonce sur un moteur, moratoire sur les fermetures de lits. Incertitudes sur les moyens, pas d'annonce sur les déserts médicaux. La santé a besoin d'un plan global, cohérent, loin des annonces à l'emporte-pièce. C'est pourquoi nous sénateur socialiste, écologiste et républicain. Nous sommes favorables à une véritable plan massif d'investissements dans le domaine de la santé en conclusion de mon intervention, je veux insister l'importance d'associer l'ensemble des parlementaires des sénateurs à la construction d'un projet global de santé pour notre pays, seul à même de garantir le droit à la société, surtout de

Madame la présidente. Monsieur le sénateur. Nous sommes d'accord au moins sur un point, la sentier est un bien commun et c'est bien parce que tous les acteurs et tous les secteurs. Ne vont pas bien, qu'il nous faut, je le redis, refonder l'ensemble de notre système de santé, c'est-à-dire à la fois l'hôpital et à la fois la ville. Le président de la République n'a pas remis en cause les 35 heures. Il a simplement dit qu'il fallait donner plus de souplesse et plus d'autonomie pour permettre au système hospitalier pour permettre à l'échelle d'organiser les emplois du temps des personnels soignants afin d'euros participer et de reprendre en compte cette qualité au travail de permettent de leur redonner du sens et de permettre. Au personnel soignant, peut être de rester à l'échelle de ce service et de ne pas je l'ai déjà dit tout à l'heure, comme c'est le cas dans trop de service actuellement. Aller de service en service, mais de rester dans le service. Quels ont s'agit la réforme de la T2A, qui doit être. Programmé dans le cadre du prochain Plfss la réflexion sera lancée. Avec des objectifs de santé publique qu'il nous faut qu'on construire et qu'il nous faut construire aussi à l'échelle des territoires, je le redis, les objectifs de santé publique ne peuvent pas être identique dans tous les territoires, ça n'est pas possible, même si nous devons assurer un socle et enfin en ce qui concerne les médecins. La convention médicale est en cours, les, les discussions ont lieu, elles auront lieu jusqu'au mois de mars nous sont avec les médecins généralistes dont je répète que nous souhaitons que la médecine de ville s'inscrivent dans une logique de gagnant-gagnant, que le médecin généraliste doit rester traitant doit rester la Pierre angulaire de notre système de santé. Ces négociations sont en cours. 650.000 personnes sous elle des médecin traitant c'est un objectif ambitieux, nous arriverons avec les médecins à répondre à ses besoins de pour nos concitoyens et enfin en ce qui concerne la délégation de tâches, elle ne se fera pas contre les professionnels mais elle se construira bien avec les professionnels et tous les professionnels, c'est l'enjeu du Clio et de la volonté partagée par tous les ordres qui a été signé. C'est ce que nous allons mettre en oeuvre avec les professionnels de santé. Monsieur fiché. Il y a cette réplique c'est pour ça qu'il faut que chacun respecte son le ces minutes. Terminer mon propos puisque ce que je voulais en conclusion c'est dire aussi qu'il était temps, dans la réflexion qui était la note de peut-être mettre un arrêt à la gestion privée lucrative des établissements de santé, à l'instar de ce qui se passe. Dans les maisons de retraite et à l'éclairage de ce qu'on a vécu avec Orpea. Je pense que c'est un système de gestion privée lucrative qui faut réinterroger pour mieux s'orienter vers le public et le privé non lucratif, je vous remercie. Merci la parole est à madame Nadia sur le goût pour le groupe Union centriste pour 4 minutes, chers collègues. Madame la présidente. Madame la Ministre, mes chers collègues. Notre système de santé traverse une crise grave profonde inédite généralisée dont les victimes sont tout autant les soignants que les patients chacun de se sent lésé oublié désespérée. Le principe est mathématique. D'un côté une demande de soin de l'autre une offre de soins. L'unité de mesurer le temps horaire, il faut réussir très vite à remettre un signe égal entre les deux membres de cette équation. Du côté de la demande de soins, il faut un travail de fond sur la prévention d'une part et la bonne orientation des patients. D'autre part éviter que ce volume ne soient gonflés par tout ce qui est évitable et par les actes redondants tout particulièrement. La prévention est une mesure qui relève du temps long. L'efficacité du parcours de soin dans le temps plus court mais très perturbée par la pénurie généralisée de soignants associer une forme de panique des patients qui leur fait rechercher n'importe quelle solution en cas de besoin. Du côté de l'offre de soins. Le volume est largement insuffisant toutes professions de santé confondues concernant l'offre de temps médical, il faut des mesures urgentes et parfois de simple bon sens qui nous remonte du terrain que vous connaissez pourtant mais qui n'arrive pas à être opérationnel. Par exemple les dossiers de médecins étrangers, européens ou non aux équivalences reconnu en France doivent être traités en urgence par les services du Conseil de l'Ordre national. Ils sont des milliers en souffrance en attente parfois depuis des mois d'une date de réunion de commission on nous sollicite tous les jours pour des dossiers de cette nature incroyable qu'on ne puisse pas faire mieux renforcer les services s'il le faut, Madame la Ministre. Pour reprendre mon équation à multiples inconnues. Je ne pense pas que le temps médical soit toujours optimisés. délégations de tâches de soins télémédecine dans certains cas allégement des tâches administratives. Il faut que les médecins puissent se concentrer sur leur principale Value, c'est-à-dire le diagnostic et cesse de perdre la moindre minute en transport ou à remplir des papiers par exemple. Le nombre de ces derniers conditionnent bien évidemment le volume de temps médical offert. Si les nouveaux praticiens pour de multiples raisons produisent globalement en 2 fois moins de temps médical que ceux des générations précédentes. Eh bien il faudrait théoriquement en former deux fois plus, même en modulant avec les autres leviers, force est de constater qu'avec 12.000 médecins formés par an au lieu de 20.000. La situation ne fera en fait qu'empirer nos facs de médecine au professeur de médecine, même avec les cours en distanciel ont-ils atteint un maximum capacitaire quand on sait que chaque année désormais des professeurs de médecine démissionnent de leur. Faute de moyens pour mener leurs travaux. On comprend qu'il faut redonner de l'attractivité à ces carrières essentiel car voir nos étudiants partir en Roumanie ou en Espagne pour se former. C'est un élitisme insupportable et un grave. Constat d'échec d'une façon plus générale l'attractivité des carrières est un sujet d'une brûlante actualité. Les médecins généralistes ne réclame pas qu'une augmentation de leurs actes. J'entends surtout qu'ils demande le dialogue la reconnaissance et les moyens d'attirer partout sur le territoire de jeunes praticiens passionné. Je me demande comment se sentent les étudiants en fin de cursus avant de faire le grand saut dans la marmite bouillonnante du système de santé français. Ce ne sont pas des primes qu'il faut leur donner mais des assurances. Nous manquons de 60.000 infirmiers et 120.000 diplômés n'exercent pas en France peut-on renouer le dialogue avec ces derniers. C'est plus immédiat que d'en former de nouveaux et comment éviter que nos futurs diplômés ne jette l'éponge au bout de quelques années ce gâchis de formations est dramatique et coûte terriblement cher l'attractivité le je l'ai dit, n'est pas que financière, nos auditions nous laisse entendre qu'il s'agit aussi à l'hôpital de gouvernance de lourdeurs administratives à cet égard, le modèle de l'hôpital de Valenciennes où les soignants semble s'épanouir et dont le budget excédentaire peut-il être une source d'inspiration. J'ai évoqué la situation des médecins, des infirmiers mais que dire des aides-soignants des sages-femmes, formées en nombre dramatiquement insuffisant des dentistes qui sont toujours en dessous des radars des kinés qui doivent bénéficier de ça. Il a, chers collègues. Merci, c'est très variable.

place. La mise en place du numerus apertus en 2019, nous avons beaucoup augmenté notre capacité à former des médecins, ce sont ainsi près de 52.000 étudiants en filière médecine qui seront formés entre 2021 et 2025 par toutes les facultés du pays, soit 10.300 par an en moyenne. Cependant, au vu de la longueur des études de médecine, nous le savons, les effets de la fin de numerus clausus ne se verront effectif pas avant 2030. Donc nous avons 8 ans difficile encore à venir. Il nous faut donc travailler autrement. Vous avez évoqué la délégation de tâches, elle est clairement une solution que nous devons approfondir contrairement aux caricatures que l'on entend parfois. Il ne s'agit pas de remplacer des médecins dont, je le redis, nous souhaitons qu'il reste la Pierre angulaire de système de santé et le chef d'orchestre par du personnel moins qualifié. Il s'agit au contraire de concentrer chaque professionnel de santé sur les tâches les métiers et la complexité pour laquelle il a été formé, pas sur des tâches, parfois un peu répétitif plus simple qui peuvent être déléguée à d'autres professionnels paramédicaux

réunion, une réunion pas plus tard que tout alors avec l'Ordre des médecins qui prend l'engagement de nous accompagner avec le CNG pour tenir ce cap de avril 2023 pour téter le stock et de travailler dans le cadre de budget l'immigration sur la nouvelle parcours. De. Du flux dont nous avons parlé récemment. S'agissant de mon espace santé. 65 millions de nos français ont aujourd'hui un espace ouvert et moins de 2% des citoyens se sont opposés à sa création, plus de 5 millions de documents sont versées chaque mois dans les espaces santé c'est un outil au service de la coopération entre le professionnel de santé ainsi qu'au bénéfice de français pour pouvoir s'approprier pleinement leur dossier médical et vous avez raison renouer avec tous les professionnels qui n'exerce plus. C'est aussi un moyen de plus rapidement les faire revenir dans le système de santé et répondre à ce manque de professionnels qui est criant et qui je le répète c'est pas un manque de moyens c'est bien mardi professionnel. Merci. Même si le pour reprendre ma conclusion, je voulais avoir un mot aussi pour les pharmaciens, tous les autres professionnels hein souffrance. Bon j'ai j'ai bien parlé d'une équation ou en en parlant de temps médical et pas un nombre de professionnels de santé, si bien que même si en forme 10.000 praticiens 10 pour En fait il donne quand même beaucoup moins de temps médical qu'avant. Donc si il donne 2 fois moins temps médical c'est pas 10% de plus qu'il faut c'est deux fois plus, donc l'équation elle est mauvaise, donc le fait d'avoir supprimer le numerus clausus clausus à sa règle pas du tout le problème, on en forme toujours pas assez même après suppression du numerus clausus 10% plus, c'est totalement hein. Visant ça va être de pire en pire voilà merci j'un collègue, la parole est à madame Corinne. Imbert pour le groupe Les Républicains pour sept minutes.

Madame le président, madame la ministre. Eh bien, chers collègues. Nous voilà donc aujourd'hui réunis pour un débat d'actualité intitulé la crise du système de santé. Malheureusement le terme d'actualité est un euphémisme quand une situation dure et se dégrade de jour en jour de mois en mois et d'année en année, on parle alors de routine quotidienne si délétère soit-elle. Le sujet est vaste et ces quelques minutes ne saurait être suffisante pour balayer les multiples causes qui ont conduit à la situation actuelle. La pandémie a évidemment aggravé la situation, avec l'épuisement des professionnels de santé à l'hôpital comme en ville, mais elle a surtout été révélatrice de la perte de notre souveraineté sanitaire.-- La crise du système et d'abord le fruit de plusieurs années de politique hasardeuse en matière de santé. Comment ne pas rappeler les coups de rabot subis par l'hôpital et par le secteur du médicament et du dispositif médical dans une logique de la recherche d'une maîtrise des dépenses de santé et de la réduction du déficit de la Sécurité sociale. Comment en est-on arrivé là. Les 35 heures non compensée appliquée à l'hôpital alors que ce dernier prend en charge des patients en 24h sur 24, 7 jours sur 7. Qu'on le veuille ou non, elles ont désorganisé des efforts du coup sans compter demander aux internes au titre de leur formation et dont la contribution est oh combien important dans le fonctionnement du coup de l'hôpital, il en a résulté une formation pendant des années très hospitalo-centrée années pendant lesquelles la médecine générale a été aussi dévalorisée. Le souci du déficit de la Sécurité sociale qui est d'abord le souci d'une juste dépense de l'argent public mais qui, depuis des années a vue Bercy prendre le pas sur l'avenue Duquesne une exception, il faut le reconnaître, la pandémie qui a conduit pour répondre à cette crise sanitaire a un déficit historique de la sécurité sociale. L'objectif national des dépenses d'assurance maladie pour 2023 rejeté dans cet hémicycle en novembre dernier, illustre l'incohérence entre d'un côté des moyens financiers importants de 150 milliards d'euros et d'un autre côté, des missions d'intérêt général, par exemple le mal identifié et le financement de l'hôpital pour laquelle il n'y a pas de débat. Faute d'information.-- Le 15 décembre dernier. J'alerte également le gouvernement lors du des traditionnelles questions d'actualité sur le thème de la souveraineté sanitaire. Entre autres le sujet des ruptures de stock de médicaments et de vaccins qui avait déjà fait l'objet en 2018 donc avant la pandémie, d'une mission d'information sénatoriale. Alors même que le monde traverse une tempête diplomatique inédite depuis la fin de la guerre froide, il semble fondamental de prendre à bras le corps cette question de la souveraineté sanitaire. Tiens d'ailleurs à saluer l'initiative de nos collègues du groupe CRCE visant à créer une commission d'enquête sur les ruptures de stocks et ainsi poursuivent les travaux sur ce sujet. À titre personnel je n'ai jamais vu une stèle situation en 40 ans d'exercice professionnel. Je suis sûr que vous êtes dans la même situation, madame la Ministre. Enfin, la question de la souveraineté du médicament est intimement liée aussi à son prix, qu'on le veuille ou non, dans un marché concurrentiel certains laboratoires préfèrent se tourner. Alors que la demande est mondiale vers des pays où les prix sont plus avantageux. Ce, ce qui a des conséquences directes. Une demande. Mondiale qui augmente, mais également des conséquences sur la capacité d'innovation dans le domaine de la recherche. Se pose ainsi la question par exemple de l'efficience dans certains cas de la clause de sauvegarde. Enfin sur la question de la fixation du prix du médicament. Je rappelle qu'un amendement avait été voté à l'initiative de notre collègue René-Paul Savary afin d'encourager les entreprises du médicament qui relocalisent. Leur site de production en Europe. Malheureusement, le gouvernement n'a pas écouté la sagesse du Sénat. Comment ne pas évoquer lors de ce départ. La question de la formation en internat de médecine générale je rappellerai une nouvelle fois c'est pas la première fois que je le rappelle, mais qu'un amendement avait été voté à la quasi-unanimité du Sénat lors de la loi de santé de 2019 hein. Transformer la dernière année de 3ème cycle de médecine générale en une année de professionnalisation dans les territoires sous-dotés. À l'issue de la commission mixte paritaire. Nous avions trouvé un accord sur un semestre, le décret n'est jamais paru et depuis lors du dernière PLFSS, le gouvernement a repris l'idée d'une 4ème année donc l'idée de la proposition du président Bruno Retailleau voté en octobre dernier d'une 4ème année de professionnalisation pour les internes en médecine générale dans le cadre de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023. 2 constats amers sur ce sujet. Premièrement que de temps perdu depuis la loi 2019. Cette mesure aurait pu rentrer en application, je le rappelle, depuis le 1er novembre 2021. Deuxièmement vous avez dénaturer cette mesure en permettant que cette 4ème année puisse en partie être réalisées à l'hôpital alors que l'esprit initial était de renforcer une médecine de ville aux abois.-- Pour rester sur le sujet majeur de l'accès aux soins. Je rappellerai l'importance qu'occupe et de que doit continuer d'occuper la médecine générale. Le peu de temps, que le président de la République a consacré dans son discours de voeux à la médecine de ville. Interroges voir est un peu choquant. L'hôpital ira mieux si la médecine de ville va mieux.-- Nous sommes face à un système de santé au bord de la rupture. Cette phrase n'est pas de moi, même si parfois à la fin d'une journée, je peux le le penser. C'est le cri d'alarme du collège de la Haute autorité de santé en avril 2022. Le collège de la HAS a en effet publié une lettre ouverte je cite à tous ceux qui oeuvrent pour la qualité des soins et des accompagnements. Le collège proposant bien sûr en face de, de ce cri d'alarme proposant des mesures à mettre en place en urgence, madame la Ministre, avez-vous pris connaissance de cet appel de la HAS et qu'en avez-vous fait. Si ce jugement est sévère et nous attriste tous c'est aussi par endroit une triste réalité. Les professionnels de santé, l'ensemble des soignants sont épuisés sont sous l'eau et je m'inquiète du jour où la digue pourrait sauter car je vous le rappelle Madame la ministre à l'effondrement de notre système de santé, aura des conséquences sur l'ensemble de la société et menacerait directement l'équilibre de ce pays. Je tiens à saluer tous ceux qui tiennent bon et qui continue avec conscience professionnelle et abnégation de prendre en charge chaque jour des patients. Je tiens également rappelé la formidable l'implication des élus locaux qui se battent sans relâche afin de faciliter l'installation de professionnels de santé dans leur commune. C'est un véritable cri de désespoir de la part des élus et des patients que nous entendons régulièrement dans nos départements respectifs. La crise de notre système de santé est évidemment majeur à l'hôpital et en médecine de ville. Nombreux sont les professionnels de santé près pourtant à vouloir sauver ce système dans l'intérêt des patients. Grâce aussi à des progrès technologiques et à des innovations thérapeutiques majeures. Mais cette crise de notre système de santé impact déjà le secteur médico-social et tous les acteurs qui intervient dans la prise en charge des personnes âgées et des personnes handicapées à domicile, ne l'oublions pas. Que dire du Ségur dans l'intention initiale était bonne, mais qui a engendré des oubliés et des oubliés des oubliés, parler de l'attractivité des métiers ne suffit pas, il faut effectivement fidéliser ceux qui sont en poste. En fait, si vous pouvez compter sur les maisons de santé prof multiple pardon pur et professionnels et les professionnels de santé qui les composent. Et il y a le courage de reconnaître que les communautés professionnelles.

Madame la Ministre.-- C'est moi. Madame la présidente.-- Madame la sénatrice.-- Je vais essayer de répondre vous avez posé beaucoup de questions au moins sur la partie concernant la pénurie des médicaments donc annoncé par le président de la République en 2021, le volet santé du plan France 2030 prévoit un ensemble de mesures législatives et réglementaires ainsi que 7,5 milliards d'euros pour faire de la France, la nation la plus innovante et souveraine en santé d'Europe. Il s'agit notamment de faire de la France un leader en matière de produits de santé innovants et de renforcer l'attractivité de la France. C'est un défi majeur que nous avons largement abordé pendant la crise sanitaire, et pour lequel nous agissons. Notre objectif, c'est de réinstaller en France et plus largement en Europe ces industries essentielles de production de médicaments, des projets de relocalisation très concrets émerge progressivement et permettront à terme de limiter notre dépendance, vous le savez, l'usine de paracétamol avec le projet séquence. L'usine de masques et de gants en nitrites. L'usine de production de médicaments dérivés du sang. À partir du plan plasma. À Arras. En 2023, l'objectif national des dépenses d'assurance maladie était fixé à 244 milliards d'euros, soit une croissance de 3,5%. Hors dépenses Covid. Il est donc difficile de parler de coup de rabot et je vous le répète le budget santé a augmenté de 20% entre 2017 et 2023. Par ailleurs, aucune économie n'est envisagée sur les hôpitaux. S'agissant de la 4ème année du diplôme d'études spécialisées de médecine générale. Il ne s'agit pas de réaliser un stade Ange au Soudan. Cette réforme a pour objectif de doter la spécialité de médecine générale d'une phase de consolidation. C'est un apport pédagogique qui vise à permettre au docteurs juniors d'acquérir de l'autonomie dans le cadre protecteur de la supervision pour pouvoir s'installer rapidement ensuite à la sortie des études, la maquette de formation du 3ème cycle des études de médecine générale et d'ailleurs en cours de révision. Dans le cadre de cette réforme.-- La médecine générale et l'hôpital doivent être réformé. C'est l'objet de la reformation de la refondation et nous sommes d'accord sur ce sujet. Merci Madame Imbert. Oui madame la présidente. Merci madame la. La ministre, vous terminez vos propos en parlant de refondation du coup je je vais rebondir, président de la République dans son, dans ses voeux à parler. D'un conseil national de la refondation local. Madame la Ministre au fait. Atteint de deux réunionite aiguë et professionnels de santé, non pas de temps à perdre. Je disais à la fin, mes propos vous savez pouvoir compter sur les maisons de santé pluri-professionnelles et sur les professionnels de santé qui les composent. Sur les communautés professionnelles territoires du elles ne sont pas la solution, certaines fonctionnent bien. Mais elles ne sont pas la solution. Oui mais le ministère via les URPS veut veulent qu'elle couvre tout le territoire national. Pourquoi dans dans le département que je connais le mieux, c'est là où il y a le plus de problèmes qu'il y en a pas parce que nous n'avons pas de temps à perdre. Voilà. Les professionnels de santé peuvent être de très très bonnes volontés, si des médecins ont changé si des patients ont changé. Vous savez, pouvoir compter sur eux pour s'organiser en proximité et les laisser faire et aller à l'essentiel.-- Merci beaucoup. Alors je lui ai donné la parole à Madame Agnès Firmin Le Bodo Ministre donc délégué chargé de l'organisation territoriale et des professions de santé. Pour conclure ce débat pour cinq minutes.-- Madame la présidente, mesdames les sénatrices messieurs les sénateurs. La crise du système de santé. Vous avez choisi d'y consacrer l'un de vos premiers débats pour cette année 23 qui s'ouvre. Et je partage avec vous, cette priorité qui est celle de s'attaquer aux difficultés structurelles qui parcourt notre système de santé comme je partage avec vous ce sens de l'urgence que sous-tend explicitement la notion de crise que vous avez-vous choisi de développer. En effet si nous sortons aujourd'hui tout juste de la violente tempête épidémique de la Covid 19 dont les vagues successives ont ébranlé notre système de santé, notre santé n'en est pas moins en crise et vos nombreuses questions et interventions le démontre. Car oui la baisse inexorable de la ressource médicale qui est la conséquence de choix politiques d'un autre temps, le vieillissement de notre population la mutation des modes de vie et des aspirations des professionnels de santé. La perte de sens de ces beaux métiers du soin, ce sont là les déterminants d'une crise systémique dans un monde qui change. Ce constat de crise ce diagnostic. Il a déjà été maintes fois été posée. Le président de la République a eu l'occasion de le rappeler lors de ses voeux aux acteurs de la santé vendredi dernier. Une fois cela dit et répété, il nous faut désormais être à la hauteur dans ce qui constitue aujourd'hui un moment charnière. Nous devons bâtir le président de la République a tracer un cap clair le 6 janvier dernier dans son allocution à l'hôpital de Corbeil-Essonnes avec des jalons de mise en oeuvre pour avancer ensemble dans ce chantier collectif. Nous avons un horizon et les objectifs. De trop combat reste celui de la lutte contre toutes les inégalités en matière de santé, qu'elle soit sociale géographique ou liés à des vulnérabilités particulières comme le handicap ou le grand âge. Un chiffre pour moi est le symbole de cette crise de l'accès aux soins. 657.000 de nos concitoyens atteints de maladies chroniques, vous l'avez évoqué plusieurs fois n'ont pas accès à un médecin traitant ou un équipe soignante cette réalité, il faut la regarder en face, sans pour autant qu'elles en deviennent moins intolérable. J'ai pu l'évoquer une bonne politique et celle qui se fait rencontrer le temps bref des crises avec le temps long des grands changements structurels. Nous avons transformé le numerus clausus en numerus apertus et corriger une erreur historique. Mais les bénéfices de cette réforme ne seront visibles que dans une décennie. Aussi notre objectif et notre défi, c'est de mobiliser tous les leviers nous permettant de gagner du temps médical pour de soignants au service des patients. Ce temps nous le dégageront en délestant les médecins de toutes les tâches, notamment administratives qui ronge sur leurs emplois du temps déjà largement surchargé. Ce temps nous le partagerons mieux entre les différents maillons de la chaîne de soins dans des organisations coordonnées où chacun a sa place pour un être le plus efficace et le plus utile. Concrètement cela pas une part par l'accélération des recrutement d'assistants médicaux dont nous voulons porter le nombres de 4000 à 10.000 d'ici l'an prochain. Cela passe par un effort inédit sur les formations paramédicales avec notamment l'augmentation de 20% des places en instituts de soins infirmiers. Et c'est nouveau paramédicaux nous leur donnerons des perspectives d'évolution de carrière et de nouvelles compétences grâce à toutes les mesures et expérimentations concernant la pratique avancée, l'accès Direct et les délégations de compétences. Les efforts de chacun. Nous nous assurons que leurs charges et plus hi-tech équitablement répartis. Hospitaliers et libéraux, cliniques et hôpitaux doivent participer avec la même intensité à la permanence des soins et seront rémunérés en conséquence. Pour la médecine de ville, comme pour notre hôpital nous oserons prendre à bras le corps des dossiers touchant au coeur de son organisation en accompagnement ces transferts ces transformations.-- Avec en particulier une direction hospitalière rénové pour mieux équilibrer les décisions. Une bascule de la rémunération à l'activité vers une rémunération fondée notamment sur des objectifs de santé publique et un assouplissement des règles relatives au temps de travail. Et cela toujours pour s'adapter à la réalité et permettre de répondre au besoin d'un univers médico-social en mutation.-- Pour nos soignants nous devons très concrètement leur faciliter la vie dans les exercices quotidiens dont l'exigence et parfois la pénibilité ne sont plus à prouver. En 1er lieu nous avancerons dans la compensation de cette pénibilité et sur le travail de nuit dans l'attente des mesures transitoires prises à l'occasion de la mission flash sur les urgences ce roman. Si inédit.-- La dureté de l'exercice en que l'enjeu majeur de prévention de l'usure professionnelle seront comme l'a dit la Première ministre hier prise en compte dans la prochaine réforme des retraites. Je me réjouis donc que nous ayons aujourd'hui ce débat essentiel dans la perspective de la refondation de notre santé publique pour laquelle certaines pierres importantes ont déjà été posées. Je vous remercie. Merci, madame la Ministre. Alors je vais suspendre la séance. Juste quelques instants pour permettre à chacun de s'installer pour l'examen du prochain point à l'ordre du jour. La séance est suspendue.

La séance est reprise. Alors en application du 5ème alinéa de l'article 13 de la Constitution. Ainsi que de la loi organique. De la loi prises pour son application, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a émis lors de sa réunion de ce jour un avis favorable. 25 voix pour, 5 voix contre à la nomination de Monsieur Patrice vers Great à la présidence du conseil d'administration de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France L'ordre du jour appelle le débat sur la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. La la. Rédaction. Alors je vais rappeler un peu la règle du ce débat. Le gouvernement aura la faculté s'il le juge nécessaire de prendre la parole immédiatement après chaque orateur. Pour une durée de deux minutes Xi môme. L'orateur disposera alors à son tour d'un droit de répartis pour une minute. Voilà Monsieur le Ministre, vous pourrez donc si vous souhaitez répondre après chaque orateur. Une fois que celui-ci aura retrouvé sa place dans l'hémicycle où une place dans l'hémicycle. La parole et tout d'abord à l'orateur de la commission qui a demandé ce débat monsieur Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances pour huit minutes. Madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Ce débat sur la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale s'inscrit dans la continuité des travaux de notre commission des finances et de la de notre assemblée depuis d'ailleurs de nombreuses années.-- Il y a bien sûr eu l'examen de la loi relative à la lutte contre la fraude en 2018 qui comprend de nombreux apports du Sénat mais aussi des tables rondes organisés par notre commission sur les Pandora Papers les comme X-Files et les amendements que nous avons pu proposer dans l'examen de des lois de finances. Surtout, nous venons d'achever une mission d'information de notre commission présidée par. Le président Claude Raynal. Et donc j'étais le rapporteur et qui a rendu ses conclusions au mois d'octobre dernier. lutter contre la fraude poursuit en fait un triple objectif dissuasif. Budgétaire et répressif j'insisterai sur la dissuasion, car être efficace dans notre lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. C'est à la fois. Parvenir à dissuader certains acteurs de tenter leur chance au mépris de nos règles communes mais c'est aussi protéger le consentement à l'impôt et. Assurer le financement par tous, dans le respect des capacités de chacun de nos services publics. La fraude fiscale et d'autant moins acceptable en période de crise. Lorsque nous demandons à tous de faire des efforts et que nous devons maîtriser nos finances publiques, dans le cadre de la mission d'information. Nous avons donc travaillé sur 4 aspects de l'efficacité de la réponse pénale à la fraude fiscale, l'amplification des efforts déployés pour lutter contre la fraude à la TVA l'impératif d'assortir les dispositifs d'accès aux données des garanties juridiques nécessaires pour assurer leur pleine effectivité et enfin le renforcement des outils de lutte contre les montages fiscaux et internationaux adhésif. Notre première conclusion était que l'arsenal normatif mis en place par la France pour lutter contre la fraude apparaît plutôt robuste de fait nos travaux n'appelle pas à une révolution fiscale, mais comme nous le souhaitions aboutissent à un bilan après l'entrée en vigueur de la loi 2018 et à des propositions concrètes, réalistes et pour la plupart facile à mettre en oeuvre rapidement plusieurs recommandations ont d'ailleurs d'ores et déjà donné lieu à des amendements présentés dans le cadre de notre projet de loi de finances pour 2023, la grande majorité a d'ailleurs été voté à l'unanimité et certains ont même passé le couperet du 49.3 je pense par exemple à l'extension des compétences des officiers fiscaux judiciaires aux escroqueries concernant la TVA ou à l'impératif de mieux évaluer la fraude. Il y avait l'avion qui en fait un enjeu fondamental. Au moment où les chiffres se multiplient dans le débat public, parfois un peu à tort et à travers. Nous avons besoin d'évaluation méthodologiquement plus étayée et plus robuste et il faudrait pouvoir estimer, Monsieur le Ministre, quel est le montant des droits fondés frauder pardon que l'administration parvient finalement récupérer 10, 20 30 % plus personne à ce stade ne peut véritablement dire il serait évidemment dommage de nous arrêter là dans le suivi des travaux de notre commission d'abord toutes les recommandations qu'ils peuvent n'ont pas encore trouvé leur traduction législative. C'est le cas par exemple de la sécurisation des dispositifs d'accès aux données ou de certaines propositions concernant la lutte contre la fraude à la TVA. certaines dispositions qui n'ont pas été retenue dans la loi de finances pour 2023 doivent être rediscutés s'agit par exemple du rôle des assistants spécialisés qui aident les procureurs dans le traitement des dossiers de fraude les plus complexes de la détaxe à la TVA des moyens des services d'enquête spécialisés ou encore sujet majeur du droit de visite des douanes. Pour résumer, il nous reste donc encore bien du travail pour donner toute leur portée aux recommandations de la mission d'information et pour améliorer la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Nous devons donc réfléchir aux véhicules le plus approprié pour les inscrire dans la loi. Il est toutefois des sujets sur lesquels d'éventuels progrès ne dépendent pas véritablement du Parlement mais bien du gouvernement et c'est notamment le cas de la lutte contre les montages transfrontaliers abusif. Enjeu majeur en ce qui le constitue une source inépuisable de fraude et d'évasion fiscale. Les évaluations de l'Observatoire européen de la fiscalité sont à cet égard sans appel. Plus de 10% de la richesse nette totale de l'Europe, soit 2300 milliards d'euros sur les détenus à l'étranger pour une perte de recettes fiscales de l'ordre de 55 milliards d'euros par an. L'OCDE estimait en 2020 qu'au niveau mondial, 11.000 milliards d'euros étaient détenus sur des comptes Offshore. Or, disons le, le poids du législateur est relativement limitée pour lutter contre ces phénomènes. Si le gouvernement n'agit pas en amont, que ce soit d'ailleurs au niveau européen ou international et je n'irai pas que le projet de taxation minimale est un 1er pas satisfaisant, même s'il est insuffisant et donc par nature perfectible. Toutefois, il n'y a encore que trop peu d'avancées sur la négociation des conventions fiscales par exemple. Pouvons-nous accepter encore que certaines conventions facilitent les arbitrages de dividendes pratique plus connu sous le nom de tu m'exprimer. Un chiffre. Monsieur le Ministre ces montages aurait coûté à la France 33 milliards d'euros de recettes fiscales en 20 ans sur la seule année 2018, un milliard de aurait échappé à la France pour un montant recouvré de seulement 277 millions d'euros. Quels sont les efforts déployés pour renégocier certaines conventions ou pour les assortir de clauses anti- abus, Monsieur le Ministre. Les services de contrôle fiscal pourtant expérimenté déterminé ne peuvent accéder à des documents essentiels à leurs enquêtes des blocages persistent dans certains pays est la transparence n'est pas toujours garantie. Les actuels liste grise ou noire de paradis fiscaux sont aujourd'hui insuffisantes.-- Que fait le gouvernement, Monsieur le Ministre, au niveau européen comme internationale pour lutter contre les paradis fiscaux et pour accroître la transparence des bénéficiaires effectifs. Quelle sera la position du gouvernement lorsqu'il s'agira de revoir la réglementation européenne. Relative aux informations sur les bénéficiaires effectifs de société.-- Alors que la Cour de justice de l'Union européenne a sévèrement amoindri sa portée à l'encontre d'ailleurs des objectifs de lutte contre l'évasion fiscale. Après cette brève présentation de nos récents constats et de nos recommandations pour l'avenir mais aussi ces quelques questions. Je viens d'adresser à monsieur le ministre, je vous propose de laisser la place au débat et je vous remercie.-- Merci, cher collègue, Monsieur le Ministre hein pour 2 minutes. Merci madame la présidente, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général mesdames et messieurs les sénatrices et sénateurs. Un mot simplement en introduction de ce débat pour dire que je me réjouis que le Sénat est inscrit à l'ordre du jour ce débat qui est un débat. Important, c'est un débat important pour le pacte social parle ici de lutte contre la fraude. C'est un enjeu essentiel pour le consentement à l'impôt et pour notre capacité à rester une société unie. C'est un enjeu politique aussi important. On a pu mesurer au cours de la dernière élection présidentielle, un certain nombre de candidats proposé la création d'un ministère de la lutte contre la fraude. Il se trouve que ce ministère de la lutte contre la fraude. Il existe, c'est le ministère des Comptes publics et croyez bien que c'est une grande priorité que nous fixons pour continuer à renforcer notre efficacité en la matière j'aurais d'ailleurs l'occasion avant la fin de ce 1er trimestre 2023, de présenter un plan de lutte contre toutes les fraudes qu'elles soient fiscales, sociales ou douanières et à ce titre je veux saluer la très grande qualité du travail qui a été menée par le Sénat et par la commission des finances dans le cadre de la mission d'information que vous avez mise on a eu l'occasion d'en débattre à plusieurs reprises dans le cadre du projet de loi de. Finances et vous l'avez indiqué d'ailleurs monsieur le rapporteur général plusieurs des mesures de ce rapport ont été intégrées dans la loi de finances. Certaines d'entre elles l'ont été. Non, malheureusement pas passer le couperet. Non pas du 49.3. Mais du Conseil constitutionnel qui les a censuré pour Cavaliers notamment et nous aurons peut être l'occasion dans des textes futur d'y revenir, en tout état de cause, nous aurons un débat qui est un débat important pour le redressement des comptes publics, puisque ça passe aussi par là, mais plus globalement qui est important pour notre pacte social et là le consentement des Français dans notre modèle de solidarité je vous remercie. Merci sur le rapporteur général La parole est donc à monsieur Rémi Féraud. Pour le groupe socialiste, écologiste et républicain pour cinq minutes.-- Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre cette à la demande de notre commission que nous débattons aujourd'hui de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Suite au rapport rendu par le président Claude rénal et le rapporteur général. Husson. Il y a quelques semaines.

par ailleurs l'historique des mesures prises ces 10 dernières années. Il faut aussi rappeler les progrès qu'ont constitué la création du parquet national financier de l'Office central de lutte contre la fraude et les infractions financières et fiscales ou bien encore la création de la HATVP. C'est grâce à la mise en place notamment de ces institutions que les avancées de notre pays en matière de lutte contre la fraude fiscale, ont été jugé positivement par certaines z'ONG. au cours du précédent quinquennat. Nous avons eu aussi étudier la loi de 2018 relative à la lutte contre la fraude et lors de nos débats. Nous avions groupe socialiste souhaite souligner les avancées du texte, comme la réforme du verrou de Bercy qui avait auparavant fait l'objet d'une proposition de loi de notre collègue Marie-. Pierre de La Gontrie. Mais aussi d'autres dispositions comme celles portant sur la lutte contre la fraude à la TVA constituaient de réelles avancées et nous nous étions d'ailleurs pas opposée à ce texte. Nous avions aussi exprimer nos regrets.-- En revanche sur la timidité du gouvernement quand tu. Sur la question des paradis fiscaux. La liste de ceux-ci, excluant de nombreux pays dont les pratiques s'apparente à un véritable dumping fiscal et notre collègue Thierry Carcenac alerter aussi en 2018 sur les effectifs de la direction générale des finances publiques dédiées au contrôle fiscal alors que le nombre d'entreprises soumises à la TVA ne cesse lui d'augmenter. La mission d'information de la commission des finances permet de dresser un 1er bilan de l'application de cette loi le 1er renseignements qu'elle en tire d'ailleurs et la difficulté d'apprécier l'efficacité de la lutte contre la fraude fiscale en France. Car si les résultats du contrôle fiscal eux-mêmes sont en hausse. Nous ne pouvons pas pleinement apprécié l'efficacité du dispositif, faute de données fiables sur l'ampleur de la hausse mais sur la réforme du verrou de Bercy. Les conclusions de la mission d'information montrent que l'équilibre trouvé en 2018, fournit des résultats encourageants avec une forte augmentation des dossiers transmis par l'administration fiscale au parquet et c'est bien la preuve que cette remise en cause partielle du verrou de Bercy était nécessaire. Sur la TVA les travaux de la commission donne raison aux inquiétudes que nous exprimons puisque la part de la TVA dans les résultats du contrôle fiscal ne cesse elle de régresser d'année en année, il y a sur ce point je crois un réel besoin que les contrôles monte en puissance et il ne faut pas prendre du retard pour que le contrôle s'adapte à l'évolution de la fraude elles-mêmes. Vous le voyez tous les principes alerte objectif que nous a défendu en 2018 sont toujours vrai aujourd'hui. J'ajouterai que ne peut pas y avoir de véritable lutte contre la fraude fiscale s'il n'y a pas une même détermination contre l'évasion fiscale et les paradis fiscaux. À cet égard, les députés de gauche se sont alarmés récemment d'une mesure qui a été inscrite discrètement dans le PLF, et je crois qu'ils ont raison. Dans une tribune qu'ils ont publié dans Le monde ils ont protesté contre la création d'une nouvelle niche fiscale, celle en faveur des captives de réassurances qui a été présenté par amendement au Sénat et adopter, quasiment sans débat en du fait du 49.3. Or ces captives sont un moyen d'optimisation fiscale. Sur la centaine d'entre elles tenues par des entreprises, moins de 10 sont domiciliés en France et le reste répare répartis dans les paradis fiscaux. Est ce que le gouvernement peut justifier d'une vraie détermination contre l'évasion fiscale quand il fait adopter parallèlement une telle mesure et alors que la France est à l'euro près. Selon le ministre de l'économie. Comment le gouvernement peut-il en plus ajouter de nouvelles mesures qui favorisent l'exil fiscal des multinationales et coûteront encore quelques centaines de millions d'euros supplémentaires à l'État. Cela montre bien, comme le disait le rapporteur général qu'il est indispensable d'agir au niveau international et je me félicite aussi de l'instauration d'un impôt sur les sociétés minimum à 15% dans l'Union européenne qui est un 1er pas mais qui doit bien s'inscrire dans une politique globale, cohérente et déterminée pour prendre tout son sens. Parce que l'évasion et la fraude fiscale mine en effet notre contrat social et démocratique ni le consentement à l'impôt, la régulation mondiale, la capacité des peuples à maîtriser leur destin et à rechercher l'intérêt général, qu'en conjuguant des mesures françaises et internationales qu'il sera possible d'établir une politique efficace en la matière et je me félicite que le Sénat contribue Marc, je vous remercie. Vous me le dites qu'on vous voulez répondre. Voilà. Merci. Vos deux minutes c'est court pour répondre à beaucoup de sujets qui sont. Abordés donc il faut choisir. Je vous rejoindrais sur la question de la fraude à la TVA qui est un enjeu évidemment majeur. Je crois que l'Insee dans sa dernière évaluation évalue la fraude à la TVA autour de 20 milliards d'euros par an, donc on voit à quel point on doit être capable d'agir plus efficacement sur le sujet. Sur ce point là il y a un chantier qui me semble absolument majeur qui est celui de la facturation électronique interentreprises qui a été adoptée par le Parlement il y a plusieurs années maintenant, la réforme va commencer à entrer en vigueur à partir de 2024, c'est une réforme majeure en termes techniques, c'est de la même ampleur que le prélèvement à la source. On en parlera probablement moins puisque ça concerne pas tous les Français, immédiatement, mais les entreprises mais croyez bien qu'on y travaille d'arrache-pied pour anticiper les choses pour que ce soit évidemment simple pour les entreprises. C'est pour ça que l'entrée en vigueur sera progressive. Il me semble que le pays qui a mis en place en premier en Europe en tout cas dans les pays comparables. Cette réforme, c'est l'Italie. Qui dès les premières années a pu bénéficier de plusieurs milliards d'euros de TVA recouvrer qui ne l'était pas auparavant, et ensuite il y a un effet comportementale évidemment des entreprises dans leur déclaration. Donc oui sur la priorité. Fraude à la TVA et je crois que le chantier de la facturation électronique est absolument majeur le 2ème sujet c'est le secteur du E-commerce qui a pris énormément d'ampleur et sur ce sujet-là, il y a des discussions qui sont menées actuellement au niveau européen avec la directive E-commerce sur laquelle on souhaite aussi avancer. Merci. La parole est à monsieur Éric Bocquet pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste pour cinq minutes, chers collègues. Madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues.-- Je pense qu'il faut d'abord saluer l'excellente initiative de notre commission des finances je le président rénale. Monsieur le rapporteur général Huchon. Pour mener cette initiative de mission d'information sur la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Près de 4 ans après la loi Darmanin entre guillemets du 23 octobre 2018, relative à la lutte contre la fraude. Il était important en effet, de faire un 1er bilan des nouvelles dispositions adoptées à l'époque et il est très salutaire, que le Parlement s'intéressent à ce sujet de manière permanente, tant l'enjeu pour nos finances publiques est fondamental. L'une des difficultés constatées ces dernières années et tant que les révélations par la faite par la presse sur ces sujets suscite indignation réactions indignées pendant 48 heures au mieux et très vite le soufflé retombe et les réactions du gouvernement ne sont pas à la hauteur des enjeux financiers colossaux impliqués. Chacun a en mémoire ici la déclaration très péremptoire du président Nicolas Sarkozy, le 23 septembre 1002, 1009 pardon. Les paradis fiscaux c'est terminé. Or ces 14 dernières années, les scandales se sont répétées. Si on fait le compte, depuis 2013 années de la tristement célèbre affaire Cahuzac qui a fait tant de mal à notre République. Ce ne sont pas moins de 15 affaires qui ont été révélées par les journalistes d'investigation et les lanceurs d'alerte. Merci à eux au nom de l'intérêt général. Et à chaque fois les mêmes montants astronomiques, les mêmes systèmes sophistiqués et trop souvent malheureusement l'implication de responsables politiques de haut niveau, ici et ailleurs.

Cette accumulation d'affaires illustrent parfaitement le caractère systémique quasi industrielle de l'évasion fiscale. Ceux-ci confère aux responsables politiques quels qu'ils soient une responsabilité majeure. Qu'en est-il donc du bilan de la loi de 2018. La mission a constaté l'insuffisante évaluation de la fraude fiscale notre rapporteur général la rappeler la loi de 2018 avait prévu la création d'un observatoire d'évaluation de la fraude fiscale. Celui-ci n'a jamais vu le jour faute d'avoir quelqu'un pour en assurer la présidence. J'avais à l'époque. Modestement ma candidature à titre bénévole soucieux que nous sommes des deniers publics. L'observatoire et Morné aujourd'hui perdus dans les Landes. Certes le verrou de Bercy fut quelque peu desserré. C'est une bonne chose, sans être toutefois complètement. Nous sommes nombreux à penser que sa suppression totale devrait être envisagée mais cela nécessiterait en parallèle de renforcer les moyens de la justice, le parquet national financier. Notamment de manière que notre justice puisse traiter comme il convient. Tous les dossiers de fraude fiscale. Je ne partage pas la satisfaction de la mission d'information qui estime que les réponses pénales et les instruments de justice que sont la CGIP, la convention judiciaire d'intérêt public que je me demande toujours où est l'intérêt public dans ce dispositif, ainsi que la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la CRPC, une sorte de plaider coupable à l'anglo-saxonne. Certes, le gouvernement met en avant les condamnations de Mac Donald ou du Crédit Suisse ces derniers mois les amendes récupérer ne représente pas la totalité des sommes éludées. Et cette méthode de négociations entre guillemets laisse entendre au commun des mortels que la loi fiscale ne s'applique pas de la même manière selon que vous êtes puissant ou misérable. Pour plagier le grand Jean de La Fontaine. Notre mission d'information a aussi examiné de manière très logique la dimension européenne du sujet. L'Union européenne considère qu'il n'existe en sauce hein aucun paradis fiscal. Je me contenterai de citer nos partenaires entre guillemets du Luxembourg mise en cause en février 2021 dans une enquête au long cours du journal Le Monde son nom au peu luxe. Nous y apprenons que le Luxembourg 55.000 sociétés offshore cumulant ensemble 6500 milliards d'euros d'actifs, 6500 milliards. Mes chers collègues, quasiment 20 fois le budget de la France et parmi ces 55.000 sociétés en tête de classement. Les Français, avec 17.000 de nos contribuables de nos contrées court citoyens qui détenait ces sociétés offshore. L'une des armes essentielles pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscale et l'indispensable transparence. Or de ce point de vue Jean-François Husson, il a rappelé l'Union européenne envoie des messages quelque peu inquiétant et contre-productif ces derniers temps. Pour en juger. Cette décision très surprenant de la Cour de justice européenne, qui considère que la communication des informations sur les bénéficiaires effectifs de société est réservé aux pouvoirs publics et aux organismes spécialement habilitées à les recevoir. Jusque-là, ces informations étaient libres en libre accès sur internet. La Cour européenne freine ainsi les ardeurs des défenseurs d'une transparence absolue. Il est clair que seule une volonté politique forte et pérenne une priorisation de ce qu'on puisse faire avancer véritablement au nom de la tenue générale je vous remercie. Oui. Monsieur le Ministre. Oui merci madame la présidente. Peut-être répondent sur un des points de votre intervention les CGIP les convention judiciaire d'intérêt public. Moi je pense que c'est un outil utile. À plusieurs titres, d'abord ça nous permet de gagner du temps. Avec des procédures qui peuvent être extrêmement longues. Ensuite. Ça nous permet de nous assurer que les finances publiques recouvre une partie très importante de la fraude, là où le fêter quand vous rentrez dans une bataille judiciaire indépendamment du fait que vous avez des appels des procédures qui peuvent être très longue. Il faut savoir aussi, face à quoi en ce bas parfois des grandes entreprises qui ont. Une armée juridique évidemment on est très outillé, aussi l'État, mais en tout cas qui peuvent faire durer les choses et que la succession d'audience et d'appel peut aussi finir par faire baisser le montant in fine et que nous réussissons recouvrer un exemple UBS. Je crois que le contentieux est pas encore. Achevée, mais on voit bien qu'entre la première condamnation, puis l'appel c'est parfois plusieurs milliards d'euros finalement en moins qui sont prévues. Moi j'ai vraiment salué l'engagement des agents et des enquêteurs de la Annie qui notamment ont permis la signature de la CGIP avec Mac Donald cet été et rencontrer pour saluer leur travail c'est un milliard 300 millions d'euros. Vous avez cité aussi l'affaire Crédit Suisse. Moi je pense que c'est un outil utile mais il nous faut et là je vous rejoindrais évidemment. Être capable de regarder si ça vaut le coup entre guillemets de signer ou il vaut mieux aller au contentieux en l'occurrence pour ses affaires. Vraiment les agents remarquables qui ont travaillé, ont considéré et on est d'accord avec eux que ça valait le coup de signer cette CGIP puisque ça nous permet de recouvrer les montants qui était. Questionné et ensuite. Ah ça nous permet aussi d'avoir une entreprise qui se met dans les clous plus rapidement que si on avait des procédures multiple sur plusieurs années. Merci. La parole est à Madame Sylvie Vermeillet. Pour le groupe Union centriste pour quatre minutes, chers collègues.-- Madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, à parcourir les multiples est vertigineuse, estimation de fraude fiscale à les comparer à nos semaines de débats pour ajuster les lois de finances. On a comme une impression de tonneau des Danaïdes. Car pendant que nos travaux se concentrent sur la création la suppression ou la répartition de tel impôt. Des dizaines de milliards nous échappe par fraude fiscale. Je remercie donc et je salue le travail majeur de la mission d'information et celui de notre rapporteur général Jean-François Husson, car compte tenu des montants en jeu il y a bien urgence à agir dans ce domaine. Je souscris sans réserve aux recommandations permettant au service de la DGFIP des douanes et de la justice d'avoir accès aux données nécessaires à leur mission de contrôle et de répression, ainsi qu'aux recommandations qui fluidifie leurs échanges respectifs et partagent les données utiles pour chacune des administrations. Il faut mettre en oeuvre en urgence la recommandation numéro 5 du rapport afin de doubler d'ici 5 ans, le nombre d'officiers fiscaux judiciaires, ce qui suppose que les salaires soient attractifs. Tout commence par là, Monsieur le Ministre. Il nous faut les meilleurs des meilleurs, pour déjouer les systèmes les plus sophistiqués qui soient. Nous en avons fort heureusement quelques-uns de ses meilleurs mais trop peu et trop étroit et sous sous rémunérés pardon au regard de ce que la grande finance peut offrir. Nous n'inverseront pas le rapport de force, si nous ne déployons pas des armes de gros calibre, cela commence donc très simplement par des agents très bien payé en nombre et avec des moyens en matière de fraude à la TVA estimée entre 20 à 25 milliards annuels je ferais 3 propositions. Premièrement les sources de fraude à la TVA sont multiples et ne pas reverser la TVA collectée la reverser à un taux minoré optimiser les opportunités du droit intra-communautaire en multipliant les opérateurs non immatriculé ou défaillants et pas seulement en matière de E-commerce et bien sûr organisé la fraude de type carrousel en raison de ce fléau Carrousel. J'ai un doute sur l'efficacité de la généralisation de la procédure d'autoliquidation de la TVA au 1er janvier 2022 car c'est justement le point de départ de cette fraude. Si les déclarations ne sont pas contrôlés les failles vont devenir des gouffres et le machine learning à disposition des contrôles DGFIP n'est pas encore assez intelligent pour prétendre vérifier la TVA au taux liquider le guichet unique de déclaration de la TVA à l'importation sera-t-il efficace. Je souhaite que nous restions très vigilants sur ce point. Deuxièmement une suggestion concernant les actifs numériques, notamment les NFT non fongibles token pour lesquels la fraude type carrousel est tentante. Essayons de ne pas prendre trop de retard sur les voleurs et adaptons notre réglementation c'est NFT peuvent être instantanément acquis et cédés entre 2 assujettis TVA l'absence de flux physique facilite la fraude comme il n'existe pas de registre officiel permettant de faire le rapprochement entre l'adresse publique détenant les actifs numériques et la dénomination sociale du bénéficiaire. Ne peut-on pas obliger les entreprises françaises, a déclaré comme les particuliers leur compte d'actifs numériques à l'administration fiscale. Troisièmement si la fraude carrousel est un enjeu important. Il y a aussi toute la fraude de base consistant à ne pas déclarer tout ou partie de ses recettes. Je me suis déjà exprimé plusieurs fois sur ce sujet car il est clair que les comptables et les banquiers savent qui trichent et qui déclare. Bien sûr il y a Tracfin. Mais les experts comptable ne vont pas faire des signalements à Tracfin pour des affaires mineures, or ces affaires mineures à l'échelle de la France représente quelques milliards de TVA. Aussi, Monsieur le Ministre, quelle est votre position sur le sujet du secret professionnel inhérents aux professions bancaires et comptable ne pense et vous pas qu'ils pourraient être exceptionnellement levés lorsque l'administration fiscale procèdent à des contrôles. Merci. Chers collègues. Me suis Ministre.-- Merci madame la présidente, madame la sénatrice, je vous laisse pour asseoir. Je vais essayer de répondre sur les 3 principaux points sur le SE-. J-F. Oui et il faut renforcer ses moyens et je voudrais d'ailleurs qu'on élargisse la réflexion au-delà des moyens à la question des. Compétences, c'est un service très utile qui permet des s'enquête judiciaire avec les services de. Bercy et la question qui se pose aussi, c'est celle des pouvoirs. On ne peut pas dissocier la question des moyens de celle du positionnement et d'ailleurs, le Sénat a bien vu ce sujet en préconisant dans son rapport une extension des pouvoirs à l'escroquerie à la TVA. Qui pourrait intégrer d'autres champs de compétence, ça fait partie de la feuille de route sur la fraude que j'évoquais tout à l'heure qui va sur laquelle on va travailler dans les les 3 mois qui viennent. 2ème. Sujet sur les NFT. Ce sont des actifs numériques et ils sont traités fiscalement comme telle. On a d'ailleurs adapter notre droit pour mieux les traiter notamment les revenus issus des. Cryptos on n'est pas pris de court par l'irruption des NFT, on sait les traiter aujourd'hui les particuliers comme les entreprises doivent déclarer les NFT qu'ils détiennent. Mais il faut probablement aller plus loin et perfectionner les obligations déclaratives et nos outils et à ce sujet-là. La Commission européenne a proposé une directive la directive 8 pour renforcer les obligations déclaratives en la matière et je crois que c'est une des priorités de la présidence suédoise pour avancer sur ce sujet et la France sera évidemment aussi à la manoeuvre enfin sur les intermédiaires financiers, moi je veux rappeler que ces professions ne peuvent opposer le secret professionnel lorsque la DGFIP leur demande des informations en tout cas lorsque la DGFIP exerce ce qu'on appelle son droit de communication et d'ailleurs elle transmettre toutes les informations elles ont même aussi une obligation de les communiquer à Tracfin lorsqu'elles ont des doutes sérieux. Et donc vraiment moi je pense qu'il peut y avoir évidemment parfois des professionnels qui ne respectent pas la loi et là il faut les sanctionner les identifier les sanctionner. Ça arrive, mais l'écrasante majorité d'entre eux exercent respecte le droit de communication qui leur est demandé, signale à Tracfin, quand ils ont des doutes. Vous souhaitez répondre. Sa collègue. d'évasion et de fraude à la TVA. Et j'ai vu que l'administration fiscale britannique. Avait. Ouvert une enquête concernant 3 NFT qui mettent en jeu 250 sociétés, donc je crois que. Voilà je je je je suis certaine que vous ne prenez pas de retard et que vous faites ce qu'il faut mais je crois qu'il faut faire une grande vigilance particulièrement sur le déploiement de ces NFT. Je vous remercie pour voir pense. Merci. La parole est au président Jean-Claude Requier pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen pour cinq minutes, chers collègues. Madame la présidente, monsieur le ministre. Monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, comme ça a été dit la lutte contre la fraude et évasion fiscale est un sujet suivi de longue date au sein de notre commission des finances, c'est mon collègue Éric Bocquet a rappelé nos discussions il y a que des années sur l'organisation de fiscale et financière. Un nuit 19 l'air déçu le groupe RDSE avait pour sa part. Organiser un débat à l'initiative de notre ancien collègue Yvon Crolet sur la fraude à la TVA transfrontalière. Un sujet tout aussi crucial. Je vois que cette thématique a été conservé dans les travaux de la mission d'information et je m'en félicite. Le montant de la fraude à la TVA et puis par l'argument ensemble des impôts est en effet considérable. Pourtant en bute encore sur la difficulté à évaluer le montant cas de cette fraude. Et ce à quelques. Plusieurs Plusieurs dizaines de milliards d'euros prix c'était l'aspect particulièrement éclairant du rapport d'information remis à l'Automne dernier je pointe je cite. Un défaut d'évaluation du phénomène de fraude préjudiciable à la juste appréciation des résultats du contrôle fiscal. On ne saurait être plus clair. Plusieurs de nos voisins. Qui ne se sentent qu'ils ne sont sont ils ne sont pourtant pas les derniers. En matière de fraude ou d'optimisation puis estimation de la fraude fiscale ou plus exactement de leur écart fiscal en dans les recettes attendues est celle effectivement recours. Il s'agit principalement des pays anglo-saxons et des pays nordiques. Cela suppose d'importants travaux méthodologiques et les contrôles aléatoires. Ce pourrait être effectivement une diminution de l'Insee. Bonne nouvelle, la première évaluation été a donné en 2022 pour la TVA. Entre 20 et 25 milliards d'euros de fraude aux parents. Cela représente un taux de fraude entre 10 et 15% sur la première ressource fiscale. Notenstein juridique en matière de lutte a pourtant évolué ces dernières années. Je pense en particulier à la suppression du fameux verrou de Bercy en 2008, à mettre au crédit du précédent gouvernement. À revoir le juge il n'avait pas l'initiative des poursuites pour hausse fiscale seulement pour blanchiment de fraude. Aujourd'hui la justice dispose de marges de manoeuvre plus importante. Même si cela a pour conséquence logique, une forte hausse des dossiers à traiter par le parquet national financier. Plus largement, la lutte contre la corruption a été renforcée depuis le vote de la loi sapin de. Denis, 16. Les entreprises, banques et même planté en France doit désormais appliquer des règles de conformité plus strictes ces cantons aussi dans le cadre d'accords internationaux comme ceux de Bâle III parallèlement. Les technologies évoluent aussi l'échange automatique de données est une réalité bien que les moyens des comptes de contournement sont aussi toujours plus sophistiqués. Les règles internationales plus strictes ont eu pour effet collatéral, le développement de la finance de l'ombre le système Betz de l'OCDE visant à lutter contre l'érosion des bases fiscales reste facultative d'hommes viennent domaines. Les propositions des vols d'évolution législative se aussi à la difficulté de procédure, j'ai pas un souci on disposition censurée, il y a quelques jours par le Conseil constitutionnel dans la dernière loi de finances. L'article 83. Qui concernaient la levée du secret professionnel, des agents des finances publiques en faveur des une détaché auprès du procureur de la République et l'article 187 qui réduisait le nombre de membres de la commission des infractions fiscales qui avait pourtant reçu, il faut avoir le Doubs. Ont été considérées comme des cavaliers. La preuve que les salariés de la rue de Montpensier peuvent se montrer aussi tatillon que quelques fois notre commission des finances a matière de recevabilité. Je terminerai mon propos sur les lacunes qui existent encore notre droit national ou européen en 2023. Certaines de nos conventions fiscales bilatérales restent avantageuse pour des investissements et investisseurs étrangers. Alors que la France est souvent décrite comme un enfer fiscal. Il est vrai que notre droit fiscal est un des plus complexes qu'est que la pression moyenne reste élevé à ce propos dispose de d'une évaluation de la fraude involontaires. Liées à l'ignorance de certaines règles fiscales À tort, réellement. Progresser dans la lutte contre l'évasion fiscale. Depuis le sommet du G20 à Londres en 2009. Si les connaissances et les moyens de lutte ce sont indéniablement renforcée. Forcer le constater que les ordres de grandeur sont restés plus ou moins les mêmes. Le mur de l'argent arrive OK il y a plus d'un siècle est pas Édouard Henriot. Encore garde encore de beaux jours devant lui. Merci cher collègue. Monsieur le Ministre.-- Le président Ruquier. Non il ne faut pas courir président. Ouais non non c'est bon on a le temps Merci madame la présidente, monsieur le président requiers vous avez dans votre intervention aborder un point qui est un point majeur, c'est la capacité d'évaluation de la fraude et notamment de la fraude à la TVA. Et ce que je veux dire c'est que c'est. Précisément à l'initiative du Parlement et à la demande du Parlement, comme vous l'avez rappelé que nous avons fait évoluer notre méthodologie d'évaluation de la fraude à la TVA. Le chiffre que j'évoquais tout à l'heure sur la fraude à la TVA estimée par l'Insee. J'ai, j'ai dit 20 milliards d'euros auraient été c'est 23 milliards d'euros. Sur une année il est précisément issue d'une nouvelle nouvelle méthodologie qui a été construite avec les services de la direction générale des finances publiques. On se base sur les contrôles fiscaux qui ont été. Effectués et c'est à partir de cette extrapolation des contrôles fiscaux qu'on fait une nouvelle évaluation on est plus sur l'ancienne évaluation qui était celle qu'on n'appelle. Des quarts de de de TVA dans c'est une méthodologie qui est qui est différente, mais comme vous je crois profondément qu'on doit perfectionner notre évaluation. C'est une question qui revient beaucoup dans le débat public, à combien se porte combien il y a de fraudes dans notre pays qu'elles soient fiscales ou sociales. C'est très dur de répondre si on était capable de répondre précisément. On saura où est la fraude et elle serait. Recouvrer et j'y vois aussi un, un, une question. Y compris démocratiques importante puisqu'on a vu je disais tout à l'heure dans le cadre de la dernière élection présidentielle, que la question de la lutte contre la fraude était très importante. Elle est souvent devenu pour reprendre les procédures que vous évoquiez tout à l'heure au programme présidentiel ce que le tabac et parfois des amendements parlementaires, c'est-à-dire un gage qui permet de faire passer toutes les propositions en fait plein de propositions et pour le chiffrage on va dire que ce sera financé par la lutte contre la fraude mais c'est combien la lutte contre la fraude, ou bien on peut obtenir. Je pense que dans le cadre de la feuille de route que je vais présenter il y a un enjeu majeur de renforcer notre capacité d'évaluation et d'objectivation du phénomène.-- C'est beaucoup, c'est bon. Monsieur le président. D'accord merci. Donc, la parole est à monsieur Antoine Lefèvre pour le groupe Les Républicains pour sept minutes, chers collègues. Madame la présidente. Monsieur le Ministre, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, la fraude est à l'impôt. Ce que l'ombre et à l'homme disait Georges Pompidou, une façon pour l'ancien président de la République de souligner l'étroite relation entre l'obligatoire contribution des citoyens aux charges publiques respectés par le plus grand nombre et la proportion d'individus qui choisira de s'y soumettre au cours de son existence. La fraude fiscale priverait chaque année l'état de 80 à 100 milliards d'euros de recettes, selon l'Insee. Des estimations approximatives impossible à déterminer précisément mais qui donne à elle seule le tournis. Elle représente en tout et pour tout près d'un quart des 450 milliards d'euros du budget voté en loi de finances pour 2023. Cette fraude porte gravement atteinte au principe de solidarité nationale et d'égalité devant la loi fiscale et les charges publiques qui figure en préambule de notre constitution, vous l'avez rappelé. Monsieur le Ministre ces préjudices pour notre société sont innombrables. Ils sont d'autant d'investissements manquer dans les politiques publiques de notre nation que de coups de couteau donné à notre contrat social. La redistribution pour nos concitoyens les plus défavorisés n'est pas pleinement opéré l'idée même de performance publique est affaibli la confiance qui doit régir les rapports entre les citoyens, les administrations se trouve durablement sapé c'est parce que notre société condamne avec la plus grande sévérité. Les faits de fraude fiscale que notre puissance publique s'est dotée au fil des décennies d'armes nouvelles pour la combattre. Le Conseil constitutionnel a fait le choix de l'ériger au rang d'objectif à valeur constitutionnelle par une décision du 29 décembre 1999. Le législateur pour sa part, à examiner puis adopté la loi du 23 octobre 2018, à examiner puis adopté la loi du 23 octobre 2018, relative à la lutte contre la fraude. Notre chambre, il y avait puissamment contribué en adoptant notamment commission à la fin du verrou de Bercy, ainsi que le renforcement de diverses sanctions pénales et administratives applicables. Notre commission des finances a souhaité ramener ce sujet au coeur des discussions, il y a un an en mettant sur pied en janvier 2022, une mission d'information relative à la lutte contre la fraude et d'évasion fiscale. Je remercie le président rénale ainsi que notre rapporteur général Jean-François Husson pour leur initiative extrêmement judicieuse ainsi que pour la grande qualité des travaux qu'ils ont rendu leurs conclusions font état d'un gain d'efficacité des instruments affectés au contrôle fiscal et ainsi d'une progression des montants recouvrés sur les 5 dernières années 10,6 milliards d'euros en 2021 contre 7 7, 3 années plutôt une hausse de 33, 38% des recouvrements face à laquelle il serait bien ingrats de bouder son plaisir et là ces montants demeurent encore bien loin de la réalité de ceux annuellement soustrait à l'État et aux collectivités. Il revient dès lors au législateur non seulement de poursuivre les efforts engagés dans cette direction, mais aussi et peut-être en 1er lieu d'interroger les motifs de persistance de cette fraude fiscale. Si l'on se fonde sur la pensée développée par l'économiste américain Richard mais en 1959, l'état d'un pourvoir 3 grandes fonctions constitutifs de sa puissance publique l'allocation des ressources, la redistribution des richesses et la régulation de l'activité économique. Partant de là, la volonté qui sous-tend l'infraction de fraude fiscale répond à une perte chez son auteur de la légitimité de cette mission et donc de son consentement en être un quelconque contributeurs futiles même marginale car en réalité, assurer le consentement des citoyens à l'impôt répond invariablement de sa juste et proportionnelle détermination par le Parlement. Demander plus à l'impôt et moins au contribuable disait Alphonse Allais, ah la belle époque un propos en substance repris par la théorie de la courbe de l'affaire qui Corel une une trop grande pression fiscale à une baisse de légitimité des prélèvements obligatoires et ainsi à un déclin des recettes publiques. Toutefois il me semble particulièrement important de le saluer, la répression de la fraude et l'évasion fiscale. Jouit en France de moyens autrement plus étendu que par le passé, la fin du monopole de l'administration fiscale sur les poursuites pénales a considérablement élargi les voies de recours du ministère public contre les auteurs d'infractions prévues par la loi de 2018, les dénonciations obligatoires au parquet de fraude fiscale supérieure à 100.000 euros, ont favorisé un rebond de 75% des dossiers transmis par l'administration en 2021, 1217 dossiers de fraude sur les 1620 recensés par la DGFIP était le fruit de cet assouplissement. Nos mettons pas non plus la fin d'une relative opacité des décisions de la commission des infractions fiscales qui n'étaient pas tenus avant 2018 de motiver ses avis en faveur de ou défaveur de poursuites. Une preuve concluante que la justice fiscale n'aurait su déroger plus longtemps à l'exigence de transparence qui régissent ses hommes et ses homologues pénal ou civil. Toutefois, il revient au législateur d'examiner encore davantage de pistes d'amélioration de notre politique en matière de lutte contre la fraude fiscale. Dans son rapport rendu en octobre 2022. Notre mission d'information a préconisé que soit estimé en loi de finances initiale, les montant approximatif de la fraude, vous les avez évoqué également Monsieur le Ministre, sur la base d'une méthodologie aussi précise que possible. Une ambition qui serait capable de donner une lisibilité nouvelles à l'action publique en matière de répression, voire même de faciliter une prise de conscience dans l'opinion publique de l'ordre de grandeur des sommes échappant à l'État et peut être même, soyons fous, de permettre un infléchissement des comportements des auteurs d'infractions. La lutte contre la fraude fiscale ne pourra jamais se vanter d'une pleine efficacité, donc des coûts continueront d'être portés au lien qui unit le citoyen, l'administration la légitimité de ce lien est une condition essentielle au retour du consentement à l'impôt. La suppression de la CVAE voté en loi de finances constitue un exemple de l'une de ces atteintes en ce qu'elle est appelée à étiolé à long terme le lien d'appartenance entre le territoire et ses acteurs économiques. Par ailleurs, si les récentes avancées ont permis de mettre fin à l'anomalie démocratique qui priver notre pays d'une police fiscale opérationnel. Les autorités en charge des poursuites judiciaires en matière fiscale manque toujours d'une plénitude de compétences, de leur service. Si le service d'enquêtes judiciaires des finances constituent bel et bien le bras armé de la répression des fraudes avec des effectifs doté des pouvoirs de police judiciaire. C'est 25 officier en poste ont une compétence qui reste cantonnée à certaines infractions fiscales seulement les privant ainsi de la plaine l'étude. Pardon de la même amplitude intervention que les officiers de police judiciaire. Regroupés sous une seule et même bannière les pouvoirs d'enquête et de poursuites sera une étape importante pour assurer la pleine performance et la police fiscale telle qu'elle est observée en Allemagne ou aux Pays-Bas. Peut-être pourrons-nous un jour tendre vers la constitution d'une véritable police fiscale et financière autonome française selon le modèle de la Guardia di financière italienne appelés à oeuvrer en binôme avec le parquet national financier. Enfin, il apparaît indispensable de renforcer la coopération entre les différents services de répression tant au niveau territorial entre l'aider Airship et les DD RDI qu'au niveau international avec les autorités de nos pays voisins. Le législateur est, on est conscient. La lutte contre la fraude a encore de beaux jours devant elle, charge à nous parlementaires de poursuivre ce combat et d'accroître la sensibilisation sur les préjudices de la fraude auprès du public. Je vois bien. Merci madame la présidente. Je veux remercier le sénateur Lefebvre pour son d'intervention et je crois vraiment comme vous. Que c'est un enjeu de pacte social que d'avoir une lutte efficace contre la fraude et je veux rappeler un point, c'est que à l'occasion de la loi de 2008 de 2018, pardon, sur la lutte contre la fraude. Fiscale et je vous remercie d'en avoir salué les effets. Ce qui a été rappelé qui me semble essentiel, c'est qu'il y a bien 2 jambes. La lutte contre la fraude d'un côté et la nouvelle relation de confiance entre l'administration fiscale et les particuliers, les entreprises notamment pour apporter de la sécurisation juridique aux entreprises pour moi les 2 doivent vraiment aller de Pair aller ensemble et je veux vraiment saluer tout le travail qui a été fait par la direction générale des finances publiques pour cette nouvelle relation de confiance qui porte vraiment ses fruits et on le voit, notamment chez les chefs d'entreprise il y a une il y a vraiment un changement qui a été perçu et c'est utile sur le verrou de Bercy comme vous je pense que la réforme est extrêmement positive, elle a permis une augmentation très forte des dossiers transmis à la justice. Je dirais simplement qu'on a aujourd'hui un enjeu, ça renvoie à l'intervention de madame Vermeillet à ce qu'on n'a eu comme débat sur le SGF dont il faut rendre en force et les moyens c'est l'enjeu de la priorisation. Il y a beaucoup de dossiers qui arrive aujourd'hui à la justice, il faut aider, accompagner les parquets pour prioriser les dossiers qui vont faire l'objet de véritables enquêtes judiciaires selon l'ampleur de la fraude estimée et donc c'est tout le débat et tout le travail qu'on va avoir sur le S. travail et une discussion qu'on a avec mon collègue Éric Dupond-Moretti pour être capable de mieux accompagner les parquets en la matière. Merci. La parole est à monsieur Pierre Jean Verzeaux laine pour le groupe les indépendants pour cinq minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. Déjà, comme les autres intervenants saluer l'initiative de la commission des finances qui nous propose d'aborder un sujet qui fait beaucoup parler qui est à l'origine de d'un certain nombre de fantasmes, mais qui est en tout cas un point très important du financement du budget de l'État. Et aussi de l'idée qu'on peut se faire de la justice devant l'impôt, notamment pour les contribuables qui eux respectent la loi et paye les impôts qu'ils doivent. Dans ce débat, vous me permettrez distinguer la fraude de l'évasion fiscale. La fraude, elle est condamnée par la loi puisqu'il s'agit de minimiser détourner, ne pas déclarer soustraire frauduleusement au paiement de l'impôt dit simplement il s'agit, par des moyens illégaux de ne pas payer l'impôt ou d'en payer une moindre pas. L'évasion fiscale elle. N'est pas définie par le droit. Elle consiste à utiliser des moyens à la limite de la légalité pour optimiser et payer le moins d'impôts possible. Autrement dit par des procédés licite, faire en sorte de faire disparaître l'impôt qu'on devrait payer en France au profit de contrer fiscal plus accueillante. Nous sommes ici dans une zone du juridique grise.-- Selon les chiffres alors comme dirait l'autre, on est chacun est venu avec nos chiffres puisqu'effectivement c'est. Par nature, chacun l'a dit très compliqué d'additionner des chiffres qu'on ne connaît pas. Même s'il y a des méthodes de calcul qui peuvent être qui peuvent être appliquées.-- Et vous l'avez dit tout à l'heure Monsieur le Ministre.

déjà hein, il faut arriver à le capter cet impôt et quand bien même nous prendrions les sommes que nous avons évoqués tout ça ne représente quelque fois que quelques pour 100. Des propositions économiques de certains candidats à l'élection présidentielle. Dis ça pour remettre. Le curseur où il doit être.-- Le débat sur l'imposition des plus riches et des grandes entreprises revient régulièrement dans le débat public et c'est tout à fait logique et je souhaite évoquer ce sujet parce que, évidemment, plus le niveau d'impôts sur les mêmes entre nous et nos voisins et les autres pays moyen de dumping, moins il y a l'envie d'évasion fiscale.-- Ce fut le cas dernièrement sur la loi de finances sur les superprofits. Il est tout à fait légitime de pouvoir réfléchir à avoir des impôts exceptionnel à des sur des années exceptionnelles. Le début du sujet. Déjà c'est l'impôt minimum et de faire en sorte que toutes les entreprises et notamment les grands groupes et recours au moins un impôt minimum et qu'on ne puisse pas optimisé jusqu'à ne payer quasiment rien. D'ailleurs sur ce sujet, nous pouvons noter l'action du gouvernement. Menée depuis quelques années auprès de nos partenaires européens et puis au sein de l'OCDE pour avoir un impôt minimum de 15% qui devraient normalement 2023 être mis en oeuvre dans 138 juridiction ayant accepté cet accord, Monsieur le Ministre, si vous pouvez nous confirmer que ces choses avancent et qu'elles vont se mettre en place dans les, dans les mois qui viennent. Et ce que je viens d'évoquer ici nous sommes dans un cadre où il y a des états qui vont autour d'une table et qu'on avec lesquels on peut discuter et puis à les pays qui ne participe à ces discussions et là c'est le sujet de l'évasion fiscale. Et les paradis fiscaux qu'on se comprenne bien évidemment s'il y a pas de paradis fiscal. Il y a pas d'évasion fiscale et donc le le le le le le le point important du sujet il est là. Ça fait plusieurs fois qu'on essaie de le réformer, ça a été dit depuis 2009 et de la crise de la crise et les résultats sont loin d'être à la hauteur de ce que nous aurions pu attendre. Évidemment ce sont des pays indépendants qui on ne peut pas donner d'ordres. Néanmoins, il peut y avoir une volonté politique internationale et coordonnée pour les faire avancer et ça a été dit tout à l'heure par une collègue. Je crois qu'il y a beaucoup à faire sur le plan bancaire. j'ai travaillé en banque je me souviens d'époque où il y avait l'embargo sur l'Iran. Les virements émis de France vers l'Iran ou vers les pays plateforme c'est-à-dire ceux vers qui ont transit des fois il y avait un nombre de documents à réunir qui est extrêmement important. Les sommes étaient bloqués plusieurs semaines entre les deux. Et à la même époque pour que des virements partent dans les paradis fiscaux, c'était beaucoup plus simple et beaucoup plus souple. Malgré les déclarations Tracfin. Donc je pense qu'il y a en tout cas de ce côté-là, pas mal de choses qui peuvent qui peuvent avancer. Donc Monsieur le Ministre, quelles sont les mesures coordonnées coercitives à l'échelle internationale pour lutter contre l'opacité des paradis fiscaux.-- Merci, cher collègue, Monsieur le Ministre. en la matière et croyez bien qu'il y a une solidarité absolue sur ce sujet-là, je veux revenir puisqu'il faut choisir en 2 minutes sur ce que vous avez évoquées, c'est-à-dire le pilier de l'imposition minimale pour les grandes entreprises et je veux saluer vraiment le progrès majeurs que ce que je veux rappeler l'historique. On nous a dit couac, le président de la République a porter ce sujet là, allô. D E en 2022 1021 qu'on n'arriverait pas à obtenir un accord à l'OCDE on a obtenu en octobre 2021, un accord à l'OCDE, avec 140 États pour la mise en oeuvre de cette imposition minimale. Ensuite on nous a dit il y aura pas d'accord au niveau européen pour le transcrire dans le droit européen et c'est vrai qu'il y avait certains pays notamment la Hongrie pour ne pas la citer, qui bloquaient qui utiliser leur droit de véto tant et si bien qu'en septembre 2022 à l'initiative de la France. 5 ou 6 pays mémoire il y avait l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas ont signé une motion une déclaration indiquant que si l'Union européenne ne transcrivent est pas dans son droit. Le pilier de ces pays, notamment la France qui était l'initiative appliquerait le pilier de quand bien même ça n'était pas transcrit dans le droit européen, ça contribue à faire bouger au niveau européen et donc il y a eu cet accord historique le 16 décembre du Conseil Ecofine et c'est vraiment un progrès majeur, c'est un progrès majeur parce que ça permet de lutter contre l'optimisation fiscale qui scandalise évidemment les Français. Une PME une petite PME, elle a pas la possibilité de minorer sur son impôt sur les sociétés en délocalisant une partie de ses profits dans des pays qui permettent une imposition moindre. C'est une vraie inégalité entre les entreprises et je le dis aussi, je suis ministre du Budget, évidemment. C'est aussi des rentrées fiscales supplémentaires pour financer nos politiques publiques donc vraiment il faut saluer cette avancée importante et la faire connaître aussi parce que je pense que les Français qui régulièrement sont scandalisés par des affaires qui émerge, c'est aussi important de leur montrer qu'quand les choses avancent donc, merci monsieur le sénateur.

Madame la présidente. Monsieur le Ministre, chers collègues. Tout d'abord comme chacun avant moi je tiens à saluer les travaux de la mission d'information. Sous l'impulsion de Jean-François Husson et et Claude Raynal relative à la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale et à vous remercier pour ce débat en séance publique. Le groupe écologiste a voté les conclusions c'est pas si souvent que notre groupe vote l'ensemble des des des des textes. Parce qu'il répond aux enjeux de civisme de dissuasion et de répression indispensable mais pour cela il faut évidemment en 1er lieu une véritable volonté politique. Le gouvernement veut-il se donner les moyens de lutter plus vigoureusement contre la fraude et l'évasion fiscale. La réponse est sans doute un peu dans le fameux en même temps jupitérien. Il y a des avancées majeures. Il n'en reste pas moins parfois des ambiguïtés idéologiques et des mesures analyser peut-être pour ne pas trop effrayer les milliardaires où les champions du CAC 40. Une attitude dure avec les fraudes des pauvres et parfois plus conciliante au nom de l'efficacité, vous l'avez justifié Monsieur le Ministre de la durée des procédures avec la fraude des multinationales ou des plus riches. C'est un sujet difficile, car la marge est étroite entre la fraude et l'évasion fiscale et elle nourrit effectivement des populismes. Dans ces marches nourrice et grandissent les populismes. Je pense à certains sujets qui m'interroge comme le choix de l'opacité. Lorsque le président Macron défendait en 2021 la clause de sauvegarde qui empêche la publication d'informations indispensables pour lutter contre l'évasion fiscale ou encore vous venez d'en parler, lorsque Joe Biden propose une imposition minimale à hauteur de 21% des 7 ou 8000 plus grandes entreprises du monde et que la France se range dans un 1er temps, plutôt du côté de l'Irlande qui n'était pas parmi les plus allant à la en la matière en décembre, l'Europe est parvenu à un accord adopté un impôt minimum global de 15%. C'est une victoire. Vous venez de le souligner et nous ne la boudons pas mais ce n'est pas assez car pour nous, il reste injuste et même inacceptable de moins taxer des multinationales que des TPE-PME dans ces écarts nourrit un sentiment d'injustice. Il est indispensable d'amplifier les actions contre l'opacification des flux financiers mis en lumière également par Pandora Papers Panama Papers makes false ou d'autres, il est indispensable de doubler comme le préconise le rapport de la mission, le nombre d'officiers fiscaux judiciaires et de leur donner les moyens de traiter la fraude à la TVA. Au passage, chacun des postes créés génèrent des recettes bien supérieurs aux coûts salariaux et monte l'intérêt du service public ne nous en privons pas là où il y a volonté d'agir. Il y a des résultats. Pendant les derniers buts débat budgétaire. Vous n'aviez Monsieur le Ministre eu de cesse de répéter, combien ça coûte, un instant combien ça perd de ne pas pouvoir mieux lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. La fraude à la TVA est estimé à deux à 20 à 25 milliards par an selon l'Insee, qui montre également que les pertes de recettes globales dues au non respect des droits fiscaux seraient de or, de 80 à 100 milliards au niveau européen. On évalue à plus de 7900 milliards d'avoir cachés dans des places Offshore échappant à l'impôt des pays d'origine, c'est près de 10 fois le montant du plan de relance européen et c'est vertigineux. N'est-ce pas la conséquence d'une attitude qui répétant sans cesse qu'il y a trop d'impôts, finit par se dire que l'impôt n'est pas une ardente nécessité de l'optimisation fiscale à la fraude fiscale la marche peut être parfois ténue et cela génère en tous les cas, cette évasion fiscale une délinquance qui se pense au-dessus des lois, au-dessus des droits et au dessus du pacte républicain et du contrat social ces fraudeurs diminue des recettes publiques et les capacités de l'État a vilain des politiques publiques ambitieuses indispensables au quotidien des. Des Français ou la transition écologique si nécessaire ou tout simplement à équilibrer les comptes publics. Monsieur le Ministre Lemaire nous a assuré qu'il serait intraitable avec ceux qui ont triché. Tant mieux car les personnalités mises en cause par les Pandora Papers, sont des gens de pouvoir ancien dirigeant élu famille royale et autres milliardaires avec une armée de juristes il maîtrise les doit s'en exonère et profite de l'opacité du système financier international. Il est donc urgent au niveau national de renforcer encore plus les moyens de l'administration fiscale au niveau européen d'étendre la liste des paradis fiscaux. En intégrant tous les pays impliqués dans les Pandora Papers. Le travail de la commission des finances, est un point d'appui utile et le gouvernement gagnerait ou plutôt gagnera à l'intégrer pleinement je veux dire vive aussi le journalisme d'investigation, la presse libre et les lanceurs d'alerte. Voilà. Monsieur le Ministre. Merci madame la présidente. Moi je veux rejoindre le sénateur brouillé. Quand il dit qu'il faut lutter contre toutes les fraudes. Qu'il ne faut pas être. Fort avec les faibles et faible avec les forts toutes les fraudes doivent être poursuivis et doivent être sanctionnés et recouvrer et je vous donner un chiffre qui est pour moi un chiffre important sur l'ensemble des montants de fraude recouvrée par la DGFIP chaque année. 40% des montants recouvrés sont issus des enquêtes de la DV Annie que j'ai cité tout à l'heure pour l'affaire McDonald's. Qui concerne cette cellule a DVA ni cette direction. Les entreprises, les très grandes entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 400 millions d'euros. Donc on voit à quel point. La, enfin la part importante des très grandes entreprises, dans les montants qui sont recouvrés par la DGFIP chaque année en l'occurrence 40% et puis bon encore une fois je. Je je je je je ne veux pas qu'on oppose une fraude à une autre toutes les fraudes doivent être combattus, je le disais c'est vrai que parfois dans le débat politique, on peut avoir le sentiment que certains considèrent qu'il y aurait que la fraude fiscale, d'autres qui aura que la fraude sociale parfois dans une logique de stigmatisation, moi c'est pas du tout mon souhait, mon souhait c'est qu'on lutte contre toutes les fraudes fiscales, sociales douanières sans stigmatisation sans instrumentalisation mais juste avec à coeur de renforcer notre cohésion et le pacte social puisque les Français je crois attendent de nous que nous luttions contre toutes les formes de fraude. Merci. La parole est à monsieur Didier Rambaud. Pour le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants pour six minutes, chers collègues. Madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. La fraude fiscale consiste à effectivement à échapper ou tenter d'échapper à l'impôt par tout moyen, c'est le détournement illégal d'un système fiscal, un peu plus de 4 ans après l'adoption de la loi du 28 octobre 2018, relative à la lutte contre la fraude. Je crois que nous pouvons affirmer que depuis 2017, notre pays a considérablement progressé en la matière. D'abord avec la réforme de ce que l'on désigne comme étant le le verrou de Bercy antérieurement, seule habilitée à initier les poursuites en cas d'infraction de fraude fiscale. L'administration fiscale est désormais tenu d'informer le procureur de la République qui dit qui décide seule de l'opportunité de poursuites pénales. Dans le cas où le montant des droits fraudés est au moins égale à 100.000 euros de plus, la coopération entre les services de Bercy et de la justice a été renforcée par exemple les dossiers de personnalités enregistré à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique peuvent être transmis au parquet sous certaines conditions, lorsque le montant des droits fraudés est au moins égal à 50.000 euros. Par ailleurs les agents de l'administration fiscale ne sont plus tenus au secret à l'égard du parquet, même pour des dossiers ne faisant pas l'objet d'une transmission. Une telle réforme permet aujourd'hui de constater qu'une action conjointe moderne et efficace entre les services de la justice et de Bercy est L'occasion de saluer le travail réalisé par les femmes et les hommes de ses services. De nouveaux outils ont également été voté en matière de de lutte contre la fraude sociale. À l'image de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et de la convention judiciaire d'intérêt public. Rappelons également que la liste des paradis fiscaux dressée par l'Union européenne a été transposée en droit français à l'échelle internationale, l'extension du projet BEPS sous l'égide de l'OCDE la 15ème et dernière action du projet consistait en l'élaboration d'une convention multilatérale outils juridiques. Innovant qui permet de gagner du temps, puisqu'elle permet d'aménager automatiquement l'ensemble des conventions liant les États, autrement dit la convention multilatérale ne se substitue pas aux conventions bilatérales mais elle les modifie une fois encore la France a été pionnière dans la mise en oeuvre de cette convention grâce à l'impulsion de la majorité présidentielle. Force est de constater que, en matière de lutte contre la fraude sociale et l'évasion fiscale, les gouvernements sociaux-Cif depuis 2017, agissent en 2020 le monsieur Ministre de confirmera l'État a récupéré près de 7 8 milliards d'euros grâce au contrôle de lutte contre la fraude fiscale. Raison pour laquelle la mission d'information conduite. Par monsieur le président de la commission des finances et Monsieur le le rapporteur général ne conclut pas à la nécessité d'une révolution fiscale mais plutôt à à un certain nombre d'ajustements et d'évolution. Une telle conclusion permet donc d'attester qu'il existe à ce à ce jour des dispositifs efficaces pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. Est-ce pour autant suffisant bien dit évidemment que non paradise Paper Panama Papers le clic Autant d'exemples qui démontrent qu'en matière de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale des progrès peuvent indéniablement être réalisé. À ce titre, certaines recommandations du rapport d'information semble. Pertinente à commencer par l'augmentation du nombre d'officiers fiscaux judiciaires pour les doubler à horizon de 5 ans. Le Service d'enquêtes judiciaires des finances, ne dispose que de aujourd'hui que de 40 officiers fiscaux judiciaires alors qu'il a été saisi de 169 affaire de fraude fiscale et de blanchiment de fraude fiscale. Pour ce qui est de la fraude à la TVA, on le sait tous, c'est un gisement important de ressources budgétaires sujet complexe du pourrions envisager de, de permettre aux agents des douanes de sanctionner directement ce type de fraude dans le cadre du dédouanement à l'importation par la création d'un délit douanier spécifique dans le code des douanes. Enfin parce que les montages fiscaux complexes. Sont réalisés en tenant compte des différents juridique d'un pays à l'autre, les solutions les plus efficaces exige une à une échelle internationale. Pourquoi ne pas envisager, à juste titre une réflexion sur la création d'un dispositif de n'même. Envers les pays qui ne jouent pas le jeu de la coopération en matière d'échange d'informations en complément des listes européennes. La complexité de la fiscalité internationale exige en effet des efforts concertés concertés pour avancer notamment à l'échelle européenne, c'est bien en ce sens que la France doit continuer d'être moteur et force de proposition comme elle sait l'être depuis 2017 avec pour objectif de renforcer la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Je vous remercie. Merci, monsieur le Ministre. majeurs de la loi de 2018 sur la lutte contre. La fraude, il y a un avant et un après en terme d'outils en terme de moyens et je crois en terme de résultats. Je veux aussi. Saluer. Le fait d'avoir mentionné. L'enjeu essentiel de communication et de partenariat entre les services fiscaux et le monde économique, les entreprises je donnerai un chiffre 20.000 rescrit chaque année qui sont transmis par l'administration fiscale aux entreprises. Avec dans l'écrasante majorité d'entre eux, un délai de transmission aux entreprises de moins de trois mois. Et aujourd'hui un taux de satisfaction des entreprises sur leur relation leur confiance dans les services. Partenariaux dès la DGFIP à 95% donc c'est extrêmement positif. Je pense qu'il faut le saluer. Vous avez salué vous avez rappelé les outils nouveaux qui ont été permis par la loi de 2018 il y en a notamment dans le numérique. Il y en a un qu'on cite souvent et qu'on a cité dans les débats sur le PLF qui le web strapping. Et sur ce sujet-là je proposerai notamment à. à. Un groupe de travail avec les parlementaires d'analyser les résultats dont on dispose, liées à l'expérimentation. Avant de statuer sur une généralisation, il y a beaucoup de d'efforts et beaucoup de progrès qui ont été réalisées par les outils numériques dans la suite à la réforme de 2018, il y a un certain qui sont passés par des expérimentations. Je pense que maintenant il faut se poser la question. De savoir lesquels. Est-ce qu'on généralise. Et je sais, Monsieur le Sénateur Rambo que vous serez au rendez-vous pour y aller travailler avec nous. Merci. La parole est à Monsieur Victorin Lurel pour le groupe socialiste, écologiste et républicain pour quatre minutes, chers collègues. La là. La là. La présidente. Monsieur le Ministre.-- Monsieur le président de la commission. Monsieur le rapporteur général, chers collègues. Je souhaite au au nom de mon groupe remercier la Commission son président Claude Raynal. Et son rapporteur Jean-François. Les membres de cette mission d'information de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale pour le travail technique d'évaluation qui a été conduit. Je considère ainsi que les préconisations émises peuvent utilement. Aider les législateurs que nous sommes à faire évoluer d'apporter l'efficacité des dispositifs de lutte contre la fraude. En la matière je crois que la prudence ne doit pas entraver notre ambition. Car au-delà des milliards d'euros de recettes récupérés par l'État, la lutte efficace. Contre l'évasion et la fraude fiscale constitue un enjeu fondamental de justice sociale. Un défi administratif et financier qui recouvre de faire des enjeux éthiques, politiques et démocratiques. Je rejoins parfaitement. L'ensemble des recommandations. Faites dans ce rapport et singulièrement celles relatives aux moyens techniques et budgétaires nécessaires pour mieux chiffrer et mieux appréhender l'ampleur de la fraude. Au-delà de la complexité des montages des schémas de dissimulation, il reste incompréhensible qu'en 2023 nos services de parviennent toujours pas à savoir si le contrôle fiscal parvient recouvrer pour 110% mais % voire plus des montants fraudés. Il est vrai depuis 20 ans la DGFIP. Et l'administration qui connaît les plus importantes baisses d'effectifs. Je l'affirme donc bien que relativement efficace et un collègue a évoqué les ambiguïtés idéologiques et philosophiques. Bien que. Efficace ni le Data Mining ni les nouveaux outils de ciblage ne remplaceront parfaitement à mes yeux le travail d'un enquêteur. au-delà, je souhaiterais aussi profiter de cette tribune pour adresser à l'Assemblée. Moi mon point d'alerte à travers les évolutions législatives récentes en matière de contrôle fiscal. Je crains. En effet, que nous n'encourageons une dérive de la philosophie même du contrôle. Une dérive consiste à avoir des comportements de fraude pénalement répréhensible requalifie aurait apprécié en tant que simple erreur ou optimisation pouvant vont faire l'objet de transactions d'argent de gré à gré et parfois dans l'opacité changeant la nature même de ce contrôle, je pense cela naturellement au recours aux convention judiciaire d'intérêt public pour les personnes morales et aux comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour les personnes privées certes le développement d'une logique préventive est louable mais faire aujourd'hui. Si j'ose dire l'absolution des fraudeurs me paraît une voie glissante et donc dangereuse. C'est la raison pour laquelle je reste particulièrement réservé quant à l'usage croissant au CGIP. Qui permettent aux grandes entreprises d'échapper à une condamnation pénale. Initialement réservé aux faits de corruption. La CIJ ont été étendu aux faits de fraude fiscale et le blanchiment de fraude fiscale en 2018 100. Par ailleurs, et contrairement aux CRPC que les condamnations de soit inscrite au casier judiciaire si je reconnais volontiers que cela permet des rentrées puis. Directe de recettes fiscales et d'éviter. De longs procédure judiciaire. Je dois avouer que la relative impunité pénale accordée à ces entreprises fraudeuses continue de me poser problème dès lors que les justifications apportées à l'utilisation de la CGIP école pour la plupart, de manque de moyens des différentes institutions concernées. Je crois donc de bonne politique de renforcer les moyens humains et matériels de la justice et de simplifier les procédures de la justice et des services. En conclusion, je souhaite une nouvelle fois remercier notre président et notre rapporteur général pour la richesse des conclusions de cette mission et souhaite ardemment. Qu'elle inspire le gouvernement pour l'amélioration de notre arsenal législatif et qu'elles nourrissent les propositions de notre autre assemblée. Je veux remettre. Merci, monsieur le Ministre. Merci madame présidente. Monsieur le ministre, Lurel. Je crois que l'enjeu de la réforme de 2018, il faut le rappeler. C'est précisément d'avoir davantage de dossiers qui sont transmis à la justice. J'ai entendu dans votre intervention, cette crainte que certains dossiers de fraude qui le justifieraient ne soit pas examinée regardé par la justice. Le fait d'avoir fait sauter le verrou de Bercy c'est ça vise précisément à transmettre, davantage de dossiers à la justice et d'être capable de distinguer aussi les fraudes d'un montant important, les fraudes à enjeu pour être il y a pas véritablement les sanctionner et les distinguer d'erreurs qui ne serait pas de la fraude mais je suis d'accord avec vous, il faut bien examiner que l'enquête soit vraiment exhaustive sur ce sujet-là et je vais revenir sur les outils dont on a parlé plusieurs fois à l'initiative du sénateur bouquet ou d'autres. Et notamment sur la CGIP sur la CGIP. La convention judiciaire d'intérêt public. Moi je veux rappeler que c'est homologué par le juge. Et d'ailleurs ces conventions, elles sont largement négocié par le PNF et ensuite le juge doit les valider, donc y compris sur ces outils qui permettent ce n'est pas qu'on avait tout à l'heure de recouvrer beaucoup plus tôt et de manière surtout certaines un montant, ils sont évidemment. Examiner et valider in fine et par l'autorité judiciaire. Merci. La parole est à monsieur Michel un évêque pour le groupe Union centriste, c'est pour 4 minutes. Madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Ben le groupe de l'Union centriste et particulièrement heureux du travail qui a été réalisé par. La commission La commission des finances, autour du président Claude rénal et du rapporteur général Jean-François Husson, concernant la lutte contre l'évasion et la fraude fiscale parce que ce sont des préoccupations que l'on défend en permanence dans le travail que l'on réalise ici il y a eu notamment lors de différentes sessions des amendements déposés par notre collègue Nathalie Goulet à ce sujet qui est très persévérante mon collègue Alain Dufour également est très attentif. À tout cela. Et donc le groupe de l'Union centriste et particulièrement à à ce que les valeurs d'équité et de transparence puisse effectivement être mise en oeuvre ici alors. Le montant de la fraude fiscale a été évaluée récemment Monsieur le Ministre par l'Insee en décembre dernier, de l'ordre de 80 milliards, dont un quart. Concernant la faute fiscal à la TVA. Alors je vais pas revenir sur la fraude fiscale à la TVA puisque. Notre collègue Sylvie Vermeillet là largement évoquée tout à l'heure. je vous rends attentif au fait que le commerce en ligne et le commerce à distance se développe considérablement dans notre pays et qu'il faut être vigilant à cet égard, nous sommes en particulier, allez avec de la commission des finances à Roissy. Voir comment travailler les douaniers nous nous sommes aperçus à cet égard qu'il leur fallait à la fois des moyens humains et des moyens techniques permettant de mieux appréhender. La nature des colis qui arrivaient par exemple pour éviter qu'il y ait de la fraude et et que. Finalement il d'évasion fiscale et c'est vrai que à un moment où les prix accuse préoccupations budgétaires dans notre pays sont fortes. Il est important que nous trouvions tous les outils permettant à la fois de renflouer les finances publiques. C'est le cas notamment par. Un effort accru sur la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale et aussi que nous soyons attentifs à ce que. Nous ne devions pas recourir autant que possible au à l'endettement. Alors. La commission des finances, monsieur le ministre a dans ce rapport présenté une vingtaine de recommandations. Elles ont été largement évoqués par. Les orateurs précédents. Néanmoins. En plus de la TVA. Je crois qu'il faut que l'anchois attentif à la question d'une part. Des. Montages financiers complexes. A très savamment évoquer tout cela ça demande une coopération qui soit accrue avec. Les. Je dirais les autorités. Douanières où les autorités. Financières des autres pays, notamment européens pour que nous puissions. Lutter efficacement contre cette évasion fiscale en quelque sorte et faire en sorte que. Tout le monde revienne dans le dans le droit chemin. Un autre sujet. Auquel il faut que nous soyons à tenter j'Monsieur le Ministre. C'est la question de la connaissance des bénéficiaires effectifs des sociétés.

à cette question des bénéficiaires effectifs des sociétés. Donc. Il paraît anormal que cela intervienne et il paraît logique que l'UNPI réintègre. Pour tout le monde la possibilité de pouvoir consulter les bénéficiaires effectifs des sociétés de façon à ce que nous puissions. Avoir une meilleure connaissance de tout cela et puis. Cela a été dit aussi dans le rapport, la question de la renégociation des conventions internationales de coopération. Je crois qu'il faut pas avoir de tabous là-dessus. Il faut qu'on puisse le faire. Merci de votre attention. Merci cher collègue. Monsieur le Ministre. j'allais dire en plein essor. Ça fait maintenant plusieurs années, mais dans le chiffre d'affaires a dépassé les 130 milliards d'euros et donc on voit l'enjeu absolue là a bien garantir qu'on est capable de recouvrer les montants dus notamment en matière de TVA. Il y a d'ores et déjà des législations qui ont été. Adoptées je pense. Évidemment ou paquet TVA commerce électronique qui a été mise en oeuvre à partir de juillet 2021 et la vraie innovation. Le vrai changement, c'est qu'il rompt les plateformes redevable de la TVA certaines activités de vente à distance, on voit que c'est un outil utile puisque je peux donner un chiffre. Entre juillet 2021 et décembre 2021 donc au tout début de la mise en oeuvre de ce paquet TVA commerce électronique à travers le guichet unique qui permet à ces plateformes de verser de manière simple à l'État, à la TVA qu'elles doivent on a recouvré 700 millions d'euros sur ses premiers mois. Donc on voit que c'est utile, il faut évidemment continuer à aller plus loin, il y a des discussions et des négociations au niveau européen qui se tiennent en ce moment pour garantir le bon encadrement fiscal de ces plateformes. particulièrement attaché à cela, nous voyons bien que pour ce qui concerne la lutte contre la fausse les résultats s'améliorent, nous arrivons à recouvrer. Plus de de ressources là dessus mais il faut continuer à intensifier l'effort et en particulier, comme je l'ai dit tout à l'heure par des moyens humains obtenus par redéploiement sur le contrôle, j'ai eu l'occasion de dialoguer avec le service inter-régionale qui s'occupe du contrôle en Bretagne et de constater qu'il travaillait particulièrement efficacement. Je crois qu'il faut continuer comme cela et qu'ils puissent disposer d'un certain nombre d'outils leur permettant. Parle de timing notamment de, de mieux appréhender les risques de fraude.-- Merci la parole est à monsieur Stéphane Le Rudulier. Pour le groupe Les Républicains pour sept minutes, chers collègues.

madame la présidente sur le le ministre, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général. La lutte contre la la fraude fiscale revient régulièrement dans dans le débat national et et pour cause, vous l'avez. Largement rappelé en introduction de de vos propos. Frauder, c'est un peut refuser d'apporter une contribution due au au financement des politiques publiques et à la solidarité nationale, c'est aussi le le consentement à l'impôt On peut légitimement s'interroger sur le le manque à gagner. Pour l'État, ça a été dit plusieurs estimations on évoque. Parfois le chiffre de 200 milliards de de de fraude fiscale c'est un chiffre qui tourne. En boucle qui a été. Notamment avancé régulièrement par le le syndicat. Finances publiques. Solidaires Finances Publiques. C'est un chiffre qui permettrait, sans nul doute d'amoindrir considérablement. Notre déficit structurel chronique si ont récupéré cet cet argent sur. Sous le tapis Voilà. Personne n'est en réalité capable de mesurer précisément cette fraude fiscale et et ce chiffre est tout de même sujet à forte caution car c'est 100 milliards évoqués ne concerne pas exclusivement la Ford fiscal au au sens juridique du terme mais correspond à une extrapolation à partir de l'ensemble des manquements fiscaux, c'est-à-dire que clairement c'est 100 milliards inclut les erreurs, les divergences d'appréciation entre l'administration fiscale et le contribuable ainsi que l'évasion fiscale et ou encore l'optimisation fiscale abusive. D'autres évaluations comme. Celle du Conseil des prélèvements obligatoires. Nous indique. Qu'on serait plus vraisemblablement en réalité autour de 30 à 40 milliards de vraies fraude fiscale entre guillemets au sens juridique du terme. Ce qui a déjà quand même considérable. Étant donné que les services fiscaux n'en détecte que 5. À 10% et étonnamment et ça a été souligné malgré l'arsenal législatif et technologiques qui s'est renforcé ces dernières années, on a parlé. De l'allégement ou en tout cas du desserrement du du de, des roues de de Bercy. On a également évoqué la facture électronique pour la mise en oeuvre en 2024 qui va sans doute largement contribué. À l'amoindrissement de la fraude. À la TVA. Les résultats annuels malgré ses efforts sur les droits et pénalités une mise en en recouvrement et encaissé franchissent péniblement la barre des 10 milliards d'euros en 2021. Preuve de l'efficacité toute relative de la seule coercition. La France est le pays de l'OCDE où les prélèvements obligatoires sont les plus élevés. C'est un élément essentiel et peut être trop souvent minorée dans nos débats dans l'explication. De la fraude. Fiscale. On se réfère. Et ça a été dit à la courbe. De l'affaire un accroissement des taux d'imposition se traduit au-delà d'un certain seuil par un un monde richement de recettes fiscales. Trop d'impôt tue l'impôt. Un pays attractif et dynamique économiquement retient ses talents et ne les fait pas fuir faire revenir des exilés politiques dans un pays d'origine, revient à garantir un cadre et un changement de cadre politique pour garantir leur sécurité. Il en est de même sur l'existe fiscale sans changement de cadre fiscal, il n'y aura pas de retour possible. Il faut savoir qu'on est dans un, dans une économie mondialisée, dans un monde interconnecté, maintenir des prélèvements obligatoires record en se révoltant à juste titre contre la fraude et surtout l'évasion fiscale se peut se révéler être une une utopie. Dangereuse ainsi. Si on se réfère notamment aux États-Unis. On fait une étude comparative 2004 2005 sous l'administration Bush, l'année où les mesures de réduction d'impôts sont entrées en vigueur les recettes fiscales du gouvernement ont augmenté de 8 et de 9%. La hausse s'est poursuivie l'année suivante avec 10% au 1er semestre, alors que la croissance de l'économie a elle été de 3,9% par an. Il en est de même au Royaume-Uni la tranche marginale de l'impôt sur le revenu passa sous Margaret Thatcher de 83 à 60% puis 40%, ce 40%, ce qui entraînera simultanément une hausse des recettes fiscales de plus d'un milliard. De livres entre 85 et 86. Ainsi, je vous l'ai dit si nous voulons faire reculer la fraude fiscale et augmenter les recettes fiscales au-delà des mesures qui ont été prises. Alors il va falloir baisser les impôts, bien que cela puisse paraître intuitivement paradoxal car je reste convaincu qu'on peut débattre de tous les moyens normatif de tous les carcans de toutes les armes possibles, la seule et la meilleure solution de façon de réduire la fraude fiscale, c'est avant tout de baisser massivement les impôts, les charges, il y en a pas d'autre encore une fois la fraude fiscale est évidemment hé bien sûr condamnable doit. Être le combat de chaque instant parce qu'elle est le refus de l'obéissance à une loi de la République a une loi démocratique mais nous ne pouvons en aucun cas la défendre ici. Force est de constater tout de même que la fraude fiscale résulte essentiellement ou. Peut être. et pour conclure j'aimerais citer Churchill qui disait ceci par rapport à l'impôt. Une nation qui essaie de prospérer par l'impôt et comme un homme dans un seau qui essaie de se soulever par la poignée c'est peine perdue alors changeons de logiciel et osons la liberté. Je vous remercie.-- Merci beaucoup. La parole est à monsieur le Ministre.-- Merci madame la présidente, monsieur le sénateur Le Rudulier. Je vous rejoins sur. La nécessaire le nécessaire allégement de la pression fiscale sur. Les particuliers sur les entreprises, c'est la politique qu'on mène depuis 2017. C'est un débat, on se fait parfois critiqué sur le sujet mais notamment la réforme de l'ISF, la suppression de l'ISF la flat tax. On a vu immédiatement des résultats avec un nombre de retour en France de personnes. Assujettis à l'IFI, en l'occurrence désormais supérieur au nombre de départs. Pour la première fois quand on a supprimé l'ISF. On a vu davantage de ses contribuables revenir en France que partir et ça ne s'est, je ne crois pas démenti Donc on voit bien l'enjeu qu'il y a à garantir. À à une attractivité aussi pour notre pays, sur ce sujet-là, ça vaut aussi pour les entreprises. c'est notamment pour ça que nous avons tenu, y compris dans la dernière lecture du PLF à réintroduire la suppression de la CVAE. Pour les entreprises qui avait été rejetée par le Sénat, parce que c'est important que cette logique on la suive aussi pour nos entreprises et pour l'industrie. Mais pour les finances publiques. C'est aussi plus de recettes à la fin si vous baissez les impôts mais vous avez plus de contribuables qui sont assujettis en volume. Vous avez davantage, c'est ce qu'on a vu sur les entreprises, par exemple on collecte plus d'impôt sur les sociétés depuis que le taux est à 25% qu'à l'époque où le taux était à 33% parce que ça permet aussi le développement de l'économie en revanche. Je ne pense pas et ça n'est pas ce que vous avez souhaité faire je crois que on puisse entre guillemets excusez des fraudes, parce qu'il y aurait des impôts trop élevés. Heureusement, nous avons un conseil constitutionnel et lorsqu'un drapeau est considéré comme confiscatoire évidemment il est censuré mais je vous rejoins sur la nécessaire. Diminution de la pression fiscale dans notre pays, c'est ce que nous continuons à faire on reste le 2ème pays en matière de pression fiscale, c'est aussi pour ça qu'on s'est opposé avec Bruno Lemaire a des propositions de créances création d'impôts, même temporaire, et dès lors que les finances publiques le permettront évidemment poursuivra cette.

le la le le rapport de la mission d'information qui a été remis en témoigne, il est une très grande qualité et il s'inscrit vraiment dans la logique et dans et dans la politique qui est la nôtre. On va tacher, notamment pour les mesures qui n'ont pu passer. Le Conseil constitutionnel dans le PLF d'en appliquer les mesures et moi je le redis je vraiment construire cette feuille de route sur la lutte contre les fraudes fiscales, sociales douanières dans les prochains mois avec les parlementaires. Je proposerai d'ailleurs aux présidents des groupes de l'ensemble des groupes des deux chambres de désigner un représentant pour travailler avec le gouvernement au contenu de cette feuille de route pour poursuit la logique que nous avons initiée dans le cadre des dialogues de Bercy qui nous ont permis de travailler tous ensemble et je vois le rapporteur général d'ores et déjà se réjouir que nous puissions ré-impulser ce dialogue tous ensemble. Je vous remercie à nouveau pour la participation à ce débat et je me tiens à votre disposition à celle de la commission de la mission. D'information de l'ancienne usine Merci, monsieur le Ministre, alors pour conclure, le débat n'a pas volé maintenant à monsieur Claude Raynal, président de la commission des finances pour cinq minutes. Merci. Merci madame la présidente, monsieur le le Ministre, mes chers collègues sera Avatar général. Ce débat a été. De de bonne tenue, je voulais évidemment remercier chacun et chacune d'entre vous. vous. Juste un peu dérapé. À la fin là sur. La question de la baisse de l'impôt. Mais bon marginal par rapport à l'ensemble des interventions que que nous avons eu. Ce soir. Je voudrais pas évidemment je avais pas prétendre à faire une synthèse de tout ce qui a été dit. Chacun. Fait son miel de ce qu'il a pu entendre, mais je voudrais de remarquer. L'intérêt qu'a eu ce rapport cette mission qui a été souhaité par la Commission et vous remercier et remercier certains. De nos collègues non membres de la commission d'avoir également participé à ce débat et d'avoir donné. Leur avis sur les sujets qui ressortait de nos échanges. quelques quelques points et principaux axes. Qui peuvent être rappelés. Mais c'était il y allait très vite. Premier axe. C'est le sujet de l'évaluation de la fraude fiscale et des zones de risque dans ce dans ce domaine. Exercice délicat. Et qui ne sera d'ailleurs de certaines matières jamais totalement abouti. Car les techniques de fraudes au fur et à mesure et vous lit. Mais connaître l'ampleur des sommes qui sont soustraites à l'impôt est indispensable évidemment en termes d'équité fiscale en tout cas d'avoir une une approche la plus la plus fine possible. Le gouvernement bien sûr doit mettre des moyens pour réaliser davantage d'études sur ce sujet. Pour sa part, la commission des finances est engagé depuis plusieurs années sur le sujet de la lutte contre la fraude à la TVA avec des mesures concrètes qui ont été adoptés notamment sur la responsabilité solidaire des plateformes en ligne pour le paiement de la TVA au départ c'était pas aussi évident que ça. De convaincre sur ce point, on a vu que ça a produit des effets, il faut aller encore plus loin, toujours dans ce domaine en développant les partage d'informations entre les administrations publiques en matière de déclaration de TVA. Un 2ème axe ce soir qui a été mis en lumière pour les travaux de la mission également d'informations et pour lequel nous attendons une implication du gouvernement parce que tous ne n'est pas. Évidemment ne passe pas par le législatif et l'approfondissement et la fluidification de la coopération entre l'administration fiscale et l'autorité judiciaire, elle est bien meilleure qu'elle n'a qu'elle n'a été mais il y a encore des progrès à faire. Depuis la réforme du verrou de Bercy, davantage de dossiers de fraude fiscale sont traitées par la justice. Or la question de la fraude fiscale par elles-mêmes. N'est toujours pas et ne peut pas d'ailleurs mais le sujet central. Peu de notre justice. Il faut quand même. Évidemment donner une impulsion. Mais aussi une formation des magistrats et des moyens dédiés pour que ce sujet prenne toute sa place tellement le sujet. Vous l'avez tous dit est extrêmement technique. Par ailleurs. Il y a évidemment des des critiques sur les instruments de justice négocier comme le convention judiciaire d'intérêt public et les comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et il me semble qu'il faut surtout déployé tous les moyens possibles pour permettre de faire revenir dans les caisses de l'État, les sommes qui lui sont dus sans bien sûr mettre de côté la responsabilité pénale. Des fraudeurs lorsqu'il est avéré. Un 3ème axe me soumettre les enjeux de coopération européenne et internationale. La fraude peut démarrer par les logiciels de caisse non-certifiée chez les petits commerçants mais la plus difficile à combattre. Et celle impliquant des mouvements transfrontaliers des internes, des intermédiaires financiers spécialisés dans ce type de montage, quand ce ne sont pas des États qui se spécialise même dans ce domaine. Il existe donc des circuits extraordinairement sophistiquée pour éluder l'impôt par le biais de montages offshores. Nous avons vu le sujet particulièrement complexe. Elle a été rappelé, et semble-t-il peu résolu dès que makes. Un important effort doit être réalisée pour lutter contre ces montages et faire rentrer dans le rang, les États qui ne coopèrent pas. En matière d'échange d'informations fiscales. Enfin, nous devons être attentifs à la conciliation entre le respect des libertés individuelles et la lutte contre la fraude. Sans tomber dans l'excès de protection des fraudeurs. Les libertés individuelles ne saurait être brandie pour échapper au contrôle fiscal. L'accès à des données librement accessibles sur les réseaux sociaux et donc celles qui ont publiquement accessibles au sens de la jurisprudence du Conseil constitutionnel permettrait des avancées concrètes. Enfin, soyez sûr. Évidemment, Monsieur le Ministre, que notre commission des finances restera mobilisée. Sur ce sujet important tant que ces questions de fraude ou d'évasion fiscale. Sont. Elles importantes insupportable en réalité et vous l'avez tous dit. À juste titre pour nos concitoyens, nous espérons que le gouvernement saura entendre les propositions du Sénat et trouver des moyens d'aller toujours plus loin sur ce sujet, je vous remercie. Merci président. Alors je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 21h 30 pour le débat sur la politique du logement dans les outre-mer. La séance est suspendue. Merci